La séance est reprise lors du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances adoptées par l'Assemblée nationale pour 2018 nous poursuivons l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances des différentes commissions : le Sénat va examiner les crédits de la mission santé.

rapporte. Merci Monsieur le Président, Madame la ministre Madame la rapporteure, mes chers collègues, cette mission santé au fond est une petite mission milliard au regard des 200 milliards qui sont pris en charge par l'assurance maladie, il y a toutefois à l'intérieur de cette mission, l'Inde médicale d'État, c'est d'ailleurs essentiellement le seul point je vais aborder dans ce propos liminaire, une aide médicale d'État, la ministre qui n'en finit pas n'augmenter et on a l'impression qu'il n'y a que pour la M1, qu'il n'y a pas de limite que dans dans la, dans cette même mission pour les les organismes de santé publique on rabote tout rond où on restreint et pour la MEC 882 millions d'euros qui sont demandés ces 110 millions en plus et c'est 50 pourcent de plus entre 2012 et 2016 2 en 2000 en 2012, on a vu qu'à cette période de 2011, 2012 1013 il y a une certaine stabilité et là il y a vraiment une augmentation exponentielle, il faut vraiment qu'on en parle, madame la ministre, c'est un un vrai sujet et pas question de comme on a pu tenter faire d'autres années de de supprimer l'article en question mais vraiment le Sénat vous appelle la commission des finances vous appellent à une refonte de cette année, meurt, nous aurons l'occasion tout à l'heure de présenter un nom de la commission qui réduit les crédits pour les ramener à à ce qu'ils étaient en 2012, pas question de supprimer de de renoncer à cette mission d'accueil de, de, de la France, mais quand même d'essayer de regarder au fond comment on pourrait trouver une solution tout en accueillant en mettant comme certaines limites, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, ça sera le sujet donc essentiel, s'agissant de la commission des finances, dont nous reparlerons tout à l'heure, voilà et je ne veux pas être plus long pour laisser un peu de temps à notre collègue rapporteur de la commission des affaires sociales, merci. Merci, monsieur le rapporteur, donc la parole est à présent Madame Corinne Imbert, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Pour 3 minutes Madame la rapporte. Monsieur le Président, Madame la Ministre, monsieur le rapporteur, mais chers collègues dans le temps imparti aux commissions, saisie pour avis, je m'en tiendrais aux 3 principales observations formulées par la commission des affaires sociales sur la mission santé du projet de loi de finances pour 2018, il ne faut tout d'abord souligné que l'instabilité qui caractérise le programme 204 constitue un sujet d'inquiétude majeure depuis plusieurs exercices des dépenses de plus en plus nombreuses sont en effet transféré à la sécurité sociale, le projet de loi de finances pour 2018 n'y déroge pas puisque l'assurance maladie, se voit confier le financement de 2 nouveaux opérateurs sanitaires de l'État, l'Agence de biomédecine et l'école Des hautes études en santé publique qui disparaissent ainsi du programme de santé, nous pouvons entendre l'objectif d'une visibilité accrue avancé par le gouvernement, mais cette évolution ne doit conduire ni un désengagement de l'État, il y a un contrôle plus difficile pour le Parlement, elle pose en tout état de cause, la question de la cohérence du programme 204 pour les années à venir. En ce qui concerne les objectifs d'économie aux opérateurs sanitaires, la commission souhaite alerter sur la situation de l'Agence nationale de santé publique, l'importance prise par les urgences sanitaires ne doit pas remettre en cause sa capacité à s'investir pleinement dans sa mission de prévention et de promotion de la santé, d'autant plus que les crédits relatifs aux actions de prévention ne sont plus sanctuarisé depuis la suppression, l'année dernière de la dotation de l'assurance maladie s'agissant du programme 183 nous revele vont l'effort de sincérité du gouvernement quant aux prévisions de dépenses être médicale d'État à la fameuse AMM, les mesures mises en place pour assurer une plus grande maîtrise du dispositif nous paraissent également constituer un motif de satisfaction outre l'introduction d'un contrôle ciblé sur 10 pourcent des dossiers à l'instruction de l'ensemble des demandes d'aimer en métropole, sera l'année prochaine, centralisés auprès des 3 tests les plus concernés, cette démarche nous paraît aller dans le bon sens et dans le sens d'une harmonisation d'une plus grande sécurité des procédures, elle devrait également permettre une diminution des coûts de gestion, il semble en août que la demande des Caisses d'accéder aux informations détenues par le ministère de l'Intérieur, s'agissant des titres de séjour était enfin entendu, nous nous en félicitons, car il y a 2 ans, notre commission avait déjà déposé un amendement en ce sens lors de l'examen du projet de loi de finances, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur, rapporteur, mes chers collègues, sous réserve de l'ensemble de ses observations, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission santé du projet de loi de finances pour 2018, je vous remercie. Merci madame la rapporteure dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque discussion qu'on prend le temps d'intervention général et celui de l'explication de vote par ailleurs le gouvernement dispose au total de 10 minutes pour intervenir, la parole est à madame Véronique Guillotin, pour le groupe RDSE et pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre Mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, alors que l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale n'est pas encore achevé, nous voici réunis pour débattre aujourd'hui des crédits alloués en 2018 à la mission santé du projet de loi de finances, comprenant les programmes de 104 et 183 le budget total s'élève pour l'an prochain à 1,4 milliards d'euros, il connaît ainsi une hausse de plus de 10 pourcent par rapport au budget 2017. Cette hausse supérieur aux années précédentes, pourrait être saluée si bénéficier ainsi à toutes les actions du programme, ce qui n'est pas le cas, je formerai certaines remarques concernant notamment la prévention en effet dans le programme de 104 intitulé prévention sécurité sanitaire, organisation de l'offre de soins, les actions relatives à la prévention connaissent toutes une baisse de leur crédit. Pour avoir suivi de manière assidue débat du PLFSS je connaît l'attachement de madame la ministre des solidarités, de la santé à ce sujet. Si l'état de santé de la population française s'améliore, ce n'est pas le moment de relâcher nos efforts, les chiffres sortis ces derniers jours sur les contaminations HIV au sein de la population, ex-homosexuel, nous le rappelle le poids des décès prématurés évitables, des maladies chroniques, restent toujours en France, très élevé, plus de 30000 décès par an sont évitables par la prévention et la simple modification des comportements aussi je souhaiterais avoir des éclaircissements sur la baisse des 5 millions d'euros de crédit prévention engagée par l'État, cette baisse n'est-elle pas en n'est-elle pas contradictoire avec la révolution de la prévention que vous avez annoncée comme un axe central de la nouvelle stratégie nationale de santé, la réduction des moyens ne va-t-elle pas mettre à mal la mise en oeuvre d'une politique de santé que l'on veut tous efficaces. fonde enfin ce fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne rêvez ne revêt plus qu'un caractère très subsidiaire par rapport au financement de la branche AT-MP concernant la haine en 2016, les dépenses totales de l'État et de l'assurance maladie tout type d'Aime confondus, se sont élevés à 863 millions d'euros, en hausse de 6 pourcent par rapport à 2015, les crédits en 2018 seront à nouveau augmentées de 108 millions d'euros afin de répondre à une hausse tendancielle des bénéficiaires estimé à 5,3 pourcent par an, bien que l'on ait enregistré une discrète régression en 2017, le dispositif AME ne semble plus être remis en cause et c'est une très bonne chose en effet c'est un dispositif utile, je dirais même indispensable à la fois pour des questions de sécurité sanitaire collective et pour des raisons humaines le respect du droit de chacun à bénéficier d'un minimum de ces soins nous soutenons donc toutefois la hausse de ce poste risque encore de s'accentuer dans les années à venir, des efforts de maîtrise que nous saluons, ont déjà été engagées, notamment en matière de contrôle et de lutte contre la fraude, toutefois l'évolution prévisible des dépenses mériterait que soit ouvert un débat en profondeur pragmatique apaisée et surtout loin de toute posture idéologique dans le seul objectif de maintenir un équilibre global des programmes de cette mission santé mais avant tout, c'est bien la reprise de l'emploi et la bonne santé de nos entreprises qui permettront à notre système de soins tout entier de mieux se porter, en résumé, la hausse du budget de la mission santé du PLF s'explique essentiellement par l'augmentation des crédits alloués au dispositif d'indemnisation des victimes de la dépakine à hauteur de 77 millions

et ses conséquences, résultat de fusions et regroupements successifs des opérateurs sanitaires parmi les 4 opérateurs restant la NSM la NSP qui voient leurs subventions augmenter tandis que Lens et l'INCa au contraire les voient diminuer pour l'INCa la baisse significative de 5 pourcent est un mauvais signal Kant le cancer touche 380 4000 nouveaux patients par an et que 150000 patients en décèdent chaque année parallèlement nos indicateurs de dépistage organisé du cancer colorectal et du cancer du sein sont bien loin des objectifs à atteindre, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous donner des explications sur cette baisse des crédits à l'Alain et peut-être nous rassurer sur ses capacités à réaliser sa mission avec des moyens réduits pour conclure, je voudrais rappeler que nous avons salué votre projet de santé du PLFSS qui va dans le bon sens, mais le budget de cette mission santé suscite de la part de notre groupe, des interrogations, j'aurais attendu une cohérence plus grande entre les objectifs ambitieux affichés en matière de prévention et leur traduction concrète sur le budget du programme 200 IV la prévention apparaissant trop souvent comme une variable d'ajustement d'un budget dont certains postes ne sont pas maîtrisés, nous serons attentifs aux débats à votre capacité à répondre à nos interrogations et, le cas échéant à nous rassurer, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent Monsieur Michel Amiel pour le groupe, la République en marche et pour 6 minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur pour avis Madame, rapporteur spécial, mes chers collègues, alors que nous venons de finir l'étude du projet de loi de financement de la Sécurité sociale et que la question du financement de notre système de protection est au coeur des débats, nous nous retrouvons aujourd'hui pour voter les crédits de la mission santé au sein du PLR. Pour l'année qui vient, ses crédits s'élève à un virgule 4 milliards d'euros pour les 2 programmes qui constituent cette mission. Cette progression de près de 14 pourcent et soyons très clair, une bonne nouvelle. Cela peut paraître paradoxal dans des temps où nous devons construire des Budgets raisonnables ou l'Ondam votée dans le PLFSS pourrait être même qualifié de rigoureux mais ses programmes sont essentiels dans notre politique de santé. Je commencerais par parler du programme 183 dit protection maladie qui contient le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est un grand sujet de crispation quoi ne peut moins. Qui constituent l'aide médicale d'État. La grande majorité de ce programme en effet près de 99 pourcent concernent l'AME, dispositif qui permet l'accès aux soins aux personnes résidant de manière irrégulière en France depuis au moins 3 mois selon un système de prise en charge quelque peu similaire à celui de la CMU. Il n'est pas la peine, je pense, de rappeler le devoir mais aussi la nécessité de soigner ces personnes dans le besoin, que ce soit de Mfoa ne sanitaire, humanitaire, mais aussi d'un point de vue de santé publique, en effet, en plus de prévenir le développement des maladies infectieuses, le traitement de pathologies un stade précoce et bénéfique pour tout notre système et permet d'éviter de lourdes prises en charge en cas de maladie plus avancé plus grave et finalement bien plus coûteuse pour la collectivité. Alors ce soir on peut de ce texte, le budget effectivement vous l'avait rappelé Monsieur Joyandet est en hausse par rapport à 2012. Il avait été disons-le clairement sous-évalué. Dans un objectif de sincérité et en tenant compte de l'augmentation constatée des bénéficiaires de cette aide ces dernières années, ainsi que des crises migratoires auxquels nous devons forcément faire face, je salue la responsabilité de cette prévision et diminuer cette enveloppe comme vous le suggérez, me semble-t-il, dans le cadre de l'amendement que vous avez évoqué tout à l'heure, aurait à nouveau me semble-t-il, le budget d'insincérité donc voient bien qu'il y a à la fois une dimension sanitaire qui nous conviennent pas, véritablement, mais aussi une dimension purement financières, puisque si ces Budgets ont été réévalués, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était tout simplement pour les faire davantage coller à la réalité financière. Concernant le Fiva je tiens ici à saluer l'engagement de l'État qui maintient ses crédits, venons-en à l'autre programme d'admission senti le de 200 prévention sécurité sanitaire et offre de soins. Ce programme dont les objectifs de prévention des risques sanitaires et d'amélioration générale de santé, notamment en matière d'égalité d'offre de soins sur l'ensemble du territoire sont claires et bien lui aussi se confronter à une rationalisation des moyens alloués. La récente création de l'Agence nationale de santé publique, via la fusion de certaines agences le transfert de l'Agence de biomédecine de l'École de hautes études en santé publique à l'assurance maladie ensemble des indicateurs importants de ce désir de simplification et de rationalisation. donc qui est au coeur de notre mécanisme de prévention et de maîtrise de crise sanitaire et a pu montrer tout son intérêt encore récemment dans les événements climatiques qui ont frappé et nous outre-mer. Ce budget est aussi à la hauteur de ce que j'appelle de mes voeux, à savoir une véritable politique du médicament via le financement de l'Agence nationale de sécurité publique, par exemple, le les objectifs de maintien du délai de traitement des AMM, les autorisations de mise sur le marché dans dans ce sens avec un objectif de stabilisation autour de 150 jours. Le budget de la mission hausse ne saurait masquer la recherche d'une optimisation maximale de la gestion de la prévention en France, aussi bien dans son organisation que dans son financement, qui apparaît en voie d'achèvement. Vous me permettrez de m'arrêter une seconde sur le sujet qui me tient à coeur, c'est celui la santé mentale, et en particulier des jeunes, ce programme est essentielle dans la mise en place d'expérimentation pour le repérage la souffrance psychique des jeunes : la mise en place d'outils à disposition des professionnels etc. Toujours sur ce programme, je m'arrêterai un instant pour nous vous va le foie sur un élément de sincérité de cette augmentation, le montant prévu pour prise en charge des dommages imputables à la dépakine via l'Office national d'indemnisation des victimes de la il apparaît que cette provision devrait répondre de manière pertinente aux premières Haendel nisation qui devrait voir le jour au début 2018. Tous ces éléments, mes chers collègues nous auraient amenés mon groupe et moi, a voté pour, pour ces crédits sensible, sincère, je répète efficient oeuvrant dans le sens de plus de solidarité et d'équité finances, enfin de l'amendement déposé par la commission des finances ne peut, à l'instar de celui de Madame Ménard, à l'Assemblée nationale, même si les intentions ne sont certes pas les mêmes ampute le budget de l'AME ici discuter de 300 millions d'euros, dans ces conditions, le groupe la République en marche et ne pourra pas voter en faveur d'un texte si l'été remanié, tels que la commission des finances le souhaite, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à madame Laurence Cohen du groupe CRC et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la discussion du budget de la mission santé de ce projet de loi de finances doit être menée en lien avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, que nous examinerons en seconde lecture demain aussi, ne faut-il pas perdre de vue les 4,2 milliards de restrictions budgétaires sur les dépenses d'assurance maladie qui sont programmées, vous avez présenté le budget de la mission santé, Madame la Ministre, comme un budget de responsabilité certes la mission affiche une hausse de crédit de 14 pourcent avec notamment une hausse de 10 pourcent des crédits du programme 204 prévention sécurité sanitaire et offre de soins et une augmentation de plus de 13 pourcent des crédits du programme 183 protection maladie mais derrière ces effets d'annonce, il y a une autre réalité qui consiste à une diminution des crédits de certaines actions une réduction supplémentaire des effectifs, la hausse de 10 pourcent des crédits du programme 204 relative à la prévention à la sécurité sanitaire et à l'offre de soins survient après une baisse de 6 pourcent en 2017 par rapport à 2016 et en poussant l'analyse, on s'aperçoit que cette hausse des crédits est bien à l'enveloppe de 77,7 millions d'euros supplémentaires prévus pour les victimes de la dépakine, ce qui est notoirement en-deçà des bouées on s'aperçoit également que l'ensemble des autres missions ont des moyens en baisse ainsi les crédits de l'action santé des populations diminue de moitié et ceux de l'action prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades se réduisent de 4 millions d'euros, tandis que les subventions des opérateurs baissent de 6 pourcent à l'heure où les inégalités d'accès aux soins vont croissantes, où il est essentiel de développer la prévention, nous ne pouvons soutenir de tels choix ces baisses successives qui peuvent apparaître comme une volonté de bien gérer l'argent public entraîne des renoncements extrêmement grave en effet comment dans ces conditions, lutter contre les maladies chroniques qui sont en forte augmentation et que dire de la prévention des addictions, autre sujet d'inquiétude : le sort réservé aux agences sanitaires depuis plusieurs années, elles subissent de plein fouet les réductions drastiques imposées au secteur de la santé ce PLF ne fait pas exception avec une réduction de 2 5 pourcent du plafond d'emplois, la suppression de 57 équivalents temps plein travaillés et une diminution de 5 des crédits de fonctionnement, soit une baisse de 6,5 millions d'euros demander toujours plus aux agences sanitaires avec moins de moyens financiers et humains n'est pas de nature à leur permettent de remplir leur mission de santé publique, outre les réductions de crédits à la santé des populations à la prévention des maladies chroniques et à la qualité de vie des malades, le programme de 104 voix également diminuer les crédits consacrés à la prévention des risques liés à l'environnement et à la l'alimentation respective ment de 7 et de 6 pourcent comment justifier de telles baisses alors que l'on connaît les risques accrus en en la matière, pollution des des eaux de l'air perturbateurs endocriniens, venons-en au crédit du programme 183 protection maladie destiné essentiellement à l'aide médicale d'État, qui affiche une hausse de près de 13 pourcent en 2018 ayant entendu dans cet hémicycle des contrevérités à ce sujet lors de l'examen du PLFSS permettez-moi de rappeler quelques faits avérés, le nombre de bénéficiaires de l'AME de droit commun, a diminué de 1,6 pourcent par rapport à 2015, l'augmentation de ces crédits est due uniquement au dynamisme des dépenses de médicaments et dispositifs médicaux qui représente 117 millions d'euros, les migrants représentent 0,2 pourcent de nos dépenses de santé, selon l'Observatoire de non-recours aux droits seulement 57 pourcent des étrangers ont recours aux prestations auxquelles ils ont droit de plus dans son rapport de 2014 sur le non-recours aux droits, le défenseur des droits, dénonce le fait que les bénéficiaires de l'AME font l'objet de refus de soins de manière récurrente à ceux qui critiquent la générosité de notre système de santé et voudrait tourner le dos à la dignité humaine, en pointant du doigt les plus fragiles, je veux répondent solennellement avec l'ensemble des membres de mon groupe, que c'est l'honneur de notre pays que d'avoir un de tels dispositifs, permettez moi de terminer mon propos sur la dotation de 8 millions d'euros de l'État au financement de fondation d'indemnisation des victimes de l'amiante Fiva pour 2018 cette dotation correspond à 3 pourcent de la contribution de la branche AT-MP, ce qui est largement insuffisant, ces 2 programmes sont dans le droit fil du PLFSS que nous regrettons dans la philosophie reste dans la réduction des dépenses publiques pour le groupe CRC les dépenses de santé doivent avant tout répondre aux besoins des patients en tenant compte des formidables progrès scientifiques et technologiques qui ont été réalisées transiger sur la prévention, le dépistage, ou encore la qualité de vie des patients n'est pas acceptable des moyens financiers existent dans ce pays pour y répondre, ce qui manque, avec le gouvernement, Philippe Macron comme avec ceux qui l'ont précédé, c'est la volonté politique de mobiliser ces nouveaux financements pour toutes ces raisons, nous voterons contre la mission santé du PLF 2018, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent Madame Élisabeth Doineau, du groupe Union centriste et pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la ministre, madame, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sortons de l'examen du 1er projet de loi de financement de la Sécurité sociale du gouvernement avec des satisfactions Madame la ministre, mais aussi quelques oppositions les discussions sur la mission santé du projet de loi de finances se dérouleront sensiblement dans le même esprit, pour le groupe Union centriste aujourd'hui si nos débats portent sur des montants financiers sans commune mesure avec ce discutés au cours du PLFSS il n'en demeure pas moins que le programme 214 relatif à la prévention à la sécurité sanitaire et à l'offre de soin et le programme 183 relatif à la protection maladie continue de jouer un rôle important en matière de santé publique. Malgré une enveloppe restreinte, les moyens consacrés à la mission santé augmente de manière significative, plus 12 pourcent pour 2018, dépassant ainsi les un milliard 4 d'euros en autorisation d'engagement cette hausse globale marque des situations contrastées au sein de chacun des programmes, le programme de 104 qui représentent le tiers des dépenses de la mission voit son périmètre d'action évoluer au gré des projets de loi de finances, le nombre d'acteurs, financé par l'État ne cesse de diminuer, soit du fait de transfert vers l'assurance-maladie, soit par fusion des établissements ainsi ce sont l'Agence de biomédecine et l'école Des hautes études en santé publique, qui opère la bascule cette année, attention à ne pas déséquilibrer durablement cette mission, le nombre d'opérateurs sanitaires est divisé par 2 en un an, notamment grâce à la création de l'Agence nationale de santé publique, la NSP, par fusion de 3 établissements, ce travail de simplification était attendue et semble opérant, je m'en réjouis, grand tation des crédits du programme, en charge de la prévention est une bonne nouvelle, 4 ans après sa dernière hausse mais elle doit être relativisé puisqu'elles visent essentiellement à financer le dispositif d'indemnisation des dommages imputables à la dépakine Madame la Ministre de la Santé milite pour passer de la logique de parcours de soins à celle de parcours de santé je partage pleinement cette analyse : nous devons quitter le tout curatif et investir massivement dans la prévention aussi je m'inquiète que ces crédits ne soient plus sanctuarisé la NSP doit s'imposer comme un acteur clé en ce domaine. Enfin, il y a 2 enjeux : dénoncer la réduction dangereuse du fonds de roulement de l'Agence nationale de sécurité du médicament, alors que dans le même temps, elle montait en compétences, je salue donc la décision d'augmenter les crédits versés à l'ANSM j'en viens maintenant au programme 183 protection maladie dont 99 pourcent des crédits sont consommés par l'aide médicale d'État, je vous remercie d'avoir rappelé et cet effet aussi par mon collègue Michel Amiel, d'avoir rappelé avec force que la haine est une nécessité humanitaire, d'abord parce que quel médecin peut refuser de soigner un patient quel qu'il soit une nécessité sanitaire pour éviter que les affections contagieuses ne s'étende, une nécessité enfin économique car plus d'une maladie et traiter précocement et moins elles coûte à la société haine est nécessaire oui, doit-on s'interdire de discuter de son fonctionnement et de son financement non la dépense d'homme a en effet progressé irrémédiablement de 40 pourcent entre 2009 et 2016 et ces crédits ont fait l'objet d'une sous-évaluation systématique sous le précédent quinquennat il convient donc de parvenir à maîtriser enfin les crédits de ce programme à court terme, l'engagement de sincérité du gouvernement en augmentant signifiait significativement le budget de la AME pour 2018 plus 13 pourcent donc à saluer à moyen terme, j'invite le gouvernement et mes collègues parlementaires dans un 1er temps à se saisir du rapport d'information sur l'accès financier aux soins des personnes en situation de précarité voté au cours de ce PLFSS pour y intégrer une étude approfondie de la M et dans un second temps, à remettre à plat la politique d'aide médicale d'État via une réforme débattue à sa juste mesure au Parlement, c'est le souhait de notre rapporteur spécial ne se Monsieur Joyandet qui propose également une réduction des crédits de l'de 300 millions d'euros sur ce dernier point, les analyses diffère au sein du groupe centriste, c'est un peu notre habitude, pour autant, la plupart sont pour s'abstenir sur cette proposition, pour ma part, j'estime que l'emploi de la menace budgétaire semble à ce stade disproportionnée, chers collègues, je ne pense pas que la fin justifie les moyens et c'est donc par un vote négatif que je me positionne sur cette proposition d'amendement en tout état de cause, il est à souligner l'effort certains sur les contrôles et je pense qu'il faut les intensifier son taux est nettement supérieure à d'autres dispositifs et la centralisation des caisses harmonie sera et garantira une meilleure maîtrise des dépenses, enfin le programme 183 n'apporte que 8 millions d'euros sur les 270 millions du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, cette participation, malheureusement, d'autant plus faible au regard de la responsabilité de l'État dans le dossier de l'amiante et je tiens à insister à insister sur cet élément comme je voulais indiquer, en introduction, Madame la ministre, les orientations que vous avez emprunté sont source de satisfaction pour le groupe Union centriste, malgré quelques déceptions qu'il conviendrait de corriger aussi les sénateurs centristes voteront sous ces réserves en faveur des crédits de la mission santé. Merci, cher collègue là. Parole est à monsieur Bernard Genier pour le groupe socialiste et républicain et pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la ministre Madame la rapporteur monsieur rapporteur, mes chers collègues, on ne peut pas entrer dans l'étude de cette mission de santé du PLF sans la remettent en perspective car le périmètre de cette mission, ça a été dit, a fortement évolué au cours de ces dernières années, successivement la Haute autorité de santé, l'Agence de traitement de l'information hospitalière les finir l'Agence de biomédecine maintenant et l'école et aux études en santé publique, ont été transférés à l'assurance maladie et donc la question est posée d'entrée de la cohérence du périmètre du programme de 104 qui devient bien difficile à percevoir, c'est ainsi le cas de la du pilotage de la politique de de santé publique, dont la hausse apparente dans le document budgétaire est en fait celle des frais de justice, et en particulier du dispositif d'indemnisation des victimes du valproate de sodium, le mouvement de fusion des agences qui a été menée par la précédente ministre de la Santé a permis la création d'un opérateur essentiel, Agence nationale de santé publique, mais encore faut-il que les moyens soient à la hauteur de ses nombreuses et essentielle mission j'y reviendrai, on ne peut qu'être également surpris que la plus importante baisse des crédits concerne 2 actions pourtant inscrit dans les objectifs de la stratégie nationale de santé, les actions auprès des publics les plus vulnérables au moins 47 pourcent et les actions en santé environnementale, moins 5,6 il faut aussi souligner qu'il ne reste plus que 110000 euros pour financer, je cite, les actions pour sensibiliser, former, mobiliser, informer, informer le grand public et les professionnels de santé aux violences faites aux femmes et à la lutte contre les mutilations sexuelles, ce n'est manifeste pendant pas dans ce budget que votre collègue, Madame Schiappa a obtenu les moyens transversaux dont elle nous a fait part ici même il y a 2 jours dans le ce cas d'budgétaire, c'est plutôt le rabot la faiblesse et la baisse des moyens consacrés à la santé environnementale et donc également un sujet de préoccupation, les facteurs d'Exposition qui sont déclinés dans le bleu santé du 3ème Plan national santé environnement sont correctement correctement décliner la surveillance aérobiologique oui bien sûr, l'amiante, le bruit, le saturnisme et le CO, oui, mais où sont la pollution de l'air, responsable de 40000 morts par an, où sont les polluants chimiques de l'environnement intérieur et de l'alimentation, où sont les perturbateurs endocriniens ou longe crucial de l'Exposition, inut Ayrault, au sujet duquel la recherche a considérablement progressé et appelle maintenant une politique nationale forte de protection de l'enfant à naître et du nourrisson, les progrès pour la santé humaine dans les décennies à venir viendront en grande partie d'une meilleure maîtrise des facteurs environnementaux qui dégradent notre santé et nous sommes là au coeur de la prévention qui est justement mise en avant par la ministre de la Santé, il est vrai, de nombreux acteurs ne sont pas dans le Champ sanitaire, l'urbanisme, l'alimentation, les transports, le logement, son 1er rang mais parce que la ministre de la Santé porte cette thématique essentielle : elle a la légitimité, la responsabilité d'impulser de produire l'expertise nécessaire et l'évaluation, elle doit en avoir les moyens, à la veille de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, quelques mots sur ce virus, la victoire est possible, les épidémiologistes convergent pour le dire et ONU-Sida le confirme qu'il a lancé une stratégie mondiale pour éradiquer le VIH en 2030, avec des indicateurs intermédiaire en 2020, ce serait, je pense, une première dans l'histoire de la médecine, arriver à vaincre un virus sans avoir de vaccins, quelle émotion, ce serait pour les chercheurs et pour nos 2 prix Nobel français, quelle émotion, ce serait pour les personnes serrées ou positive pour les associations qui luttent depuis tant d'années pour celles et ceux qui ont été victimes, directement ou indirectement de l'épidémie, cette perspective d'éradication, elle doit nous rassembler, il ne faut pas tarder à compléter les mesures prises pas mal Marisol Touraine sur la presse sur les auto-tests et intensifier le dépistage dans les populations clés les HSH les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres sommes les migrants, les travailleuses du sexe, les personnes transgenres, c'est la clé du succès, malheureusement, j'allais dire le niveau de l'épidémie est trop faible pour entraîner une mobilisation suffisante de la société et il est trop élevé pour qu'elle s'éteigne avec encore 6000 contaminations par an, nous avons donc un défi commun à relever et les élus que nous sommes, nous avons là une belle responsabilité celle d'entraîner notre société dans un dernier et fructueuse fort, enfin, je ne voudrais pas terminer mon propos sur le programme de 104 100 redire quelques mots de l'Agence nationale de santé publique L à encore, en émergence, mais cette émergence et prometteuse ces principes fondateurs sont bons, une approche de la prévention intégrée qui concernent l'ensemble des politiques publiques et valorise les échelons locaux un continuum entre l'épidémiologie et la prévention, une gouvernance ouverte à la fois scientifique également participative et citoyenne, il faut prendre garde à ce que des ressources trop peu diversifiée, une réduction du plafond d'emplois, une articulation encore insuffisante avec les autres acteurs dont les ARS fragilise une agence qui doit devenir une grande agence de référence en santé publique, j'en viens pour terminer au programme 183 et à l'aide médicale État. Tous ceux qui analyse ce régime avec les lunettes de la santé publique et de parcours de soin arrivent efficient arrivent à la même conclusion : il faut intégrer le dispositif au sein de l'assurance maladie, c'est l'analyse de l'Inspection générale des affaires sociales depuis plusieurs années et c'est celle de l'Académie de médecine depuis quelques mois. Tous ceux qui regardent ce régime avec les lunettes de l'efficience économique, je voudrais vous le soulignez Monsieur le rapporteur de la commission des finances, arrivent à la même conclusion et retiennent les économies d'échelle que produirait cette intégration, c'est l'avis de l'Inspection générale des finances, et puis il y a ceux qui regardent la même avec les lunettes de leur position sur la politique migratoire et qui, selon leur opinion veulent soit le maintenir et les tendre soit le supprimer ou le coupent en morceaux sans qu'on comprenne bien d'ailleurs que le fondement sanitaire des coûts qui sont proposées. Moi je vous dis qu'il est temps d'agir de façon rationnelle, avec une connaissance précise des éléments concernant tant la santé les parcours de soins, les données économiques de l'AME et les conséquences sur ces 2 plans, d'une éventuelle intégration du dispositif dans l'assurance maladie, c'est pourquoi j'ai déposé un amendement demandant au gouvernement de mener ce travail d'expertise et de nous permettre de ne pas en rester au statu quo actuel, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Joël Guerriau. Du groupe, les indépendants pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre. Mais, chers collègues, vous savez, une grande partie des crédits du système de sécurité sociale, ont déjà été votées à l'occasion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale mais cette mission n'en est pas pour autant moins importante, elle vise tout au contraire, à poursuivre les efforts engagés au cours de ces dernières semaines avec une trajectoire vers un équilibre des finances de la Sécurité sociale à l'horizon 2020, cette mission porte malheureusement en elle les germes de véritables problèmes financiers du fait d'une sous-budgétisation chronique de certaines dépenses, il est donc nécessaire de remettre à plat ses dépenses et d'envisager un apurement de ses comptes, il est urgent d'accorder une âme, une attention scrupuleuse à l'examen de ces crédits, cette mission a aujourd'hui une triple vocation premièrement elle encadre les moyens consacrés à la prévention à la sécurité sanitaire et à l'offre de soins, deuxièmement, prévoit les crédits accordés à certaines agences sanitaires et troisièmement à la bonde le financement de l'aide médicale d'État en augmentation chronique depuis 2009 pourcent au cours de 8 dernières années avec un budget courant de 923,7 millions d'euros, les crédits de cette mission sont en augmentation de 12 pourcent par rapport au ouvert en 2017 avec une dotation actuelle de 1,4 milliards d'euros à l'heure d'une réduction des dépenses publiques, cette hausse des dépenses sociales et tout à fait préoccupante et mérite que notre assemblée se penche avec attention sur l'utilisation des deniers publics au sein du programme 204 consacré aux dépenses de prévention, l'évolution à la hausse des crédits ce speak par une volonté de doter financièrement un nouvel acteur chargé de centraliser l'ensemble des opérateurs encadrés par cette mission. En effet, l'Agence nationale de santé publique agira désormais comme Opéra. De référence, réduisant le nombre d'établissements subventionnés par cette mission de 8 à 4 opérateurs le groupe les indépendants République était. Voir salue cette mesure de simplification. Mais s'étonne que rationalisation ne rime pas avec réduction des Budgets, la décision de transférer à l'assurance maladie, le financement des 2 autres opérateurs de ce programme, l'agence de bio-médecine et l'École de hautes études en santé publique va dans le même sens et recueille en conséquence notre soutien. Même remarque sur la mise en place d'un système financier et comptable commun sur une étude de faisabilité d'une stratégie immobilière commune ces efforts de simples. Question sont tout à fait louable au sein du programme 183 sur le financement de l'aide. Médicale d'État, dispositif, ce dispositif ne peut plus continuer en l'état, le nombre de bénéficiaires de cette aide aide augmenter de 44 pourcent depuis 2009, c'est une dynamique inquiétante, une réforme, cela a déjà été dit dans cet hémicycle désormais incontournable, le rapporteur spécial préconisait un recentrage des soins pris en charge sur un. Panier de soins réduit, traitement des maladies graves, soit à la grossesse médecines présente. Qui veut, ce qui nous semble une mesure tout à fait utile et nécessaire, équilibrée dans la perspective du maintien de cette aide,

doit rapidement nous être présentées, merci de votre attente. Monsieur le président, monsieur le rapporteur spécial de madame la rapporteur pour avis madame la ministre, mes chers collègues, dans le cadre de l'examen des crédits de la mission santé du projet de loi de finances pour 2018 je souhaiterais aborder 2 aspects : la prévention, en particulier pour les enfants, adolescents et jeunes adultes, mais aussi la protection pour ce qui est de la prévention, je souhaite attirer votre attention sur la nécessaire reconnaissance des troubles dys en milieu scolaire et donc leur dépistage ces troubles spécifiques dyslexie 10 calculent il dyspraxie, dysphasie, trouble de l'attention touche un secteur isolé du cerveau d'autres secteurs comme l'Intelligence sont préserver les enfants 10 mettent en place des stratégies de compensation qui leur demande un coup intentionnel énorme diverses études montrent qu'un à 2 enfants par classe serait atteint l'école apparaît aussi comme lieu incontournable pour repérer et accompagner le plus précoce et mort le dépistage du diabète, en cette journée toute récente du 14 novembre consacre dépistage de cette pathologie, 3 millions de personnes sont concernées dont de plus en plus de jeunes, il est indispensable de sensibiliser la population risque de diagnostic tardif chez l'enfant et l'adolescent, on constate une très nette évolution du nombre de jeunes touchés par une nouvelle forme de diabète qui n'existait pas jusque dans cette population. Les risques pour la santé sont multiples, sans compter les conséquences psychologiques, la prévention est donc un axe majeur pour retarder l'entrée dans cette maladie, votre collègue de l'Éducation nationale, monsieur Blocher a annoncé ici même hier soir vouloir remettre sur pied la médecine scolaire, faire passer la visite médicale pour tous les élèves de 6 ans il a annoncé avoir engagé un travail interministériel avec vous, Madame la Ministre de la Santé, notamment pour que les médecins non scolaire puissent contribuer à la médecine scolaire et pourquoi pas proposer à terme afin d'attirer davantage de personnes vers la médecine scolaire, cette discipline comme spécialité lors du concours de l'internat en effet se former aux mesures de prévention n'est pas une priorité, aujourd'hui, au cours des études de médecine, je souhaiterais que vous nous indiquer, madame la Ministre, les actions que vous souhaitez engager dans ce domaine je d'ailleurs dans ce budget que celui consacré à la AME augmente de 75 millions d'euros en 2000 à 930 923 millions d'euros pour 2018, tandis que celui de la prévention dont on note une diminution de 4 millions d'euros pour votre population pour notre population jeune va donc diminuer, c'est pourquoi j'adhère totalement à l'amendement de notre collègue de la commission des finances à l'orage, Alain Joyandet, rapporteur au fond et portant diminution cette pour ce qui concerne la protection, je souhaite que vous nous disiez les actions du gouvernement envers les associations de protection, en particulier des jeunes homosexuels en errance être rejeté par sa famille et particulièrement déstructurant et peut conduire au suicide, bon nombre de jeunes se trouve contraint de quitter le domicile familial, son subside et en méconnaissance de leurs droits, j'ai été interpellé par des associations, notamment par le refuge créé en 2003 et reconnue d'utilité publique qui propose un hébergement et un secours d'urgence aux jeunes homosexuels et transsexuel âgés de 18 à 25 ans, est en situation de rupture familiale, du fait de l'Orient, l'orientation sexuelle, or la liste d'attente pour ces appartements relais et de plus en plus importante et ne peut être satisfaite dans le meilleur des cas, ces jeunes gens sont pris en charge par des structures d'urgence de droit commun, peu adaptés à ce public fortement exposée aux préjugés et discriminations au sein des populations marginalisées dans le pire des cas, ils se retrouvent dans la rue et structures d'accueil dédié sont donc en recherche de financement pérenne, quels sont les crédits alloués et quelle est leur évolution, enfin je souhaite attirer l'attention sur le soutien de ce qu'on appelle les aidants devant organisées bénévolement le quotidien de leurs proches, ils ont plus souvent le budget familial, car la maladie dans le cas, parce le patient atteint d'Alzheimer par exemple progressé les besoins évoluent, outre qu'il est extrêmement compliqué d'être aidant, lorsqu'on est en activité professionnelle, pensez-vous pouvoir ventilés dans ce budget, des dispositifs d'accompagnement financier autre dossier récurrent pour conclure, le manque de places dans les instituts médico-éducatifs les IME ainsi que les nombreuses difficultés qui découlent de cette carence cette situation génère une forte angoisse pour les parents et leurs enfants, elle ralentit et compromet leur avenir elle prive enfin nos territoires de structures adaptées, ainsi que la création d'emplois qui s'y rapporte, concurrence exercée dans ce domaine par les centres d'accueil, notamment en Belgique, qui traîne de nombreuses personnes qui ne peuvent pas bénéficier de places en France, merci de nous dire également si le dispositif de la marge d'amorçage pour ces structures va pouvoir fonctionner pour finir je veux évoquer le rapport de la Cour des comptes, tout récent, depuis hier et intitulé de l'assurance maladie, assurer l'efficience des dépenses, la responsabilité des acteurs, le rapport évoque aussi la possibilité de former les jeunes diplômés exercer dans des qu'zone sous-dense pour une durée déterminée de remplacer donc la carotte par le bâton, le changement de méthode Paris radical mais n'est pas loin de certaines des propositions nos collègues lors du débat du PLFSS me semble-t-il. Pour évoquer la difficulté que nous avons concernant ce désert médical chroniques notamment dans mon département, une petite illustration des difficultés d'attractivité à l'installation, être limitrophe d'une grosse ville avec facultés de Sting comme Reims mais dépendant d'une autre RS que celle des routes de France, à savoir celle du grand test qui est à Nancy, de fait, les étudiants de laine font leurs études en médecine à Reims, mais on l'obligation de faire leur stage dans le périmètre de leur université soit le grand test, les actionnaires peuvent donc faire le stage dans leur département, à 20 kilomètres de là, la bonification financière allouée aux maîtres de stage ne pouvant à 7 heures être payés par une autre adresse que celle du lieu d'études de lutter contre la désertification médicale, notamment dans les départements à faible densité, c'est un appel du pied, si vous me permettez l'expression, Madame la ministre pour modifier ce qui paraît être bien une absurdité, il ne faut, il ne faut pas oublier que le stage effectué par l'étudiant décide à 60 pourcent de son lieu d'installation, je ne veux enfin pour finir, vous dire que même si c'est un peu hors sujet, je ne peux que me satisfaire du tiers payant qui de généraliser devient généralisable, je vous remercie. La parole est à madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées pour 10 minutes. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, madame, rapporte le rapporteur tout d'abord, veuillez excuser l'absence d'Agnès Buzyn, il m'a demandé de la remplacer, car elle est partie en Guadeloupe, suite à l'incendie qui a ravagé le CHU de Saint-Martin, pardon de Pointe-à-Pitre, le budget de la mission santé que nous examinons traduit l'attachement du gouvernement au pilotage de la santé publique et à la préservation, dans l'intérêt de tous, des dispositifs d'accès aux soins, ouvert aux personnes en situation irrégulière, il porte comme l'ensemble du projet de loi de finances, un engagement de sincérité cet engagement conduit à remettre à niveau des dotations budgétaires précédemment sous-évalué et à faire évoluer en forte hausse des crédits de la mission, il augmente en effet 174 millions, soit une hausse à périmètre constant, de 14 pourcent entre 2017 et 2018 je souhaite commencer par évoquer l'aide médicale d'État, le gouvernement est attaché à préserver la même l'aide médicale d'État, en plus de protéger et d'apporter des soins ces bénéficiaires Directs permet, en effet, la protection de la population et la prise en charge à un stade précoce de certaines affections à risque de transmission. La prise en charge précoce des soins évite par ailleurs ailleurs une prise en charge ultérieure plus lourde et plus coûteuses les crédits de l'aide médicale d'État seront augmentés de 108 millions et porté à 923 millions en 2018 afin de financer dans une volonté de budgétisation sincère une dépense de guichet tendancieux dynamique, nous observons, il est vrai un léger infléchissement des effectifs bénéficiaires sur les derniers trimestres connu qui a permis de revoir à la baisse la prévision d'exécution pour 2017 toutefois, le gouvernement a souhaité construire ce PLF en retenant une prévision prudente et une dépense croissante à son niveau tendanciel celui constaté en moyenne sur les dernières années, nous souhaitons par ailleurs renforcer l'efficience de la gestion de la comme vous l'avez souligné comme toute prestation la Meuse doit être contrôlé et gérer au mieux par les organismes qui va servir ainsi à compter de mai 2000 2018, les 3 caisses d'assurance maladie de Paris, Bobigny et Marseille assureront l'instruction de l'ensemble des demandes des demandes d'AME en métropole cette mutualisation permettra, outre des économies de gestion, d'améliorer l'accès aux dispositifs par la réduction des délais d'instruction et l'harmonisation des procédures, elle permettra également de renforcer le pilotage et le contrôle des dossiers. Je veux évoquer après la AME le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante 2ème composante du programme 183 les crédits du budget de l'État destiné à doter le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sont reconduits à hauteur de lui millions, il s'agit bien sûr d'une contribution annexe pour le fond, le lequel est financé principalement au titre de l'Exposition professionnelle par la branche accidents du travail, maladies professionnelles de la Sécurité sociale, à cet égard, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit de doter le fonds de 270 millions en 2018 sa dotation correspond à ce qui est nécessaire pour faire face aux engagements du fond à l'égard des victimes de l'amiante et de leurs ayants droit, la mission santé comprend également le programme 200 consacré à la prévention à la sécurité sanitaire et à l'offre de soins ces crédits un peu moins de 500 millions ne couvre bien sûr qu'une petite partie de l'investissement collectif en matière de santé c'est vrai en matière d'organisation sanitaire c'est vrai également en matière de prévention puisque les prix crédits du programme qui a abondé le fonds d'intervention Régionale des agences régionales de santé ont été transféré cette année à l'assurance maladie, en réponse à vous madame la sénatrice les crédits prévention sont bien en hausse de plus de 3 pourcent par ailleurs mais ces crédits finance des composantes essentielles de notre dispositif de protection et d'expertise santé je tiens remarquer que la prévention sur le sur le le programme crédit tabac passe de 32 à 132 millions en 2018 par ailleurs sur l'autre programme le projet de budget qui vous est présenté procède à une simplification du financement des agences sanitaires en transférant à l'assurance maladie, le financement minoritaire de l'Agence de biomédecine et de l'École de hautes études en santé publique, cela permettra d'achever le travail de des croisements des financements de l'État et de l'assurance maladie commencer cette année avec la NSP, cette rationalisation permet également, au-delà de la simplification des circuits financiers, un recentrage de l'État sur les agences ayant à titre principal des missions de sécurité sanitaire 4 opérateurs de santé reste financé par l'État par le biais de la mission santé l'Agence nationale de santé publique, l'Agence Nationale de Sécurité des médicaments et des produits de santé, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Institut national du cancer, les crédits qui leur sont affectées sont en progression de 4,4 millions la négociation budgétaire a permis de prendre en compte le repassage nécessaire des agences afin de retrouver une trajectoire d'équilibre à moyen terme, tout en mettant en oeuvre les économies attendues des opérateurs de l'État dans le cadre du redressement des comptes publics. Dans les années qui viennent, l'Agence nationale de santé publique aura un rôle déterminant à jouer dans la déclinaison de la stratégie nationale de santé 2017, 2022 actuellement soumises à la consultation publique. Cette stratégie est bâti autour de 4 axes : prévention, égalité d'accès aux soins innovation pertinence ses qualité le 1er de ces axes fait du renforcement de la prévention tout au long de la vie, notamment pour la prise en charge des jeunes comme vous l'avez signalé Monsieur le Sénateur amiable qui est un domaine essentiel et dans tous les milieux, un objectif prioritaire pour lequel MSP est un acteur incontournable

au budget de l'INCa la NSP continuera également d'avoir un rôle primordial en matière de gestion des situations sanitaires exceptionnelles, compte tenu de l'accroissement des risques qui pèsent sur la santé publique sa mobilisation sans précédent pour la gestion des conséquences du cyclone Irma aux Antilles, en témoigne : plus de 450 réservistes sanitaires mobilisés sur place et 10 tonnes de matériel acheminé à côté du financement des grands opérateurs de santé le programme porte également les dépenses d'indemnisation des victimes de la dépakine pour un montant total de 77 millions contre 10 millions en RFI 2017 lors de la mise en place du dispositif satin modernisation et comme vous le savez, assurée par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, les premiers dossiers sont examinés depuis ce mois et le dispositif sera pleinement opérationnel avec les premières indemnisations dès 2018 ce sont là, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, les axes les plus saillants d'un budget qui participe avec l'ensemble des dépenses mobilisés par ailleurs dans le cadre du PLFSS à la mise en oeuvre de la politique de santé et d'accès aux soins du gouvernement, je vous remercie. Merci madame la ministre. Nous allons donc procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission santé figurant à l'état de.

Oui, merci Monsieur le Président, Madame la ministre Madame la rapporteure mais, chers collègues, il s'agit de l'amendement qui consiste justement à réduire les crédits de de alors c'est pas une arme un madame la ministre, c'est simplement une façon pour nous d'appeler vraiment cette fois-ci, y a une un véritable remise à plat de l'aide médicale d'État, je rappelle qu'il s'agit de l'aide médicale pour les immigrés en situation irrégulière, il s'agit pas de supprimer notre mission d'accueil, je veux juste dire que si on regarde un peu ce qui s'est passé dans les années d'avant, dans les années précédentes, il s'agit. Ah non plus, d'un amendement qui consiste à les crédits en concordance avec les besoins, parce que, en 2012 on a dépensé 588 millions pour cette aide médicale et on avait inscrit 588 millions donc on voit bien qu'il y a là il y a la possibilité de faire les choses comme il faut et et sans qu'on ait de sous-budgétisation je rappelle aussi que, en 2012, quand on a vu l'explosion il y a eu un certain nombre de raisons, parce que les conditions d'attribution de de l'AME on change, on pourrait peut-être y revenir tout à l'heure, il s'agit donc par cet amendement uniquement de revenir à une dépense qui soit dépenses raisonnables et a appelé le gouvernement à mettre sur la tête, je crois que les différents orateurs presque presque sur tous les bancs, ont tous dit qu'il fallait absolument revoir les conditions d'octroi et le périmètre de ses têtes médicale d'État, ce que nous demandons avec cette amendement ce que demande la commission des finances c'est que on mette vraiment à plat les conditions d'octroi de la qu'on revoit le périmètre peut-être avec des soins qui soient des soins, certes un peu moins, un peu moins nombreuses qu'on qu'on fasse face à notre à notre responsabilité de santé publique de soins d'urgences de maternité ne rien changer pour les enfants mais enfin là, on est quand même dans une consommation de soins qui est très très importante et il nous semble que nous nous avons la possibilité de changer cela et de revenir à une une consommation de de crédit qui soit un peu plus raisonnables, d'autant qu'on voit bien dans la mission, les autres organismes de santé publique sont rabotés et on a le sentiment qu'il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas contrôlée et qui continuent à filer comme ça sans que sans qu'on se pose la question de savoir si on peut faire autrement, je rappelle que le Sénat en 2015 sous l'impulsion de Roger Karoutchi avait déjà voté une réduction des crédits, qui était un appel à cette refonte de la M1 depuis il s'est rien passé donc on voudrait vraiment maintenant en adoptant cet amendement et j'appelle nos collègues adopté cet amendement, je ne fais pas d'illusions sur ce qui se passera après à l'Assemblée nationale, mais je pense qu'adopter cet amendement, ce serait vraiment un véritable appel une véritable demande à ce que c'est à émotion a remise vraiment à plat et qu'on voit comment, comment faire en sorte de continuer notre mission d'accueil tout en étant un petit peu plus raisonnable sur le plan sur le plan budgétaire et j'allais dire, même un peu plus équitable et on le voit bien dans la mission que nous étudions aujourd'hui. merci, monsieur le rapporteur, et je profite de ce début de séance pour demander à chacun à chacune de respecter les temps de parole, s'il vous plaît, un amendement 216 rectifier identique qui est défendu par monsieur Karoutchi. Seul président Madame la ministre, comme toujours dans dans ce genre de débat, il y a la réalité, et puis il y a le propos, le propos, il peut être soit démagogique soit extraordinairement critique parce que naturellement, dès qu'on touche à la santé il y a un côté extrêmement compliqué, la réalité elle est d'une simplicité totale et le rapporteur Alain Joyandet bien vient de le dire de manière très claire

Alain Joyandet aimablement rappelle que j'ai fait voter un amendement 2015, je me souviens d'un débat avec Madame Touraine à la commission des finances en 2014, ou elle l'avait pris l'engagement de remettre sur la table, la manière dont l'AME était attribué la manière dont la AME distribués, il s'agit pas de dire qu'on veut ne plus contrôler examiner l'état de santé, la capacité des enfants, des femmes, des des qui sont sur le territoire national par rapport à leur état réel, le problème c'est que on sait bien, et on voit bien que l'AME explose, que personne, en réalité, n'a la volonté politique, parce que c'est une question de volonté politique

parce que là, elle menait pas qu'en Île-de-France et à Marseille, la MEC partout sur le territoire national je j'attends de voir comment les choses vont être attribuées dans quelles conditions administratives, ça va l'être, la réalité c'est que : qui peut croire et j'ai souvenir de Madame Touraine, me disant jamais, vous m'entendez, monsieur le sénateur, jamais la haine le dépassera 7 à 800 millions d'euros, nous sommes à plus de 900 alors voilà, c'est plus d'un milliard l'année prochaine, c'est combien dans 5 ans si personne ne se décide simplement remettent sur l'établi, la manière dont la AME est attribuée donc madame la ministre. Tout va bien, si vous remettez sur l'établi si on revoit les conditions d'attribution si on veille à ses conditions d'attribution et, si on revient 300 millions d'euros, ça vous laisse unanime à plus de 600 millions d'euros, plus de 600 millions d'euros, c'était le niveau en 2014. Merci, cher collègue, quel est l'avis de la commission. Qui a déjà exposé son avis, l'avis du gouvernement. Je vais compenser par le le temps que j'ai à peine dépassé tout à l'heure pour Excel même amendement que celui de la Commission, donc forcément, nous sommes favorables. Merci, monsieur le rapporteur, quel est l'avis du gouvernement dans la minute. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, Monsieur le Sénateur, vous proposez de réduire de 300 millions la dotation de l'État finançant l'aide médicale d'État, au-delà, c'est l'AME elle-même dans sa configuration actuelle que vous souhaitez, remettre en cause le gouvernement bien sûr il est défavorable, je tiens à rappeler que la haine est un dispositif qui se justifie par des considérations humanitaires mais aussi sanitaire et économique et me protège les personnes concernées en leur permettant un accès aux soins préventifs et curatifs, ce qui limite la dépense de santé résultant d'une prise en charge tardive des pathologies, ce n'est donc pas une bonne idée de l'imiter comme vous le souhaitez, la même au sol prise en charge d'urgence car, dans ce cas, les personnes seront pris en charge plus tardivement, avec un coût des soins plus importants, enfin, le gouvernement est attaché à la sincérité du budget et la réduction de sa dotation affecterait très fortement cette sincérité pour toutes ces raisons, le gouvernement est défavorable à cet amendement. Madame taillé pour Lyon pour l'explication de vote. Monsieur le Président, Madame la ministre, messieurs, mesdames les rapporteurs Badia, pas de mesdames et rapporteur d'ailleurs mais chers collègues. Pour nous, la la haine est indispensable pour plusieurs raisons : elle permet l'accès aux soins à des publics qui en ont particulièrement besoin, elle a un rôle primordial et cela a été rappelé en matière de santé publique, en évitant que les affections contagieuses non soignée, ne s'étende, elle protège aussi de soins aussi de soins trop tardif, alors vous souhaitez réduire de 300 millions cette enveloppe est d'ailleurs et d'premièrement, on a du mal à comprendre puisque vous vous trouvez que cela résout un problème de sous-budgétisation, c'est ce que vous dites, un appel à réformer les les modalités de pour que les bénéficiaires de l'AME soit soit soit soit défini mais ça a déjà été fait en 2010 une majorité des républicains, a mis en place un certain nombre de choses et quatre observer un accès aux soins réduit pour des publics en difficulté et une augmentation en fait des coûts liés aux soins des personnes qui, après, finalement, ont dû y recourir parce que les affections se sont aggravées, vous parlez enfin régulièrement quand on vous entend sur ce type d'amendement du modèle allemand, mais le modèle allemand effectivement excluent un certain nombre d'affections et notamment les affections chroniques, donc moi je me souviens que un des premiers actes de de Valérie Pécresse effectivement à la région Île-de-France, qui était de supprimer le bénéfice des de de l'accès aux transports, aux bénéficiaires de l'AME c'est bien souvent un petit peu ce genre de public que vous visez auquel vous souhaitez retirer des droits alors qu'ils garantissent une politique de santé publique, qui est de de meilleure qualité, qualité, qui est finalement destinés à à protéger tant ces personnes qui sont particulièrement vulnérables que les Français dans leur ensemble, dont, bien entendu, nous nous opposons à cet amendement. j'ai bien écouté les auteurs de l'amendement et Roger Karoutchi, mais c'est une double négation du principe de réalité, d'abord c'est un amendement d'insincérité budgétaire sur un plan strictement financier. Puisque vous vous réjouissez que le le gouvernement et enfin à l'arrêt véritable auteur et sans rien modifier le vote de cet amendement ne modifierait strictement aucune des conditions légales d'attribution la vous donner un coup de rabot violent de 300 millions d'euros, donc vous faites un amendement d'insincérité budgétaire, c'est quand même un petit peu surprenant, deuxièmement, sur le fond, sur le fond, bah si ça me choque, voilà vous pouvez on peut prêcher tous ces son contraire si on veut, mais à ce moment là on parle pas du principe de réalité, le principe de réalité, c'est celui-là, par ailleurs, la question qui est posée des conditions d'octroi il faut là aussi se se conformer à la réalité, la réalité c'est que tous ceux qui soignent, qui prennent en charge des personnes autistes de la même saveur que les conditions d'octroi actuels sont en-deçà du cadre légal, il est compliqué, il est long d'obtenir une AMM, le délai est bien supérieure à 3 mois dans la vraie vie et le renouvellement annuel induit des ruptures du dispositif qui sont récurrentes et qui font que de nombreux professionnels de santé, de facto, à leurs à leurs frais des personnes titulaires de l'AME parce que en aucun cas en aucun cas les professionnels de santé n'abandonne des personnes qui ont besoin de soins et les hôpitaux sont confrontés à la même situation, avec des remboursements par l'État qui sont fréquemment pas à la hauteur des frais engagés au type de l'aide médicale État alors évidemment il faut accepter de regarder dispositif massivement là il faut réfléchir au cadre légal dans lequel on insère ce sera l'objet d'un amendement suivant que je vous présenterai mais si on refuse de mettre sur la table les conditions du dispositif et son lien avec l'assurance maladie qui existait avant 1993 avant 1993 ce dispositif était dans l'assurance maladie, pourquoi ne pas y revenir, pourquoi ne pas accepter de mettre sur la table les déterminante en terme sanitaire en terme économique du rattachement du dispositif de la même à l'assurance maladie. Merci, cher collègue Monsieur Rambeau investigation vote. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, notre le groupe la République en marche vote aura fermement contre cet amendement,

mais tout simplement vous dire qu'on doit dépenser ce que nous devons faire parce que nous avons encore une conception universaliste et humaniste de la santé merci. Madame Doineau, explications de vote. Oui monsieur largement expliqué tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur cette proposition d'amendement, en réalité, si nous pouvons partager des constats notamment de refonte du système de, de, de, de revoyure, il faut quand même admettre que les efforts qui ont été faits en matière de contrôle monte une certaine efficience justement de ce dispositif, il faut les poursuivre, il faut sans doute regarder très précisément, quel est le le panier de soins à apporter aux personnes qui ont besoin effectivement de d'avoir cette attention particulière mais pour autant est-ce que la fin justifie les moyens, et notamment de réduire, sur le plan budgétaire, je l'ai dit, il ne faut pas le faire parce que c'est une finalement une réponse d'insincérité que nous proposons, or nous avons été nombreux dans cet hémicycle, a toujours critiquer quand les lignes budgétaires n'étaient pas à la hauteur des besoins, donc c'est un peu contraire aux positions qu'on nous avions auparavant et par ailleurs, ces populations sont effectivement plus nombreuses donc mécaniquement, nous avons besoin d'une d'une ligne budgétaire plus importante, je voudrais pas m'étendre sur, par exemple, la présence de mineurs non accompagnés, mais ils sont là beaucoup plus nombreux qu'il l'était auparavant et en tout cas la population migrante est là et il faut leur apporter, c'est soit parce que c'est aussi, et pour eux et pour les accompagnants qui parfois sont aussi en dans une mise en danger si jamais nous n'intervenons pas sur ces problèmes de santé, donc, pour ces raisons, le groupe Union centriste dans sa majorité, ça se tiendra, pour ma part je je serais contre cette proposition d'amendement et et donc c'était, comment dirais-je, des positionnements assez partagée, mais plutôt sur l'abstention pour le groupe Union centriste merci. Merci, cher collègue Madame Doineau.

on voit les les chiffre le nombre de bénéficiaires de l'AME de droit commun, a diminué de 1,6 pourcent par rapport à 2015 et puis il faut rétablir une réalité aussi j'des exemples européens qui sont développés pour les justifier le désengagement des États membres européens quant à la couverture santé universelle, au nom de restrictions budgétaires, a lieu en Allemagne en Irlande au Royaume-Uni notamment les conséquences de ces mesures de restriction de l'accès aux soins des migrants se sont avérées néfastes pour les personnes vulnérables, notamment dans les pays tels que le Royaume-Uni, qui s'en sont servis comme finalement un outil de contrôle de l'immigration, le rapport de Médecins du Monde sur l'accès des réfugiés en Europe en 2016 est extrêmement éclairant sur la situation sanitaire ainsi de nombreux obstacles à l'accès aux soins ont été observés

ont limité leurs déplacements, de peur d'être arrêtés, contrairement au mythe de l'extrême droite sur les motifs de l'immigration, seuls 3 pourcent des patients déclare avoir quitté leur pays d'origine, entre autres, pour des raisons de santé, alors je suis désolé mais ces 2 amendements contribue à présenter la prise en charge des personnes éligibles à la à la comme un coût exorbitant pour nos dépenses de santé et donne dangereusement du poids aux arguments de la droite extrême, vouloir réduire les prestations de l'AME pour en faire une aide médicale à minima ou, comme l'a dit le rapporteur Joyandet raisonnable, je sais pas ce que ça veut dire finalement ne peut avoir que des conséquences négatives au plan humain comme ça ni. Claire ou encore économique, c'est ce que j'avais dit dans mon propos introductif, c'est ce qui a été dit par bon nombre de, de, de, de nos collègues et c'est d'ailleurs ce qu'a affirmé également madame la ministre, donc pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas ces 2 amendements. Merci, cher collègue, monsieur Baeza. Presque cassé de vote. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Me semble que dans cette assemblée, tout le monde sera d'accord pour reconnaître qu'un dispositif d'accès aux soins d'urgence pour les étrangers, compréhensifs, lui assure régulière et tout à fait nécessaire pour des raisons humanitaires, on l'a dit, pour des raisons sanitaires évidentes aussi qui contribuent à à protéger nos propres populations croit que ça, ça fait consensus mais pour que un dispositif aussi indispensable puissent être défendu devant nos compatriotes, il faut qu'ils restent raisonnables et en effet, quand en 5 ans de temps, on a un quasi doublement de la dépense, on peut s'interroger sur les causes de ce quasi-doublement en 5 ans, moi, je veux pouvoir continuer à défendre ce dispositif devant mes compatriotes et pour ça il faut qu'il soit encadré et que l'évolution de sa dépense encore une fois, restent raisonnables, d'autant que nous oublions pas que certains de nos compatriotes vont à l'étranger pour obtenir des soins qui soit leur souhaite accessible financièrement, notamment en matière dentaire, je parle pas évidemment du tourisme médical pour les soins ou la chirurgie esthétique mais bel et bien de soins nécessaires du point de vue dentaires comment leur expliquer qu'on a pratiquement l'expert, le doublement de nos dépenses pour l'aide médicale d'urgence et que dans le même temps on ne peut pas assurer leur propre prise en charge et puis 2ème point je voulais aborder ici ou également, c'est que je n'a été évoqué les flux migratoires qui est, on le sait bien, avec les mineurs étrangers isolés de plus en plus nombreux dans nos départements, on aura l'occasion d'en reparler, ces populations sont plus en plus nombreuses mais si cet amendement avait aussi pour effet de mobiliser l'État pour les reconduites à la frontière, dont on sait que le taux est particulièrement faible des personnes en situation irrégulière, il aurait aussi cet Avantage c'est pour cette raison que je voterai évidemment ces 2 amendements merci. Monsieur Karoutchi pour explication de vote. Oui, monsieur le président, Mesdames, ministre, c'est exactement le même débat qu'il y a 3 ans, avec les mêmes réactions et avec la même réaction du gouvernement qui consiste à dire : comment la main sur le coeur, comment vous pouvez nous dire ça et puis après, il se passe C'est-à-dire, vous prenez des engagements sur le thème : rassurez-vous, si vous êtes humains, on laisse les dépenses parce que naturellement il faut soigner accueillir et tout le monde est d'accord et le gouvernement systématiquement dit mais je comprends que par rapport à l'opinion publique, je comprends que par rapport à l'ensemble des Français, je comprends par rapport à la maîtrise des dépenses de santé qu'on impose à tout le monde, hé bien effectivement, il faut qu'on ait une meilleure maîtrise sans remettre en cause, mais une meilleure maîtrise de la et une fois qu'on a dit ça dans cet hémicycle, on sort de l'hémicycle, bonjour chez vous, il se passe plus rien. Et d'année en année on nous dit : ah bah tiens il faut rajouter 100 millions et et immédiatement, quand on dit bah c'est pas exactement ce qui a été dit, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, on nous dit : comment, comment vous voulez pas soigner les gens, c'est scandaleux, inadmissible et on nous redit ah bah alors, d'accord, si ces amendements passent pas naturellement, on va s'engager à une réforme à contrôler à soigner bien entendu mais à maîtriser et puis il se passe rien, parce que c'est compliqué, parce que finalement il y a pas de volonté politique, alors Madame la Ministre, évidemment, ces amendements ni Alain Jourdan, ni moi n'avons d'illusions à l'Assemblée nationale, même s'ils étaient ici, il passerait pas, ce sont évidemment des amendements d'appel et évidemment des amendements pour dire au gouvernement : attention, comme l'a dit notre collègue Bazin, à un moment, les gens l'opinion publique va dire ce système coûte 1 milliard alors que nous on doit faire des économies, on doit faire attention, etc, c'est plus possible, si vous voulez défendre le système en place, il faut forcément qu'il y a une meilleure maîtrise, une meilleure coordination et le fait que cette dépense restent maîtrisables pour nos finances publiques, s'il se passe rien et que, d'année en année vous revenez chaque fois en nous disant, ben la dépense augmente, il faut ajouter 100 millions à à un moment le système explosera de lui-même et de l'intérieur, donc je vous le dis, c'est pas une question de gens qui ont des sentiments humains et de gens qui n'en ont pas, c'est si vous voulez sauver le système maîtriser le. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, je voudrais dire à notre collègue, je crois que c'est la République en marche qui est ou quelqu'un qui a parlé d'insincérité budgétaire si on adoptait ces amendements, c'est pas vrai, c'est pas vrai, parce que les choses peuvent aller très vite, si aujourd'hui on décide une réduction budgétaire et comme l'a dit Madame le ministre de la ministre si tout de suite derrière, on s'attaque au périmètre de de la prestation, je vous rappelle juste que entre 2010 et 2012, on a fait baisser de 100 millions d'euros, la consommation des crédits, on a quand même accueilli les gens, on les a quand même soigner, aucun d'entre eux qui est arrivé en urgence n'a été soigné, je suis acteur de la de la politique de santé local du président de mon hôpital depuis 20 ans, je suis pas plus, j'ai pas

en un an en 2012, on passe de 588 millions à 700 44 ans non, c'est-à-dire plus de 26 pourcent pourquoi parce qu'on décide de supprimer le ticket modérateur, il y a pas ticket modérateur, on voit bien quand même, et donc on crée un appel d'air formidables et ça va très très vite, donc si on réduit les crédits et que derrière, évidemment, on reprend la politique, je pense qu'on peut être tout à fait, tout à fait cohérent, je veux dire aussi à notre collègue d'abréger le nom du groupe, madame la présidente, juste vous dire quand même que quand vous signaler la petite baisse de 2 sur un an la de du nombre de bénéficiaires, il faut quand même savoir que le nombre de bénéficiaires a augmenté

voilà, c'est ça la question qui est posée par cette par cet amendement, je pense qu'on peut tout à fait et d'ailleurs vous pouvez-vous vous rapporter au au au texte de notre de mon excellente collègue Madame Imbert qui vous donnera tous ces chiffres, s'est pas je ne sais pas, on raconte pas des histoires, il y a un vrai sujet, Madame la Ministre est-ce qu'on s'y attaque est-ce qu'on s'y attaque pas, il faut être généreux, mais c'est quand même l'argent public dans un moment où la France n'en a plus est-ce que c'est le seul endroit où on s'occupe pas de de contrôler et de de réduire un petit peu la prestation juste une seconde, comme j'ai pas utilisé montant tout à l'heure pour dire à notre collègue centriste que les contrôles se font y a eu 15000 qui ont été faits ces contrôles montrent que l'application des textes et tout à fait juste aller et les effet donc c'est pas la question, le le contrôle montre ça immonde, que les gens bénéficient de cette prestation dans le cadre des textes tels qu'ils sont adoptés, pour l'instant donc les contrôles oui il montre qu'il y a pas d'excès, mais il y a pas d'excès dans le cas de la politique actuelle et ça ne produit aucune économie budgétaire. Merci, monsieur le rapporteur. Madame Dindar m'a semblé que vous avez levé la main. Oui, j'ai collègues la politique marche avec la rigueur budgétaire, je n'en doute pas, mais la politique marche aussi avec une certaine philosophie autant la France met en place des allocations universelles de solidarité, autant il me semble que nous avons tous droits les être humain a le droit à la santé et aux soins de manière universelle, c'est en tous les cas le principe philosophique que nous devons défendre, c'est pour ça que avec beaucoup d'amitié, je dis à mon collègue que je voterai compte ces amendements. Merci, cher collègue. Je vais donc mettre aux voix, ces 2 amendements identiques, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe, la République en marche sur les amendements identiques 171 et 216 je vous rappelle que l'avis de la commission est favorable, l'avis du gouvernement est défavorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 65 du règlement, le scrutin sera ouvert dans quelques instants.

Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos, j'invite les secrétaire a procédé au depuis, mode de scrutin.

donc le le résultat du scrutin numéro 34 sur les amendements identiques ne ressent 71 et 216 rectifier, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs au groupes politique et notifié à la présidence Nombre de votants : 337 Nombre de suffrages exprimés 312 pour l'adoption 164 contre 148. Le Sénat a adopté.

Qui s'abstient, l'article 29 est adopté, j'appelle en discussion les amendements tendant à insérer des articles additionnels qui sont rattachés pour leur examen au crédit de la mission santé. Après l'article 62 bis. L'amendement 103 rectifier madame Darcos. Oui, merci Monsieur le président, mes chers collègues, je vais être un petit peu long mais je pense que ça vaut le coup pour vous d'entendre des explications un peu longue sur sur cet amendement, l'État est censé jouer un rôle essentiel en matière de protection et de promotion de la santé, comme en témoignent les initiatives lancées pour lutter contre la maladie de Line ou encore pour mobiliser la recherche française dans le cas des crises sanitaires mondiales telles que zika, où Ebola toutefois au delà des effets d'annonce, ils nous font nous interroger sur les moyens réellement alloués à nos chercheurs, l'exemple de l'INSERM est éclairant à ce sujet, cet institut de recherche et vu confier, pas moins de 9 plan missions depuis 2014, il a notamment été chargé du lancement du consortium réactive dont l'objet est de coordonner la recherche en cas d'émergence infectieuse, il a également reçu mission de piloter le plan France médecine génomique 2025 sur le séquençage du génome humain et de mettre en oeuvre le volet recherche du plan maladies neuro-déjà dégénérative, l'INSERM a encore été sollicité pour le plan de lutte contre la maladie de la reine, le plan anti-bio résistance le plan maladies rares 3 enfin l'opérateur de recherche porte un projet pilote dans le cas du plan cancer, un autre concernant les déficiences intellectuelles, ainsi qu'un dernier projet relatif aux maladies fréquentes, comme le diabète, pour l'ensemble de ses missions des financements des ministères de la Santé et de la recherche était attendue. Malheureusement, ils ne sont pas au rendez-vous, pas un centime. Dans son rapport spécial sur le projet de loi de finances pour 2017 notre collègue Michel Berson, rapporté que 43 millions d'euros correspondant au coût de son engagement nouveau n'avaient pas été versées depuis les financements nécessaires pour permettre à l'INSERM de répondre aux sollicitations d'État dans les prochaines années, ont dû être évalués et s'élève à près de 50 millions d'euros de telles charges pèsent évidemment sur le budget des opérateurs publics de recherche qui sont souvent conduits à devoir opérer des redéploiements internes, humains et matériels, une question se pose inévitablement au regard de cette situation, comment mobiliser et motiver les équipes sur le long terme constituer des cohortes avec une telle absence de visibilité financière l'amendement que nous vous proposons a donc pour objet de demander une évaluation précise des modalités de financement des plans de santé publique, nous souhaitons également qu'au terme de cette évaluation des propositions soient formulées afin de lever l'ensemble des obstacles juridiques et budgétaires altérant la capacité d'intervention des opérateurs publics de recherche j'associe bien évidemment mon collègue Alain Joyandet mais également Jean-François Rhein à cet amendement, je vous remercie. Merci, cher collègue. Quel est quel est l'avis de la commission je trouve que celui-là sera très très utile et je suis co-signataire Hatier personnelle mais la commission a adopté cet amendement, donc avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur, quel est l'avis du gouvernement. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous souhaitez un rapport sur les plans nationaux de santé publique et particulièrement sur le financement du volet recherche de ces plans, le gouvernement partage votre constat différents plans de santé publique ont été annoncés au cours des années écoulées sans que le financement des mesures prévues et toujours été suffisamment identifiée en amont, notamment pour celles qui concernent la recherche, il souhaite donc que désormais tout plan identifie les opérateurs qui devront le mettre en oeuvre et les ressources qu'ils pourront mobiliser pour ce qui concerne la recherche, la ministre des solidarités et de la Santé souhaite créer un programme national de recherche en santé publique, dont la programmation sera concertée avec l'ensemble des ministères concernés, en particulier le ministère de la recherche et de l'univers du l'innovation et avec les principaux opérateurs de recherche, ce programme de quoi reprendre de façon transversale des besoins de recherche identifiés dans les différents plans de santé publique mais seuls pourront y figurer des actions de recherche dont les financements seront identifiés afin d'éviter une programmation hors sol et n'intégrant pas la réalité des contraintes financières que connaissent des équipes de recherche, la production d'un rapport n'est peut-être pas le meilleur moyen de faire progresser ce sujet au bénéfice des explique pétasse des explications et des assurances que je viens de vous donner sur l'action du gouvernement, je souhaiterais donc que vous acceptiez de retirer votre amendement, sinon je serais défavorable, je vous remercie.

Oui, Monsieur le Président, la ministre, en fait, la question s'est posée puisque Madame Darcos s'est est venu exposer les principes de son amendement en commission des finances, et en tant que rapporteur spécial de la recherche, on l'a auditionné et je pense que son son idée bonne, puisqu'on est en plein changement de paradigme dans tous les sens aujourd'hui avec cet amendement à la proposition de ce rapport, le message de Madame Darcos dire est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui la recherche comme un moyen très utile de faire de la prévention médicale. moi je crois que oui et sincèrement cette idée qui au départ ne faisait pas unanimité et qui a demandé réflexion est tout à fait intéressante, se dire qu'on pourrait financer demain avec quelques crédits ou d'assurance maladie ou au travers l'assurance sociale des crédits sur la recherche dès lors qu'avait spécifiquement associés aux grandes pandémies ou alors à des maladies plus largement, c'est assez intéressant et ça demande réflexion, donc je pense qu'il n'est pas inutile de pouvoir travailler au travers, hein, un rapport qui associerait le monde de la recherche, bien sûr, les autorités sanitaires et des autorités de de la vie publique en général, sur cette question qui est qui, à mon sens fondamental. Donc je soutiens en tant que membre aussi de la commission des films des finances

il tomberait, entre guillemets, on n'aurait pas besoin forcément d'avoir cette étude mais comme dit mon collègue, je pense que ça fait trop d'années, et vous n'y a pour rien mais d'insincérité budgétaire ou des des promesses ont été faites et où surtout des gens, je pense à la magie de la une, parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup des os aussi à Sion, qui sont créés depuis quelques années, ils n'ont pas pour l'instant ils espèrent tous un vaccin, il y a pas une Corse qui a pu être organisé il y a urgence, on ne peut pas attendre et donc d'une certaine manière, je fais un peu pression à en maintenant cet amendement pour que les choses puissent se décider assez rapidement, on a encore des possibilités législative pour le faire, mais c'est vraiment un appel au secours, j'allais dire, on a levé une sorte de mini-se condamne l'État et donc je pour l'instant, je le maintiens. Merci, cher collègue, monsieur, je me pour explication de vote. Merci monsieur le président, c'est une vraie question : qui est qui est et qui, vous le savez, va plus loin en fait et bien plus loin que l'amendement que vous que vous déposez Joerg d'ailleurs que vous vous focalisez vous paraissez focalisé je ne sais que c'est pas le cas, mais sur l'INSERM je pense que ça n'est pas très adroit, en l'occurrence, mais cette question du financement de la recherche et du financement de la recherche en santé puisse être ça comme ça dont il s'agit je crois nous amène nécessairement à poser la question de la fiscalité en la matière, nous sommes dans un pays où, traditionnellement, ces financements relevés quasi exclusivement de la sphère publique et comme vous le notez la sphère publique a du mal à faire face maintenant à ce financements, la question se pose pour les IHU par exemple et pour l'avenir d'un certain nombre Didier hachures, à l'heure où un une nouvelle génération d'IHU arrive maintenant et donc vous savez que le modèle anglo-saxon est bien différent du nôtre et j'ai le sentiment que nous sommes en train, doucement, de quitter un modèle ou en tout cas de l'euphémisé sans dire vers quel autre modèle on va et ça, ça me paraît être une question centrale qui doit être posée sur la table par par la collectivité nationale votre amendement quand je l'élu sous soyez assurés que je lui avec beaucoup d'attention et plusieurs fois pour et j'ai essayé de, de, de, de comprendre si c'est ça qui vous motive de poser l'ensemble de cette question et à ce moment-là, moi je vous suis dans cette volonté-là et non pas simplement de poser la question particulière de l'INSERM et de quelques autres programmes de santé qui là est une façon, pardonnez-moi l'expression, mais on n'est pas sur le grand bout de la lorgnette. Merci, cher collègue, le seul enjeu. Madame la ministre, monsieur le président, hé bien moi je voterai cet amendement parce que je crois, comme il est expliqué effectivement par son auteur, je crois que c'est, c'est c'est important au salut les rapports Alain Joyandet, l'a dit, c'est pas évident effectivement à l'accepter tous les rapports, mais celui-là est important parce que, et je crois qu'il faut vraiment c'est un amendement qui permet aussi de faire un appel et puis de se dire que, il faut qu'on se penche sur certains sujets, je crois que vous avez donné un très bon exemple madrilène, je peux vous dire que, franchement, c'est quelque chose qu'il faut impérativement développer et mettre en place quand on voit et tout le retard que l'on a par rapport à certains pays et vous savez, quand vous êtes confrontés à ce genre de maladie, hé bien je peux vous dire que vous avez une réaction qui est complètement différente de celles et ceux qui n'ont pas remettre en cause, mais s'interroge sur l'utilité de cette amendement, je vous remercie. Merci, cher collègue Madame quand Oui, nous allons soutenir cet amendement, mais aussi parce que je trouve que non seulement la question de de Madame Darcos c'est extrêmement importante, mais y compris, il faut pas que nous soyons hypocrite, ici on n'a pas tellement de possibilités au plan législatif, d'aller plus loin sur cette question là que de proposer un rapport parce que il y a l'article 40 qui a été un véritable couperet, donc le rapport évidemment à chaque fois les mêmes arguments, encore un rapport encore un rapport mais là elle soulève une question notamment en santé qui est essentiel et il me semble important effectivement d'avoir des données de réfléchir ensemble, de confronter les points de vue qui peuvent être divergents, nous au niveau du groupe communiste républicain et citoyen plusieurs fois on a proposé d'essayer de réfléchir à un grand pôle public du médicament et de la recherche, c'est une idée qui peut être mis en débat qui peut évoluer etc, dirais-je dans cette proposition de rapport l'ouverture à des pistes de réflexion parce que quand même la recherche ce ne se porte pas bien du tout, et quand on a affaire à des chercheurs, au niveau de la santé, on s'aperçoit qu'il nous appelle, bien souvent au secours et pour aider des tas et des tas de, de, de maladie, donc moi et ainsi que l'ensemble de de mon groupe, nous allons soutenir cet amendement.

Merci monsieur le président, donc, cet amendement est relatif à l'aide médicale État et à l'évolution du dispositif donc je je prends note avec avec déception de la décision du Sénat. En renvoyant à l'Assemblée nationale, sans illusion, mais je trouve que ce n'est pas une une façon satisfaisante de procéder de couper les crédits de l'AME qui évidemment, seront rétablis par l'Assemblée nationale et heureusement parce que ils dépasseront ce qui serait à l'heure prévue, mais il faut pas arrêter là le débat, j'en suis, j'en suis bien d'accord et donc quel choix avons-nous simplement d'étudier des pistes de réforme du dispositif de l'aide médicale État la principale piste qui est sur la table et qui est défendu, encore une fois, par ceux qui s'intéressent à la santé publique qui est défendue par l'Inspection générale des affaires sociales qui est défendue par l'Inspection générale des finances en ce qu'elle estime qu'il y a là un puits d'efficience et de rationalisation de la dépense, même si ça n'est pas l'essentiel : dispositif aime mais j'entends cette préoccupation, l'Académie de médecine, je le rappelle, donc le 20 juin dernier dans un rapport très documenté, très 10 constat circonstanciés estime également que l'insertion du dispositif AME dans l'assurance maladie permettrait d'améliorer l'efficience du dispositif et son efficacité en termes de parcours de soin et de soins délivrés, je demande que le gouvernement mette cette piste de réflexion sur la table qui produisent oui également, là aussi, un rapport sur cette question mais pour éclairer notre assemblée et pour que nous puissions prochainement revenir sur le sujet, mais à partir de ces éléments objectifs objectiver quel impact en terme de santé quel impact en terme de coût du dispositif d'un d'un dispositif d'aide médicale État pris en charge par l'assurance maladie, ce n'est pas une révolution, c'était le cas, vous le savez, je le rappelle, avant 1993 1993 et j'allais dire, c'était le cas il y a eu bien plus de temps pendant lequel au ce dispositif était au sein de l'assurance maladie que d'autant qu'il a hors de l'assurance-maladie, donc je vous invite à voter cet amendement pour que nous puissions à partir de ce rapport délibéré de nouveau sur cette question, chaud, merci. Merci, cher collègue, quel est l'avis de la commission. et donc le fait de la noyer dans dans dans le reste de notre comptabilité je pense que ça ne serait d'abord pas une source de de clarté et puis en plus vraisemblablement toutes les raisons d'un élargissement et donc on irait à l'encontre je crois des amendements que nous avons voté tout à l'heure, c'est pourquoi la Commission a donné un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, quel est l'avis du gouvernement. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, cet amendement fait à 2 objets bien distincts, la couverture maladie des plus précaires et l'intégration de la ME dans l'assurance maladie et mon appréciation sera différente sur ces 2 sujets, parlons de l'accès effectif aux droits des personnes les plus précaires, je rappelle qu'un rapport d'information sur l'accès financier aux soins des personnes en situation de précarité et d'ores et déjà prévue à l'article 44 heures du PLFSS pour 2018 et portera notamment sur les bénéficiaires de l'AME, je pense que cette partie de votre amendement est donc satisfaite concernant, à présent, l'intégration des bénéficiaires de l'AME, l'assurance maladie, je ne peut-être que beaucoup plus réservé même l'assurance maladie relèvent de 2 logiques différentes : la ME a pour but de soigner des personnes démunies en situation irrégulière vivant sur notre territoire et relèvent à ce titre de l'action sociale et humanitaire financés par l'État, notre système de sécurité sociale et fondé lui sur des contributions obligatoires des assurés en contrepartie d'une couverture universelle face aux aléas de santé ce rapport propose d'examiner la fin de cette distinction primordiale, c'est une question lourde d'implications et l'on peut craindre que l'évolution suggéré n'aboutissant à l'effet inverse à celui escompté en affaiblissant l'adhésion à notre système de protection sociale, le gouvernement n'est donc pas favorable à cette avant Merci, Madame la Ministre, je mets donc aux voix l'amendement 206 rectifier bus qui a fait l'objet de d'un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances adoptées par l'Assemblée nationale pour 2018 : nous poursuivons l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances des différentes missions : le Sénat va examiner les crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. La parole est à monsieur Arnaud Bazin, rapporteur spécial de la commission des finances pour sa minute.

Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, ma mission Solidarité, insertion et égalité des chances, qui porte les politiques publiques de solidarité et de cohésion sociale de l'État en faveur des personnes les plus fragiles et doté de 19 milliards 400 millions d'euros de crédits de paiement en 2018 ces crédits progressent ainsi de 8,7 pourcent par rapport à 2017, soit une augmentation d'un peu plus d'un milliard et demi. Cette augmentation est principalement due au dynamisme des dépenses d'intervention que sont la prime d'activité, l'allocation aux adultes handicapés et les mesures de protection des majeurs qui représentent 80 pourcent des crédits de la mission. Madame la Ministre, ce budget n'est pas à la hauteur des enjeux de la mission tout d'abord, malgré la volonté louable de sa série station des crédits que nous constatons, après des années de sous-budgétisation des risques de dépassements budgétaires sont à prévoir en 2018, notamment pour la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés. S'agissant de la prime d'activité, l'enveloppe budgétaire prévu pour 2018 est d'ores et déjà en deçà des dépenses exécutées sur 2017 alors que les bénéficiaires ne cesse d'augmenter, l'année 2018 ne dérogera malheureusement pas à la pratique des années précédentes d'ouverture massive de crédits en loi de finances rectificative pour faire face aux besoins de ces dispositifs. Par ailleurs autre insuffisance de ce budget, la non-compensation des crédits issus de la réserve parlementaire alors que 6,6 millions d'euros avaient été ouverts en 2017, à ce titre sur la mission Solidarité, il s'agit d'un manque à financement important notamment pour les associations d'aide alimentaire, les Restos du coeur ont ainsi bénéficié de près de 700000 euros et la Banque alimentaire de près de 200000 euros, c'est pourquoi la Commission adoptée sur ma proposition, un amendement visant à rétablir ses crédits vitaux pour le tissu associatif. En outre, alors que l'égalité entre les femmes et les hommes a été érigée au rang de grande cause nationale du quinquennat par le président Macron la légère augmentation du programme dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes masque cependant des situations contrastées: le budget pour 2018 est ainsi marquée par une baisse regrettable d'un 1000000 800000 euros de crédit il y a la lutte contre la prostitution cette baisse compte revient ainsi à l'application effective de la loi du 13 avril 2016 mettant en oeuvre un parcours de sortie de la prostitution. Nous saluons donc la volonté de faire de ce programme une priorité politique mais faut-il encore qu'elle se traduise par des actes, je soutiendrai donc les amendements déposés par nos collègues visant à rétablir les crédits de l'action relative à la lutte contre la prostitution. Par ailleurs, bien que des enveloppes exceptionnelles étaient prévues dans ce budget, elles paraissent insuffisantes à couvrir les dépenses engagées. Il en est ainsi du Fonds d'appui aux politiques d'insertion le FAP et doté de 50 millions d'euros seulement et surtout du financement exceptionnel de 66 millions 800 1000 euros alloués au département au titre du remboursement des dépenses d'aide sociale à l'enfance pour l'accueil des mineurs non accompagnés supplémentaire entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017. Les départements ne peuvent plus faire face à l'afflux croissant de ces mineurs non accompagnés qui était, rappelons-le, 2500 fin 2014 et dont le nombre aujourd'hui est estimé à 25000. Malgré l'annonce du 1er ministre fin octobre devant le congrès de l'Assemblée des départements de France, de prendre en charge par l'État, les dépenses d'évaluation et de mise à l'abri en attendant cette évaluation, aucun crédit n'a été inscrite dans le budget, à ce titre pour 2018, c'est une source d'inquiétude pour les départements qui sont aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile, subissant l'organisation de véritables filières et accueillant de plus en plus de personnes majeures, les conduisant engagé d'importantes dépenses d'évaluation sur ce sujet, l'État doit plus que jamais prendre ses responsabilités et assumer ces dépenses qui relève de la politique nationale, d'immigration, nous attendons donc ainsi de la mission en cours sur le sujet qu'elle aboutisse à une clarification et à une traduction budgétaire rapide nous souhaiterions à cet égard, Madame la Ministre, connaître l'état d'avancement de cette mission. Malgré ses insuffisances que je regrette la commission des finances, a décidé d'adopter ces crédits puisqu'ils ont été rectifiés pour partie par 3 amendements adoptés par la commission, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Éric Bocquet rapporteur, rapporteur spécial de la commission des finances pour 5 minutes. Madame la Ministre, Monsieur le Président, c'est la commission des finances collègue mon collègue Arnaud Bazin parfaitement souligné les insuffisances budgétaires dont souffre cette mission mais il ne s'agit malheureusement pas des seuls madame la ministre, à la hausse des crédits de la mission s'avère à l'analyse des crédits budgétaires et une véritable augmentation en trompe l'oeil, évoquons d'abord les revalorisations de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés, ces revalorisations, que nous saluons masque en réalité des réforme paramétrique constituant autant de mesures d'économie au au détriment des populations les plus fragiles. Ne pouvant revenir sur les revalorisations promises lors de la campagne présidentielle, il semble, Madame la Ministre, que le gouvernement est trouvé dans ces réforme paramétrique des moyens discrets d'économies budgétaires, ces mesures sont d'autant plus regrettable qu'elles ont fait l'objet d'aucune concertation avec les acteurs, avec les acteurs concernés, pardon, et notamment les associations de personnes handicapées, qui nous ont exprimé leur plus vive inquiétude à ce sujet lors des entretiens, ces mesures d'économies concernent les 3 plus importantes dépenses sociales de la mission, la prime d'activité, la hache et la protection juridique des majeurs, elles conduisent ainsi de façon regrettable atténuer voire neutraliser les effets de revalorisation annoncée. Parmi ces réformes, l'exclusion au 1er janvier 2018 des bénéficiaires des rentes athée et MP de pension d'invalidité de la prime d'activité cette mesure d'économie, justifiée par le gouvernement, par le faible nombre de bénéficiaires actuels estimée environ 10000 personnes est à la fois injuste et injustifiée, Madame la Ministre, injuste car cette mesure touche encore une fois, les plus fragiles et va à l'encontre de l'objectif essentiel d'intégration professionnelle des personnes en situation du handicap et injustifiée, puisqu'en réalité, ce ne sont pas 10000 mais 250000 personnes qui seraient potentiellement concernés par ce dispositif, qui n'existe que depuis le 1er octobre 2016 et qui a fait l'objet d'aucune campagne d'information, c'est pourquoi la commission des finances du Sénat à l'initiative de mon collègue Bazin et moi-même, a adopté un amendement de suppression de l'article 63 rattaché à l'émission qui porte cette mesure d'économie, cette discrète réforme de paramètres n'est malheureusement pas la seule, le gouvernement prévoit également un rapprochement des règles prise en compte des revenus d'un couple à la hache sur celle d'un couple au RSA dès 2018 et à compter de 2019 la disparition d'un des 2 compléments de ressources de la le complément de ressources, d'un montant de 179 euros par mois, rappelons-le, il s'agit là d'un regrettable alignement par le bas de l'allocation adulte handicapé, conduit par le gouvernement qui, au nom de l'équité ignore totalement les difficultés d'une personne en situation du handicap non, selon nous, là, je n'ai pas un minimum social comme les autres, outre les personnes en situation du handicap, ce budget touche de plein fouet les personnes soumises à des mesures de protection dont la moitié se situe déjà en dessous du seuil de pauvreté, ce budget prévoit en effet la mise en oeuvre au premier avril 2018 qui ne réforme du barème de participation des personnes protégées, augmentant la part financée par les personnes protégées afin de compenser la baisse du financement public, il s'agit là d'un regrettable, désengagement de l'État, outre ce discret coup de rabot budgétaire au détriment des plus fragiles, la hausse du budget de la mission également la baisse à périmètre constant de près de 2 pourcent des crédits du programme 124 qui porte l'ensemble des crédits de soutien des politiques des ministères sociaux et la contribution de l'État au fonctionnement des au fonctionnement des agences régionales de santé. Les ministères sociaux ainsi que les agences régionales de santé sont ainsi touchés de plein fouet par des mesures de restriction budgétaire, justifiée par le respect de la trajectoire financières fixées par le gouvernement, la poursuite de ses économies et particulièrement de la réduction des effectifs au sein des ARS interroges sur la capacité de ces organisations, a fonctionné de façon viable ainsi pour ces différentes raisons, j'avais à titre personnel, émis un avis défavorable à l'adoption des crédits de cette mission, la commission des finances, a finalement décidé d'adopter ces crédits, telle que modifiée par les amendements évoqués, je vous remercie de rétention.

6ème mission budgétaire de l'État, elle arrive systématiquement en tête des ouvertures de crédits supplémentaires demandés dans les lois de finances rectificatives successives. Avec plus d'un milliard d'euros de rallonge l'exercice 2017 ne fait pas exception au principe cela et le caractère fondamentalement imprévisibles de la dépense publique en matière de solidarité et appelle du Parlement une vigilance particulière sur la sincérité des crédits demandés pour l'exercice à venir, la prime d'activité nous fourni depuis 2 ans, l'illustration, voilà une prestation sociale dans le succès, certes, ne se dément pas mais dont l'objectif repose sur une ambiguïté. Nouveau Millenium sociale ou incitation financière pour retour à l'emploi. Pour la très grande majorité de ses bénéficiaires, il semble plutôt remplir le rôle d'un supplément du RSA les chiffres figurant au bleu budgétaire confirme nos craintes, le taux de sortie de la connectivité n'atteint pas les 4 pourcent. Ilnur escale assumer désormais assuré son pilotage en tant que telle. Un grand sujet qui est aussi un grand projet tête pleinement évoquer la réforme engagée par le gouvernement de la location d'2 adultes handicapés. La revalorisation substantielle de ce montant, qui passera à 900 euros ici pour les normes 2019 est une bonne nouvelle, depuis le plan pluriannuel de revalorisation de la hache, lancé en 2008, peu de projets aussi ont bien sûr la matière ont été lancés, je tiens néanmoins mesdames et ministre à vous exprimer mon attachement au caractère spécifique de la hache et au danger qu'il y aurait à quelqu'un sur cette prestation, les critères généraux des autres minima sociaux qui sont, pour la part, conçue pour inciter à la reprise, inactivité. Le rapprochement initié de la tâche et du RSA sous le prétexte de réunir sous des principes communs, les différents leviers de la solidarité nationale présente selon moi le danger de la perte d'une spécificité à maintenir de plus nous serons vigilants à ce que vous puissiez apporter les corrections nécessaires pour que les différentes évolutions des périmètres d'éligibilité, la fusion du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome Elana pacte limité sur les allocations des personnes handicapées, nous connaissons, Madame la Ministre votre mobilisation et votre engagement. Face à l'immense défi encore à relever de la construction d'une société vraiment teasing de Thonon à vous assurer du soutien du Sénat dans la poursuite de ce combat, outre ces observations générales sur les 2 principaux programmes budgétaires de la mission, j'ai déposé au nom de la commission des affaires sociales, un amendement visant à rétablir le niveau des crédits de l'action du programme 137 relatif à la lutte pour la prévention de la prostitution et contre la traître de traite des êtres humains sous réserve de l'attention de l'amendement et en tenons compte de nos remarques qui parfois peuvent nous inquiéter, notamment dans la réforme de l'âge, c'est un avis favorable, que la commission des affaires sociales a émis à la direction de ces crédits, je vous remercie. Dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque discussion qu'on prend le temps d'intervention général et celui de l'explication de vote par ailleurs le gouvernement dispose au total de 10 minutes pour intervenir, la parole est à Madame Patricia Schillinger pour la République en marche et pour 6 minutes. Monsieur Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les crédits de paiement, la mission Solidarité, insertion et égalité des chances du projet de loi de finances pour 2018 élèves à 19,4 milliards d'euros, soit une augmentation de 1,5 milliard d'euros par rapport à 2017, cette progression de 8 il y a plus de 7 pourcent représente un effort considérable concentré sur 2 programmes de la mission, le programme 300 cas d'inclusion sociale et protection des personnes, en hausse de 14,38 pourcent et le programme fend Handicap et dépendance, en hausse de 6,93 pourcent comme le PLFSS ce 1er budget du quinquennat porte la double marque de la sincérité et de la lutte contre les exclusions, nous nous en Cilicie sincérité, d'abord en anticipant autant que faire se peut, le dynamisme des dépôts des dépenses d'intervention qui représente 92 pourcent des crédits afin d'enrayer la sous-budgétisation chronique de cette mission lutte contre l'exclusion et cela veut dire solidarité surtout, puisque les 2 principales mesures budgétaires de cette mission concerne la hausse de la prime d'activité et la revalorisation de l'allocation 11 adultes handicapés, ce sont là vie là des choix forts en soutien du pouvoir d'achat des salariés dont les rémunérations sont les faibles et qui exprime la solidarité de la nation avec les plus fragiles d'entre nous au sein du programme 304, soulignons la revalorisation de la prime d'activité dès septembre 2018 de 20 euros par mois pour les allocataires, dont les revenus sont compris entre 0 5 et 1,2 SMIC un point de vigilance dans le programme 304 concerne l'action 14 sur l'aide alimentaire, en effet, la disparition de la réserve talent parlementaire va impacter en particulier les Restos du coeur et les banques alimentaires comme le rappellent les rapporteurs spéciaux, ce sont près de 700000 euros dont bénéficie de Euro dont bénéficiaient les Restos au titre de la réserve en 2017 pour les banques alimentaires, alors que la campagne d'hivers Deep débutent les financements publics nationaux comme européens ne doivent pas faire défaut, nous comptons sur vous, Madame la Ministre, pour défendre une position volontariste dans les négociations européennes sur l'avenir fonds européen d'aide aux plus démunis, enfin, au sein de la mission 340 je veux saluer l'augmentation sans précédent du budget alloué à l'accueil et l'orientation des mineurs non accompagnés en Irak pendant 117 millions supplémentaires, le gouvernement prend la mesure de l'urgence à gérer dans le dans les départements avec près de 25000 mineurs pris en charge en 2017 au-delà de l'urgence humanitaire et budgétaire, l'État assumera à l'avenir, l'évaluation et l'hébergement d'urgence, de ces jeunes jusqu'à la confirmation de leur minorité, le 1er ministre fille est engagée s'agissant du programme handicapé dépendance dont les crédits en hausse de 6,6 pourcent sont portées à 11,3 milliards d'euros, l'objectif est de permettre aux 12 millions de Français touchés par le handicap de choisir librement leur mode de vie, l'allocation adulte handicapé, concerne 85 pourcent des crédits du programme avec 9,7 milliards d'euros sa revalorisation exceptionnelle en novembre 2010 de 860 euros plus de 900 euros par mois, enfin 2019 devrait permettre à 34000 personnes supplémentaires de bénéficier de cette aide, cela représente un effort budgétaire nouveau de plus de 2 milliards d'euros sur le quinquennat parallèlement les règles d'appréciation des revenus des bénéficiaires en couple seront rapprochés rapproché rapproché de celle d'autres prestations concrètement 876000 bénissez Sierre bénéficieront de la hausse, à taux plein, 155000 bénéficiaires en couple bénéficieront d'une hausse de leur pouvoir d'achat et pour cette il y a 20 pourcent de bénéficiaires, l'effet sera nous saluons cet engagement exceptionnel au service de la solidarité, quelques mots pour terminer sur le programme égalité entre les femmes et les lol quelques mots car, bien entendu, ni la discussion de cette mission budgétaire, ni même l'ensemble des missions d'un projet de loi de financement ne pourront épuisé cette priorité, culturelles, sociales, éducatives, économiques et j'en oublie, le président de la République en a fait d'ailleurs la grande cause nationale du quinquennat l'action de toutes les administrations, qui doit être le fil rouge de des politiques publiques, elle doit mobiliser les Budgets dans chaque ministère, évidemment ce de cette mission sont stabilisées pour 2018, si certains s'en inquiètent, je préfère relever le volontarisme du gouvernement en matière d'égalité professionnelle de conciliation des temps de vie et de lutte contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles madame la Ministre, le groupe la République en marche votre heure votera les crédits enfin faire et solidaire, qui de plus s'inscrive dans une trajectoire de croissance pour atteindre ben tiens virgule 5 milliards d'euros en 2001, il y a tant à faire pour réformer et protégé, nous sommes prêts, Madame la Ministre. Merci, cher collègue. La parole est à présent Madame Nassimah Dindar du groupe Union centriste pour 6 minutes chers collègues. Monsieur Monsieur le Président, Madame la Ministre, mais sur l'aéroport de rapporteurs spéciaux et pour avis, chers collègues, parce qu'elle porte les crédits de politique, s'adressant aux plus fragiles de nos concitoyens, les publics vulnérables comme les publics précaires la mission, insertion, égalité des chances que nous portons en discussion générale aujourd'hui est une mission capitale cette importance n'a retrouvé en termes financiers 6ème on l'a déjà dit en masse budgétaire près de 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros destinés à qui, aux plus démunis pour l'aide alimentaire, l'aide sociale à l'enfance, mais également aux jeunes majeurs aux mineurs non accompagnés aux femmes victimes de violences aux travailleurs précaires aux personnes porteuses de handicap à la vie associative, oui, cette mission est essentielle car elle porte pour la République, la mission de la solidarité nationale aussi mon groupe salue l'augmentation des crédits en hausse de 8,7 pourcent qui porte sur les 4 programmes et les rapporteurs ont eu l'occasion de le dire tout à l'heure, ce budget aussi, je veux le rappeler, se veut plus sincère et nous reconnaissons posséder pense particulièrement dynamique, la difficulté de prévoir les crédits nécessaires à l'attribution des 2 principales allocations c'est-à-dire celles pour les personnes porteuses de handicap la hache mais aussi la prime d'activité, ce que rappelle d'ailleurs le rapporteur qui redoute encore une fois, pour cette année une sous-budgétisation sans en faire grief, nous craignons cependant des artifices et ajustements justement en contradiction avec les annonces faites par le gouvernement

Pour que chacun comprenne des personnes porteuses de handicap peuvent être exclus du versement de la prime en fonction du taux du nombre horaire dont ils vont bénéficier, travailler. Ce qui remet en même temps en cause le caractère universel de cette allocation, notre groupe soutiendra dès lors l'amendement des rapporteurs visant à supprimer l'article rattaché à cette mission. En contrepartie, le gouvernement prévoit une augmentation des crédits alloués à la hache, sur laquelle je m'attarderai un peu plus comme mes collègues, je salue cet effort qui s'adresse à des personnes particulièrement vulnérables. Je rappelle que l'allocation adulte handicapé, fera de manière différenciée en fonction du taux du handicap de l'âge et de revenus notamment et les crédits annoncés pour 2018 c'est à 9,7 milliards d'euros. L'augmentation de ces crédits c'est Split par la revalorisation de la ceux que nous saluons et qui devrait atteindre les collègues l'ont rappelé tout à l'heure un maximum de 900 euros en 2019. Comme cependant je m'inquiète des conséquences du gel des compléments de ressources pour les couples. Comme eux, je m'inquiète de l'alignement des règles prise en compte des revenus d'impôt bénéficiant de l'allocation adulte handicapé sur celle applicable à un couple qui touchent le RSA le diable se cacherait-il dans les détails. Au fond, nous ne sommes pas, je veux le rappeler dans la même logique, Madame la Ministre. Quand nous parlons de la précarité dans l'emploi que soutient que doit se tenir la prime d'activité, d'ailleurs, même les étudiants ou les contrats d'apprentissage sont susceptibles de toucher la prime d'activité, nous ne sommes pas dans la même logique, quand nous parlons des porteurs de l'handicap qui soutient la vulnérabilité dans le parcours de de vie le plan personnalisé de compensation d'accompagnement de la personne, droit à la compensation inscrit dans l'esprit de la loi de février 2005. Pour rappel, cette loi établie, c'est la différence entre les ressources pour vivre et de l'autre la compensation financière des dépenses entraînées par le handicap. Vous l'aurez compris, madame la ministre de l'article 63 du PLF opère bien un rétrécissement et un cloisonnement des publics qui lui qui va à l'encontre de l'objectif d'une société inclusive. Je ne crois pas, pour ma part, un seul instant que le gouvernement est voulu trouver des moyens discrets d'économies budgétaires, je crois, et le groupe Union centriste avec moi, je crois, et le le groupe appelle plutôt à une coordination des dispositifs et existant entre la hache, lâche le complément de ressources, la N-VA l'allocation d'invalidité, le complément de l'allocation invalidité entre les aides PCH qui soit versée par les MDPH entre les compléments versés sur la E par les Alpes par la Caisse d'allocations familiales pour les jeunes de moins de 20 ans c'est véritablement un marasme de différents dispositifs qui existent pour les personnes porteuses de handicap, j'ai presque envie de dire que c'est tout aussi compliqué que de se retrouver dans les couloirs du Sénat oui je crois qu'une simplification et coordination de toutes les aides humaines animalière technique de frais d'aménagement ou même de logements : ce que la N-VA accompagne ceux qui ont alors un homme, je m'en individuel ou d'un véhicule doivent pouvoir être simplifiées pour cette raison et parce que la difficulté ne peut se transformer en discrimination notre commission demande la concertation avant la fusion N-VA et complément de ressources souhaitée par le gouvernement.

Jusqu'à la majorité puisque pour pour les enfants atteints d'handicap irréversible, puisque cela n'ont pas été concernés par les réformes du décret de février 2017 qui allonge la durée jusqu'à 20 ans 10 et 20 ans la la la la rachat été concernés, mais pour les parents qui ont des enfants porteurs de handicap, c'est encore la croix et la bannière puisque tous les 2 ou 5 ans, ils doivent refaire des demandes de de de renouvellement de la hache la protection et l'accompagnement des enfants et des familles vulnérables, a fait donc aussi, et je veux le rappeler ici pour l'accompagnement des mineures dans ce programme 304 de, de, de, de, de, de, d'un effort particulier, financier par le gouvernement, je veux vraiment le le soulignée et cette proposition puisque nous passons ce qui était de 31,9 millions d'euros en 2017 à 143 millions d'euros pour conclure, économie 18 la prise en charge des mineurs non accompagnés, pourra être ainsi faciliter et les départements qui en assurer la charge jusqu'ici salue cette initiative, la collecte Élisabeth Doineau l'avait souligné, c'est pour cela que notre groupe, nous allons voter avec les réserves que nous avons faites sur les amendements, nous allons voter favorablement pour ce budget présenté par la mission, solidarité, je vous remercie. Merci, cher collègue. J'ai une petite faiblesse c'est ma voisine de l'océan Indien, pardonnez-moi. La parole est à monsieur Jean-Louis Touraine du groupe socialiste et républicain pour 7 minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. D'abord quelques remarques générales, l'examen du PLF intervient dans un contexte de croissance retrouvée. Grâce aux politiques conduites durant le précédent quinquennat les efforts de tous les économies réalisées les réformes structurelles autorise de l'optimisme et des recettes supplémentaires. nous devrions être au moment de la juste répartition des fruits savoureux la dynamique restaurée et la plus grande partie de la corbeille a déjà été attribué avec plus de 5 milliards d'euros aux particuliers fortunés déjà repus sur la mission Solidarité, insertion, égalité des chances. L'augmentation des crédits de la mission peut paraître confortable, en réalité, elle s'établit à 2 1 pourcent par rapport aux dépenses réalisées par Ainsi, la solidarité n'est pas au hit-parade des priorités du gouvernement, et pourtant c'est le plus sûr moyen d'assurer par la cohésion sociale annulant collectif pour une nouvelle croissance, ce que confirme aujourd'hui le FMI. Les cadeaux aux plus riches oblige malgré le surcroît de recettes en modérer les bénéfices pour les plus modestes. Et à le dissimuler derrière un discours flatteur qu'aucun de nous ne renierait si on ne reprenait en sous-main ce que l'on a accordé la prime d'activité fournit une fois de plus, l'illustration d'une politique en parfait trompe l'oeil. La prime d'activité a été un vrai progrès pour les travailleurs modestes à la contribué à réduire le taux de pauvreté et à augmenter le pouvoir d'achat, elle a remplacé la prime pour l'emploi et le reste, RSA chapeau dont le taux de recours était inférieur à 35 pourcent. Le nombre de bénéficiaires a crû très vite avec une moyenne d'environ 155 euros il y a constitué une incitation retour ou au maintien dans l'emploi ainsi dans une conjoncture difficile 9 pourcent des allocataires du RSA socle sont devenus éligibles à la prime d'activité en 2017 et 79 pourcent des bénéficiaires ont conservé leur emploi, la prime d'activité promise à une augmentation de 20 euros par mois mais. Enfin, 2010 18 bien sûr, les dépenses réelles de 2017 atteignait 6 milliards 5 2018 connaît une inscription à même hauteur, ce qui laisse entendre une volontaire sous-estimation ou alors une réduction non avouée du périmètre des bénéficiaires, c'est déjà le cas avec la suppression de la prise en compte comme revenu du travail des rentes AT-MP. Les rendant inéligible, la prime d'activité, ceci est une grande violence. à l'égard de ceux qui justement sont les victimes de leur travail. Pour la prime de Noël, 476 millions d'inscrits, alors que l'année d'ici 2017 se soldera par une dépense de 556 millions même sous-évaluation pour le RSA jeunes c'est 8 millions en 2016 presque 10 millions en 2017, seuls 5,4 millions nous sont proposés en 2018 à propos de sous-évalué, évaluation, permettez-moi d'évoquer un souvenir. Le débat passionné sur la fameuse prime d'activité débat au cours duquel s'était lancé en 2016, la majorité sénatoriale voulait entrer tenter de montrer sa capacité à proposer des économies, ce qu'on lui conteste et en même temps, plaisir suprême. Pouvoir qualifié d'insincère le PLF 2016 elle avait voté un amendement dans la conclusion était celle-ci : le présent amendement se veut plus réaliste et retient un taux de recours égal à celui du RSA, soit 32 pourcent et donc une réduction de 650 millions d'euros, ce qu'elle avait voté la vérité cruelle parfois le taux de recours sera fin 2017. De 70 pourcent. Tromperie encore que les commentaires autour des crédits pour la hache du programme 157 en réalité ils n'évolueront que de 3,9 pourcent par rapport à la consommation réelle. Et l'augmentation est entâchée de quelques artifices regrettable. L'obsession d'alignement par le bas. Ou par décalages calendaires reporte l'augmentation de la rage au 1er novembre comme la plupart des mesures sociales. Les mesures fiscales, elles, tels que la CSG sont applicables dès le 1er janvier prochain-t-elle déferlement de report en fin d'année constitue pour le budget 2019, une véritable bombe à retardement alignement encore par le bas, sur le RSA pour les coupes de bénéficiaires de l'AAH jusqu'alors chacun recevait son à Château au taux plein le coefficient multiplicateur demain sera de 1 virgule 9 puis de 1 virgule 8 diminuant les ressources du ménage reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre, en communiquant seulement sur ce qu'on a donné est devenu une règle que nous saurions. Que dire de la primauté exceptionnelle prise par le verbe sur l'action. C'est un fossé. Que dis-je un ravin. Un océan qui sépare parfois le discours de la réalité ainsi l'égalité entre les femmes et les hommes est érigée au rang de grande cause nationale, alors les crédits de l'action en faveur de l'égalité professionnelle, politique et sociale entre femmes et hommes diminue de 12 pourcent. Ils sont amputés de 35 pourcent ces crédits sur l'action 15 portant sur la prévention et la lutte contre la prostitution. Et l'avenir pour les plus modestes et les collectivités ne se dessine pas sous les plus heureux auspices de nombreuses questions restent en suspend les allocations individuelles de solidarité grèvent dangereusement les Budgets des départements, la négociation engagée par Manuel Valls sur la renationalisation du RSA n'a pas abouti. Et la réduction des ressources. De laisser le CNS a affecté au département vont encore passer de 70 à 61,4 Les déclarations du président de la République lors de la conférence des territoires en faveur du regroupement des allocations individuelles de solidarité le reprise en main par l'État n'augure rien de bon pour la population la plus vulnérable de notre pays. Il apparaît bien. Que la tentation libérale d'un welfare à l'américaine minimale des dispositifs d'insertion réduit au profit de petits boulots sous statut d'auto-entrepreneur demeure manifestement présente chez certains. Déjà la diminution drastique des contrats aidés dans la LFI pour mai 2018 en est un signe précurseur. Beaucoup de générosité pour les riches. Un peu de compassion pour les pauvres. Rendent inacceptable pour nous, les propositions de la mission Solidarité.

Madame la ministre, Madame le Ministre, Mesdames et messieurs, mes chers collègues, les crédits de la mission Solidarité, insertion, égalité des chances élèveront donc à 19,4 milliards d'euros pour 2018, comme l'a rappelé le rapporteur pour avis, notre collègue mouillé, traduisant une augmentation notable de ce budget de 8,9 pourcent par rapport aux crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2017, de manière générale, cette mission a connu une augmentation structurelle de son niveau de dépenses au cours de 8 dernières années, de 2009 à 2017, le montant des crédits de paiement à périmètre constant, est donc de 11,5 milliards à 19,. Un milliard d'euros, nous pourrions nous enthousiasmer, voyant dans cette augmenté. Sion de crédits notent une attention accrue des pouvoirs publics sur ce sujet de société, mais la question n'est malheureusement pas si simple, c'est une mission très importante pour les finances publiques et pour notre système de protection des plus vulnérables, cette mission se place en conséquence aussi. 6ème rang des missions budgétaires de l'État à untel, niveau de dépenses, il serait légitime de. Pouvoir compter sur un pilotage sans faille, pourtant ces dépenses souffrent d'un éparpillement des responsabilités, nous avons parfois le sentiment d'avoir mis à la mer à navire sans pilote, il y a un grave dysfonctionnement sur lequel notre groupe souhaite alerter le gouvernement et le Parlement en effet la mission Solidarité un certain. Son égalité des chances. Il est au coeur de l'action publique en matière d'attention portée aux personnes les plus en difficulté, pourtant, lors de son discours, le rapporteur a évoqué une sous-budgétisation systématique du programme depuis 2012, le gouvernement affirme avoir trouver des remèdes. Nous analyserons attentivement vos propositions de programmes de cette mission, méritent une attention plus particulière, le programme s'cas d'inclusion sociale et protection des personnes, caractérisé par une hausse de 15 pourcent de ses crédits marquée par l'augmentation de la prime d'activité, c'est un signe fort pour revaloriser le travail, mais il ne faut pas que le gouvernement récidive dans ses erreurs de chiffrages qui ont eu de lourdes conséquences budgétaires, les 2 dernières années, le programme 157 Handicap et dépendance est lui aussi marqué par une hausse de 7 pourcent de ses dépenses, intégrant l'annonce d'une revalorisation de l'allocation adulte handicapé notre groupe approuve cette. Mesures importantes en faveur des personnes en situation de handicap, notre groupe aimerait. Enfin, attirer l'attention du gouvernement sur le projet de sujet des mineurs non handicapées ils seront presque 25000 en 2018, soit 2 fois plus qu'en 2016 sous la responsabilité sociale et financière des départements, une charge de plus en plus lourdes et à terme insoutenable pour nos collectivités territoriales, les crédits consacrés à l'accueil de ces jeunes autre augmenter de 6 741 pourcent entre 2017, 2018 il y a urgence à anticiper les effets de l'accueil de ces personnes sur notre système de sécurité sociale et à trouver de nouvelles sources de financement pour assumer ces dépenses, est éminemment politique de réglé dans les plus brefs délais, ils nous proposerons plusieurs amendements pour tenter de résoudre ce défi, monsieur le Président, Madame le Madame la Ministre Mesdames et messieurs les sénateurs, Sarko lègue le groupe les indépendants républiques et territoires s'abstiendra sur le vote des crédits de la mission Solidarité, insertion, égalité des chances, si notre groupe salue les initiatives prises par le gouvernement en matière de solidarité, il ne peut s'accommoder de la sous-budgétisation chronique de cette mission concernant les mineurs non accompagnés, ce budget affiche une trajectoire qui nécessitera un suivi approfondi et une meilleure anticipation en matière d'accueil. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Marc boutiques du groupe RDSE pour 6 minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, chers collègues, la mission Solidarité insertion il été des chances s'est dotée en 2018 de 19,4 milliards d'euros en crédit de paiement, la plaçant comme cela déjà été dit en termes d'inscriptions budgétaires au 6ème rang des missions de l'État. L'importance de cette mission ne se mesure pas uniquement en termes financiers, elle recouvre en effet un ensemble de mesures essentielles qui traduisent le volontarisme des politiques d'insertion et de solidarité de notre pays. Si ces dispositifs qui associe à la fois des notions de prévention d'aide et d'incitation sont indispensables, leur évaluation, c'est-à-dire le niveau de satisfaction des objectifs auxquels ils doivent répondre, s'avère souvent difficile, ce qui rend l'appréciation de leur pertinence ou de leur efficacité très approximative, à cet égard, on peut s'interroger, me semble-t-il, sur la faiblesse du niveau de sortie de certains dispositifs comme la prime pour l'emploi, où le taux de sortie pour dépassement de revenus n'est que de 4 pourcent ce qui voudrait dire que le caractère incitatif de cette mesure pour favoriser le retour à l'emploi reste très limité. Les augmentations budgétaires concernent principalement les dépenses d'intervention qui représente plus de 90 pourcent des crédits et qui porte sur 2 dispositifs majeurs : la location aux adultes handicapés et la prime d'activité, hache qui mobilise, elle, seules 9,7 milliards d'euros enregistre une progression de 40 millions d'euros pour financer la hausse de 50 euros par mois à partir du 1er novembre 2018, la prime d'activité qui représente 5,1 milliards d'euros, est en progression de 240 millions d'euros pour couvrir la majoration de 20 euros par mois du montant forfaitaire à compter d'octobre 2018 ces évolutions mairie de 3 remarques : elle correspond pleinement aux engagements pris par le président de la République et le gouvernement bon pas toutefois les date de déclenchement de ces revalorisations en fin d'année, reporte l'essentiel de l'effort budgétaire sur l'année 2019, et les années suivantes, enfin la modification des périmètres définis pour accorder ces aides suscite quelques interrogations et il ne faudrait pas en termes d'applications que certains publics fragiles sont trouvés exclus, ce qui donne lieu à certains amendements qui ont été adoptés par la commission des finances du Sénat un amendement qui ont l'Avantage de sécuriser certains publics et de rapports, je dirais de de revenir à certains dispositifs, mais au prix d'un rabotage sur un certain nombre d'autres programmes qui ne sont pas forcément une excellente opportunité. L'augmentation des crédits s'appuie également sur des enveloppes exceptionnelles comme le fonds d'aide à l'insertion doté de 50 millions d'euros et des dépenses d'aide sociale en France pour les mineurs non accompagnés, pour un montant de 60 6,8 millions d'euros crédits alloués au département au titre du remboursement de 30 pourcent des dépenses engagées. Sur ce dernier point, il s'agit d'une véritable explosion du nombre de bénéficiaires qui serait estimé à 25000 en fin d'année 2017 alors qu'il n'était que de 2500 il y a 3 ans, vous imaginez donc ce que représente le reste à charge pour les départements dont les finances sont un déjà par ailleurs très largement sollicitées en matière de social et de solidarité, cette progression rapide non maîtrisée qui impacte très fortement. toutes les collectivités mais surtout un petit nombre de collectivités quelques départements de métropole et 2 départements ultramarins en particulier Mayotte et la Guyane, relève d'une politique nationale d'immigration acceptée ou subie, dont l'État doit assumer l'entière responsabilité en termes financiers, cette situation alarmante, a d'ailleurs fait l'objet au printemps dernier d'un rapport d'information de nos collègues, Élisabeth Doineau et Jean-Pierre Godefroy dénommé mineurs non accompagnés, répondre à l'urgence qui s'installe et qui préconisait une trentaine de mesures allant d'une meilleure maîtrise de l'immigration à l'approfondissement des partenariats avec les départements. Enfin, le programme concernant l'égalité entre les femmes et les hommes enregistrent une légère augmentation de crédits qui ne semble toutefois pas à la hauteur des ambitions du président de la République et du gouvernement d'en faire une grande cause nationale du quinquennat je modéré quand même cette appréciation en précisant que ce programme faisait depuis plusieurs années l'objet d'une sous-consommation récurrente de ces crédits. Enfin, on peut noter avec satisfaction les efforts accomplis avec une baisse de 27 millions d'euros sur les dépenses support, les dépenses de personnel lié à une optimisation des moyens de fonctionnement en conclusion, même s'il demeurent des interrogations et des inquiétudes sur l'évolution budgétaire pour les années à venir de certains programmes l'augmentation d'1,5 milliard d'euros. Qui, peut-être, s'avérera insuffisante, mais l'augmentation de cette mission en 2018, en progression donc de 8,7 pourcent ce qui n'est pas négligeable représente sans doute une approche plus sincère, un effort conséquent dans le contexte actuel ainsi avec les membres du groupe RDSE je vous invite, chers collègues, approuver les crédits de cette mission. Merci, Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Michel Forissier, pour le groupe, les Républicains et pour une minute. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, chers collègues, s'il y a un domaine où l'effort de la nation ne doit pas faiblir, c'est bien celui de la solidarité, donc j'ai de cette mission est de permettre à tous ceux qui sont en grande difficulté de garder l'espoir, même si vous certains ce n'est qu'une lueur d'espoir par l'expression de la solidarité républicaine, les crédits de cette mission 40 de 19 milliards et demi à peu près augmente, notamment en raison de la revalorisation de la prime d'activité de 20 euros par mois et de l'allocation aux adultes handicapés de 50 euros par mois à taux plein, on ne peut que se réjouir de ces progressions cependant les rapporteurs de la commission des finances et de la commission des affaires sociales on noté parallèlement des de rabot des économies décidées sans concertation qui touche les populations les plus fragiles, c'est toute l'ambiguïté de ce budget ou des mesures très concrètes et populaires voisinent avec des restrictions plus discrète, tout d'abord, concernant la prime d'activité qui remplace l'ancienne prime pour l'emploi et le reste R c'est ça activité le dispositif monte bien en charge avec un taux de recours à 75 je ne m'attarderai pas sur le risque de sous-budgétisation hélas récurrent je souhaite davantage rappeler votre attention sur la trique 63 qui vient exclure du bénéfice de la prime d'activité, les personnes titulaires de pensions d'invalidité ou de rente, suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, nous avons bien entendu, on nous dit : si on les arguments avancés par le gouvernement, la prime s'écarterait de son objectif initial d'incitation à l'emploi, en intégrant ces publique et le taux de recours serait trop faible pour ce qui concerne le principe d'incitation à l'emploi, je note qu'il est d'ores et déjà bien peu effectif puisque seulement 4 pourcent des titulaires de la prime d'activité sortent du dispositif pour avoir dépassé les conditions de ressources, reconnaissons-le, la prime d'activité fait aujourd'hui surtout figure de minimum social et ne respectent guère la philosophie ayant motivé la création du RSA quant au taux de recours qui serait trop faible, il n'appartient au gouvernement, au gouvernement d'ailleurs d'assurer des actions d'information auprès des publics concernés, bref, ces raisons ne me semblent pas suffisantes pour priver les personnes modestes d'un complément de ressources dont elles ont fortement besoin notre groupe suivra donc l'avis de la commission des finances en votant la suppression de l'article 63, je ferai un constat similaire concernant l'évolution de la vétusté et bien évidemment à l'effort budgétaire

cependant 2 mesures viennent neutraliser la portée de la prochaine revalorisation, il s'agit en 1er lieu du gel du plafond de ressources pour un couple percevant la hache la justification étant d'aligner leur régime sur les règles applicables aux recevant le RSA près d'un quart des allocataires de la rage sont concernés, à l'image de notre rapporteur Philippe mouiller, je déplore que le gouvernement pratique un alignement par le bas de la en suggérant une parenté entre les 2 prestations alors que la situation des personnes handicapées doit rester spécifiques de plus une seconde réforme ne figurant pas dans ce PLFSS car envisagée pour 2019 forêt fusionner les 2 compléments de la le complément de ressources complétant encore d'incapacité supérieure à 80 pourcent disparaîtrait au profit d'une augmentation de la de la majoration pour la vie autonome ici également sans concertation et sans assurance du maintien d'un niveau équivalent, on comprend bien sûr l'inquiétude des associations je rappelle d'ailleurs que si la loi est de 860 euros en 9 en 2018 et de 4 900 euros en 2019 le seuil de pauvreté et 2015 euros par mois la seraient toujours en dessous, notons considéré que les handicapés vivent en-dessous du seuil de provoquer concernant les autres programmes de la mission, je veux dire un mot sur l'amendement du rapport Philippe mouillée augmentant les crédits dédiés à la lutte contre la prostitution, je voudrais en effet souligné l'incohérence qu'il y a de diminuer de 26 et demi pourcent les crédits de cette action alors que les dispositions de la loi du 13 avril 2016 doivent être mises en oeuvre cette année la loi en effet prévu un parcours de sortie de la prostitution, comprenant une aide financière et un accompagnement social et professionnel, le décret d'application tardé à paraître et il a fallu un an pour l'obtenir mais rien n'empêche maintenant d'appliquer le dispositif, encore faut-il disposer de fonds nécessaires, je ne sais quel sort sera réservé à l'amendement de notre commission une fois parvenu à l'Assemblée nationale, on peut s'en douter, aussi nous avons de nous donnons-nous rendez-vous dans quelques mois, madame la ministre, pour faire le point sur le déploiement du parcours de sortie de la Poste qui tue, dernier point, je me réjouis qu'un amendement du rapporteur Arnaud Bazin tente de réparer les conséquences de la suppression de la réserve parlementaire certes à l'Assemblée nationale, un amendement du gouvernement arrive introduit 25 millions d'euros à destination des associations, via le Fonds pour le développement de la vie associative, cependant, nous sommes loin du compte, comme on dit, le compte n'y a pas, ce sont 147 millions qui étaient attribués au moyen de la réserve parlementaire de 61 millions destinés aux seules associations donc le coup de rabot et de 36 millions au passage dans le domaine de la solidarité, les associations d'aide alimentaire, les associations venant en aide aux personnes vulnérables et celles oeuvrant pour les droits et la défense des femmes sont fortement impacté et ne peuvent fonctionner avec la faible compensation prévue par le gouvernement, je ne vais pas rouvrir le débat que nous avons, il y a quelques mois ce sera inutile, mais encore faut-il que le gouvernement prenne ses responsabilités et propose des solutions, je crains bien sinon que ce soit nos petites communes qui paye la note comme d'habitude. Pour conclure en 1000 ces réserves, notre groupe, constate l'évolution positive des crédits de la mission, ce n'est pas un concert de lamentations qu'attendent nos concitoyens les plus fragiles, mais des décisions politiques qui les aident à surmonter leurs difficultés quotidiennes, madame la ministre, pour l'instant, nous sommes satisfaits de la qualité de votre écoute, nous espérons maintenant que vos réponses démontreront que vous nous avez entendu notre vote sera donc conditionnée par l'adoption des amendements déposés par nos rapporteurs dans un esprit de justice sociale dans la tradition et l'esprit du Sénat et, enfin, que ce budget respecte son objectif de protection des populations les plus fragiles, je vous remercie, je compte sur vous Madame la milice. Merci, cher collègue là. Parole est à Madame Laurence Cohen, du groupe CRCE pour sa minute. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la mission Solidarité, insertion et égalité des chances et l'un des piliers de la politique sociale menée par l'État, aussi nous jugeons positives, l'augmentation des crédits de un virgule 5 milliards d'euros par rapport à 2017 alors que les inégalités sociales grandissent et que les révélations sur les concentrations des richesses entre les mains de quelques puissants les rendent de plus en plus inacceptable, il est indispensable que l'État à établir ou rétablir la justice sociale, dans cet esprit, nous nous félicitons de l'augmentation de la prime d'activité de 20 euros à partir du 1er octobre 2018 dans le programme inclusion sociale et protection des personnes, mais nous souhaiterions que le gouvernement fasse du non-recours à cette prime, qui représente 4,2 milliards d'euros de prestations une urgence quant au programme Handicap et dépendance, il voit ses crédits augmenter de 6,9 pourcent par rapport à l'an dernier en raison de la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés, qui va passer progressivement de 860 euros à 900 euros, c'est donc une bonne nouvelle pour les bénéficiaires de la même si nous regrettons que le montant demeure en dessous du seuil de pauvreté, mais ces mesures positives ne doivent pas occulter les reculs contenues contenues dans 7 millions comme l'a notamment souligné notre collègue Éric Bocquet le gouvernement 6 une erreur en apparence prévoit en réalité de l'être pour un nombre plus restreint de bénéficiaires puisqu'il modifie les conditions et les plafonds de lâches c'est décision justifiée par un mélange des genres, puisque le gouvernement applique les critères des minima sociaux sur la roche, alors même que cette allocation ne fait pas partie des minima sociaux, versée à ses bénéficiaires au type de la solidarité nationale il faut redire ici que c'est une allocation versée aux types de la contention du aux personnes handicapées qui se trouve dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer un emploi, ou dont les pensions nature contributives sont d'un niveau insuffisant, ce sont 108000 couples qui vont ainsi perd le bénéfice de la avec la baisse du plafond du cumul à taux plein pour un couple d'allocataires, la fusion des 2 compléments de ressources de la page va entraîner une perte de revenus de 75 euros à 179 euros, c'est la double peine pour les personnes en situation de handicap, enfin je tiens relayé l'inquiétude des établissements et service d'aide par le travail, à qui le gouvernement avait promis la subvention 2000 emplois supplémentaires mais à qui a finalement décidé de, de réduire de 6 pourcent quand on sait que sur les 3,5 millions de personnes handicapées 500000 sont au chômage, cette décision est parfaitement injuste quant au programme 137 qui a été beaucoup commenté ces derniers jours, si le montant des crédits en faveur de l'égalité femmes-hommes est effectivement en légère hausse par rapport à 2017, nous continuons de dénoncer son insuffisance regard des enjeux au regard de la priorité gouvernementale affichée de plus au sein de ce programme, comment ne pas s'insurger devant la baisse des fonds destinés à financer le dispositif de sortie de la prostitution qui sont amputés de 25 pourcent, nous avons été alertés comme notre rapporteur par de nombreuses associations féministes et nous partageons totalement le fait que la loi de 2016 votée de haute lutte ne puisse être mise en oeuvre qu'à condition d'en avoir les moyens, or l'enveloppe destinée à l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle a fils est réduite de 1,5 millions d'euros, alors même que cette allocation est centrale dans le dispositif pour reprendre pied et retourner dans le droit commun, vous savez bien, mes chers collègues, quelle est censée suppléer à la baisse de revenus résultant de l'arrêt de la prostitution et que ces parcours de sortie donne accès à un logement ou d'allocation à des papiers, le cas échéant à des cours de français des formations, autant dire que sans A6 aucun parcours de sortie ne peut aboutir, l'amendement du rapporteur votée à la à la commission des lois répare cette baisse mais en privant d'autant le programme 124 qui concerne les politiques sanitaires, sociales de sport, ce n'est pas un transfert d'enveloppes, qu'il faut mais mais une hausse du budget, d'où d'autres abstention sur cet amendement aussi permettez-moi de réitérer mes doutes sur la réalité de la priorité gouvernementale concernant la lutte pour l'égalité entre les familles, en fait, je voudrais évoquer la situation des mineurs isolés, désormais nommé mineurs non accompagnés, l'augmentation des crédits consacrés à leur accueil passe ainsi de 20,1 millions en 2017 à 132 millions d'euros en 2018, comment ne pas se réjouir d'une telle hausse tant qu'il est vrai que de plus en plus de départements tire la sonnette d'Allah, mais cette générosité du gouvernement s'accompagne d'une mesure extrêmement grave puisqu'il va instaurer pour les jeunes exilés non accompagné d'un régime particulier, obéissant aux droits des étrangers plutôt correct de protection de l'enfance, nous sommes avec les membres de mon groupe, très préoccupé par cette décision, tout comme le défenseur des droits et de nombreuses associations de protection de l'enfance, d'autant que la volonté du gouvernement de confier à l'État, l'accueil d'urgence et l'évaluation de l'âge de ces jeunes jusqu'à ce que leur minorité soit confirmé, est un véritable transfert de compétence du département à l'État la convention internationale des droits de l'enfant, considère qu'un mineur isolé doit se voir accorder la même protection que toute autre enfant définitivement ou temporairement temporairement privé de son milieu familial, pour quelque raison que ce soit je conclurai mon propos en soulignant qu'il est nécessaire de mobiliser les moyens à la hauteur des ambitions que l'on se donne ce seul critère, s'il est important, ne saurait être suffisant, ainsi, malgré l'augmentation des crédits globaux de cette mission nouveau votre nous voterons contre, car comme je viens de le montrer, elle comporte des dispositions qui constituent de nombreux et inadmissibles recule, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées pour 10 minutes madame la Ministre. Monsieur le président, Mesdames et sénatrice Monsieur le Sénateur, messieurs les rapporteurs tout d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de Madame Buzyn Madame Schiappa qui ont été retenus, je vous remercie de l'ensemble de vos interventions relatives au budget de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances de la loi de finances pour l'année 2018 que donc je vous j'ai honneur de vous présenter aujourd'hui ce budget est le reflet d'un parti pris et d'une priorité, ce parti pris, c'est celui de la sincérité budgétaire qui est le préalable indispensable à une action publique efficace et des choix politiques clairement assumé cette priorité, c'est celle qui va nos concitoyens les plus fragiles et qui exprime la solidarité nationale. Les crédits de cette mission en son temps, essentiellement consacrée au financement des dispositifs d'aide aux populations les plus défavorisées au travers du programme 304 inclusion sociale et protection des personnes 157 Handicap et dépendance, ainsi qu'au soutien de l'égalité entre les femmes et des hommes les moyens de fonctionnement du ministère représente moins de 8 pourcent du total des crédits de la mission, le budget de la mission augmentera en 2018 de 20,5 milliards, soit plus 8,7 pourcent par rapport à 2017, c'est un effort considérable et cet effort est destiné pour l'essentiel aux bénéficiaires de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés, il s'ajoute, je veux le rappeler à l'Europe à la revalorisation prévue par le PLFSS d'ici au 1er janvier 2020 du minimum vieillesse d'un total de 100 euros par mois, s'agissant du programme 157 Handicap et dépendance, il est porté à 34 milliards, soit plus 6,9 pourcent d'augmentation entre 2017 et 2018 ça peut augmentation massive traduit la priorité pour le quinquennat que constitue que constitue elle permet de concrétiser l'engagement du président de la République en faveur de la revalorisation de l'allocation pour adulte handicapé, handicapé, afin de donner à tous leur juste place dans le projet national et de lutter contre la pauvreté subit des personnes auxquelles leur handicap interdit ou limite fortement l'accès au travail, la revalorisation de la vache permettra de porter en 2 temps, vous l'avez rappelé le montant de l'allocation à 900 euros par mois fin 2019. Il s'agit d'un investissement de plus de 2 milliards et demi d'euros sur le quinquennat que fait la nation au profit de la participation des personnes et leur inclusion pour permettre à chacun une vie plus libre et plus digne,

vous m'avez alerté sur les 2 mesures accompagnant cette revalorisation, en particulier celle consistant à rapprocher, et non pas aligner les règles de calcul de l'allocation pour les couples trop différente de celles des autres minima, j'entends dire que de ce fait, les coupes seraient exclus de la réforme et c'est faux et je tiens à vous rassurer ainsi, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Sénateur Forissier sur ce sur ce sujet : plus de 155000 bénéficiaires en couples vont bénéficier pleinement de la revalorisation, soit plus de 180 euros par mois, le niveau de revenu garanti un couple va rester par cette mesure strictement préservé et stable à hauteur de 1620 euros, soit un montant supérieur au seuil de pauvreté,

s'agissant de la simplification annoncée des de complément de ressources ne sera effective qu'en 2019 nous nord, nous aurons l'occasion d'y revenir dans le prochain débat budgétaire, je souhaite simplement vous rassurer sur les 2 objectifs qui nous guideront et ainsi répondre à Madame la sénatrice Dindar supprimer toute double évaluation et flécher les financements sur ceux pour lesquels la charge de logement et la plus élevée, simplifier et ne plus surévalué concernant le programme 304 je veux en 1er lieu évoqué l'augmentation de la prime d'activité, elle est, vous le savez, pour plus de 2 millions et demi de foyers aux ressources modestes un complément de revenus importants: près de 160 euros par mois en Maurienne, alors que le montant moyen de ressources des foyers bénéficiaires et de l'ordre de 1050 euros, elle est aussi un dispositif important pour faire en sorte, comme il est dit parfois de façon raccourci que le travail paye, conformément aux engagements du président de la République, la prime d'activité augmentera de 20 euros à partir du 1er octobre 2018. Je veux rappeler que l'augmentation, réalisé en 2018 va compléter une 2ème mesure favorable au pouvoir d'achat, la suppression des cotisations salariales, chômage et maladie en contrepartie de la hausse de la CSG, qui va se traduire par exemple pour une personne au SMIC par un gain de pouvoir d'achat de 263 euros par an lorsque la mesure sera pleinement monte en charge, il ne s'agit pas d'ailleurs avec cette augmentation de la prime d'activité que de la 1ère étape d'une hausse qui se poursuivra au cours des années suivantes pour porter la revalorisation de la prime d'activité à 80 euros, au niveau du SMIC. En 2018, 5,1 milliards seront donc consacrés à la prime d'activité, ce qui représente une augmentation de 16 pourcent par rapport à l'année 2017 cette augmentation prend en compte pleinement l'évolution tendancielle de la prime en opérant pleinement l'effort de sincérité, demandée par la Cour des comptes, la très forte progression des crédits s'accompagne de mesures destinées à modérer l'impact budgétaire, vous les avez relevé relevé ne remettent pas en cause, je le dis clairement l'économie globale de la prime et l'impact favorable des mesures adoptées pour les bénéficiaires, toujours au titre du programme 304 le parti pris de la sincérité porte également, le gouvernement a proposé d'augmenter de façon très importante, les crédits consacrés aux mineurs non accompagnés sur ce dossier important sensible les engagements du président de la République et du 1er ministre sont très claires : l'État doit faire plus et mieux pour accueillir les mineurs étrangers isolés et des départements dans cette mission, le nombre de mineurs pris en charge par les conseils départementaux, a augmenté de façon très importante entraînant la saturation des dispositifs et un coût croissant pour les départements, or, même si la protection de l'enfance et de la compétence des départements, l'État a une responsabilité forte au travers de sa double compétence de conduite de la politique migratoire et de protection de l'enfance exercée par l'autorité judiciaire. La situation actuelle révèle aussi la nécessité d'une harmonisation nationale des conditions d'évaluation de la situation des demandeurs d'emploi des demandeurs, pardon, compte tenu des disparités constatées entre les départements, c'est pourquoi le 1er ministre a lancé conjointement avec le président de l'association des départements de France, Dominique Bussereau, une mission d'expertise pour identifier des solutions opérationnelles permettant d'améliorer l'efficacité, la cohérence et la soutenabilité budgétaire de la phase d'évaluation et de mise à l'abri des mineurs non accompagnés. Dès 2018, l'engagement de l'État se traduira par un renforcement très important des moyens dans le projet de loi de finance qui passe de 15 millions en loi de finances initiale pour 2017 132 millions en PLF 2018, je tiens à rassurer aussi la sénatrice Schillinger et monsieur Baeza que pour leur dire que les crédits à l'aide alimentaire augmente de 7,7 millions. Je souhaite à présent évoquer le programme s'entraîne cette dont Marlène Schiappa porte la responsabilité par ses enjeux et objectifs, la politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes participent à la politique d'inclusion sociale pour permettre à chaque citoyen et à chaque citoyen de participer pleinement à la vie de la société, et notamment en exerçant un emploi l'égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause nationale pour tout le quinquennat elle porte un engagement fort sur tout le territoire en mobilisant l'ensemble du gouvernement dans une approche résolument en interministériel, sur les 3 champs prioritaires que sont la promotion et l'égalité professionnelle et la conciliation des temps de vie la lutte contre toutes les formes d'agissements et de violences sexistes et sexuelles, un État exemplaire grâce à l'efficacité des politiques ministérielles et interministérielles en faveur de l'égalité. Les actions réunis par le document de politique transversales totalise près de 420 millions en progression par rapport à 2017, à l'issue du Tour de France, égalité en mars prochain, le président de la République réunira en comité interministériel et validera un programme gouvernemental qui sera mis en oeuvre jusqu'à la fin du quinquennat dans déjà les crédits du programme 137, égalité entre les femmes et les hommes sont en hausse de 8 pourcent par rapport à la loi de finances de 2017, j'insiste sur la CSeries de sincérité de ce budget, qui représente de surcroît un taux de réserve de précaution de 3 pourcent contre 8 pourcent en 2017 qui donnera plus de marge de manoeuvre dès le début de l'année pour garantir la bonne consommation des crédits du programme je souligne aussi le que le niveau global de subventions aux associations dont le rôle est essentiel sur l'ensemble du territoire, c'est pourquoi l'engagement du gouvernement est aussi de pérenniser ce niveau de crédit tendanciel 2018, 2022 je n'oublie pas, enfin, que le projet de défendu devant la représentation nationale porte des supports budgétaires des femmes et des hommes qui travaillent dans nos ministères avec les programmes budgétaires 124 de soutien politique sanitaire, social du sport, de la jeunesse et de la vie associative, ce sont 18276 employes de l'administration centrale des services déconcentrés du ministère des agences régionales de santé ainsi que la masse salariale correspondante qui sont concernés, le projet de budget 2018 s'inscrit dans une perspective fixée par le président de la République de réduction du nombre d'emplois publics, or les départements ministériels prioritaire ce contexte Jean va donc requérir davantage d'efficience, nous allons tous ceux qui travaillent ensemble pour conclure, Mesdames et messieurs les députés, mais sénateur mais budget que nous vous présentons est un budget rigoureux dans son élaboration et un budget sincère, je vous remercie. Nous allons apprécier à présent procéder à l'examen des amendements pourtant sur les crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, figurant à l'État B.. à l'article 29 États B l'amendement 205 défendu par monsieur le rapporteur Bazin. Merci Monsieur le Président, Madame la ministre, cet amendement tire les conséquences de l'amendement de suppression de l'article 63 vous êtes proposé article rattaché à la mission cet amendement visait à ne pas exclure de la prime d'activité, les bénéficiaires de pensions d'invalidité de rentes accidents du travail, maladies professionnelles, mesure qui devait permettre une économie de 20 millions d'euros, selon le gouvernement, le présent amendement prévoit ainsi de compenser la suppression de cette moindres dépenses en diminuant les crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement et d'immobilier des ministères sociaux porté par le programme 124 en effet, les gains de productivité déficience attendu en 2018 ça je sens de la politique d'achat, dans le cadre de la nouvelle gouvernance des achats de l'État et surtout de la politique immobilière nous permettent cette proposition par ailleurs, ce programme fait l'objet d'annulation régulière par le gouvernement, gestion en 2016, 154 millions et demi en autorisations d'engagement et 48 et demi en crédits de paiement, le dernier décret d'avance de juillet 2017 avait procédé à une annulation de 59 millions d'euros en autorisation d'engagement et de 69,7 millions d'euros en crédit de paiement dont 22 millions en en autorisations d'engagement et crédits de paiement pour les dépenses support aura RS du programme 124 donc le présent amendement vous propose de tirer les conséquences de l'amendement de suppression de l'article rattaché à la mission en majorant leur l'action 11 donc de 20 millions d'euros en autorisation d'engagement et crédits de paiement et de réduire à due concurrence les crédits du programme 124 en diminuant d'un 1000000 d'euros l'action dysfonctionnement des services d'un 1000000 d'euros l'action 11 systèmes d'information et surtout de 18 millions d'euros l'action 12 affaire immobilière, donc c'est un amendement qui a reçu un avis favorable de la commission des finances.

le gouvernement est opposé à la suppression de l'article 63 en conséquence, il est opposé à l'amendement que vous proposez de plus la budgétisation du programme 124 est déjà très contrainte des dépenses de fonctionnement courant hors immobilier, systèmes d'information et ARS sont ainsi prévus en baisse de 7,4 pourcent et celle de communication de 10 pourcent vous propose ainsi de minorer les crédits inscrits à l'action 12 affaire immobilière, alors que ces derniers couvrent des dépenses obligatoires telles que l'ensemble des dépenses locatives des ministères sociaux en conséquence, il est par nature impossible de réduire ses crédits de 18 millions correspondant à 20 pourcent des crédits inscrits en PLF pas par ailleurs une minorité une minoration de un 1000000 sur les crédits inscrits en paix la FA l'action 11 systèmes d'information serait de nature à mettre en péril l'action des ministères sociaux en matière de modernisation et de sécurisation de leur système d'information, alors même que cette action a été reconnues comme prioritaires, enfin, il convient de signaler que les crédits du père du programme 124 ont été réduits de 900 dans le cas d'une mesure de rabot adoptée en 2ème délibération à l'Assemblée nationale pour gager les ouvertures pratiquées par ailleurs sur d'autres programmes, dans ces conditions je ne peut-être quatre défavorable avec à votre avant moi. Monsieur Touraine pour explication de vote. Merci Monsieur le le président. Bien entendu, nous sommes favorables à l'objectif visé par l'amendement,

pour autant. La proposition qui nous est faite, c'est de prendre sur des programmes sociaux pour augmenter, d'autres programmes sociaux, ce qui paraît tout de même difficile à accepter, alors on nous dit qu'il y a déjà eu des diminutions dans les années passées, notamment de 118 millions d'euros de crédits de paiement mais on peut pas continuer tout le temps comme ça jusqu'à ce que Morse ensuivie ya ba a bien un moment où il faut s'arrêter parce que les besoins sont supérieurs eux qui sont affectés par conséquent sur l'objectif, nous sommes d'accord sur les moyens de transfert d'un programme social un autre programme social, nous ne pouvons pas être et, par conséquent, nous abstiendrons.

l'amendement de suppression de l'article 63 mais je pense qu'il s'est dit suffisamment de choses à cette tribune pour que ne soit pas nécessaire de développer longuement la nécessité de revenir sur cet article 63 qui exclut donc de du bénéfice de la prime d'activité Les de pension d'invalidité, les rentiers AT-MP, chacun a pu, à travers les arguments développés, je pense, se faire son idée sur l'aspect injuste de cette mesure qui est apparu, en tout cas aux membres de la commission des finances que vous avez dit favorable à cette délibération ensuite sur les les reprises de crédit sur l'autre programme qui nous permettent de financer cette mesure, j'ai j'ai détaillé l'importance des rendus de crédit près de 60 millions une année près de 70 millions l'année suivante, cette année, on peut supposer qu'il y aura des rendus de crédit de la même nature 6 mais en tout cas en or de grandeur et je pense qu'il y a pas d'il y a pas péril en effet à proposer cette reprise de crédit pour financer ces 20 millions que représente donc la fin de l'article 63. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté. Nous passons à l'amendement 225 défendue par monsieur le rapporteur de Merci Monsieur le Président, Madame la ministre, cet amendement vise à compenser la suppression des crédits issus de la dotation d'action parlementaire dite réserves parlementaire dont bénéficiait la mission Solidarité, en effet, on l'a déjà évoqué ces crédits n'ont été que partiellement compensée dans le coeur du projet de loi de finances pour 2018 sur les 147 millions d'euros ouvert au sud de la réserve parlementaire 61 millions d'euros étaient destinés aux associations par le biais de crédits ouverts sur la plupart des missions du budget général Sport, jeunesse, vie associative Solidarité, insertion, égalité des chances, cohésion des territoires etc l'abondement du fonds pour le développement de la vie associative, à hauteur de 25 millions d'euros par le biais d'un amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale sur la mission Sport, jeunesse et vie associative ne suffit donc pas à compenser les l'intégralité de la réserve par ailleurs le gouvernement n'a pas indiqué clairement quels seront les associations destinataires de ces crédits supplémentaires abondant le FDD DVA, indiquant seulement que ces crédits seront prioritairement destinés aux associations ne bénéficiant pas du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires, donc a priori des petites associations, sans faire injure à ces nationalisations, bien évidemment, dans ces conditions, cet amendement vise à majorer les crédits de la mission du montant des crédits-t-elle couvert, répartis en 2017 au titre de la réserve parlementaire, soit un montant de 6 1000000 662320 euros et nous proposons que ces crédits soient imputés de façon détaillée, je pense que vous avez le texte de l'amendement, je ne vais pas tous vous les citer mais on arrive au total indiqué de plus de 6 1000000 600000 euros, la non-compensation de ces crédits pour 2018, en effet, en difficulté, et cela a été dit tout à l'heure à plusieurs reprises, toutes les associations bénéficiaires de la réserve notamment les Restos du coeur avec près de 700000 euros, les banques alimentaires 200000 le Secours populaire, mais aussi l'APF, la Croix-Rouge, le mouvement du nid et d'autres afin de financer ces dépenses supplémentaires le présent amendement propose de réduire de 6 1000000 662320 euros, les crédits du programme 124 conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, etc en autorisations d'engagement et crédits de paiement, diminuant de 500000 euros l'action dysfonctionnements des services 412320 euros l'action 12 affaires immobilières de 500000 euros l'action 14 communications de 500000 euros l'action 15 affaires affaires internationales et européennes, et enfin de 750000 euros l'action 16 statistiques études et recherches Merci monsieur rapporteur et quel est l'avis du gouvernement. Monsieur le président, Mesdames et messieurs, je comprends la loi sur la confiance dans la vie politique, acte fondateur du quinquennat mis en effet fin à la réserve parlementaire toutefois pour répondre aux inquiétudes concernant les besoins des associations et nous entendons bien sûr, notamment les plus fragiles, vous l'avez rappelé le gouvernement a proposé d'abonder à hauteur de 25 millions d'euros supplémentaires, le fonds pour le développement de la vie associative, cet amendement au projet de loi de finances 2018 a été adoptée le 2 novembre dernier ces aides seront en effet fléchée sur les associations les plus petites, les plus fragiles ne disposant justement pas de salariés qui pourrait en être bénéficiaires seront une vraie aide pour elle, je pense que cette réponse vous satisfera que je souhaiterais donc vous retiriez votre amendement, faute de quoi ils seraient défavorables.

Oui merci monsieur le président, moi je avec moi, avec mon groupe, on pense que il s'agit pas de de faire un transfert et de d'essayer de prendre dans telle ou telle enveloppe pour amputés des crédits dompte l'émission ont besoin je pense par exemple à la mission égalité entre les femmes et les hommes, grande, grande, grande cause nationale, on va retirer pour essayer d'abonder effectivement une perte due aux associations, le gouvernement a fait un mauvais choix, il faut qu'il assume et c'est pas nous, au niveau du sénat de d'essayer de transférer finalement à moyen constant essayer finalement de déshabiller Paul pour habiller Jacques ou déshabillée Paulette pour habiller Jacqueline, donc on est contre cet amendement. Merci, cher collègue Monsieur Touraine pour explication. Oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être développé, c'est l'argument que j'ai moi-même exprimé il y a quelques instants, savoir que ça, ça n'a pas de sens, d'enlever à certains articles à certaines actions sociales des crédits pour les mettre sur une autre ce serait simplement avoir des des préférences qui seraient des préférences de sensibilité et ce que nous n'avons pas dans cette assemblée, mais il n'en reste pas moins. Que l'objectif qui est visé. Qui est de considérer que la réserve parlementaire qui n'est plus distribué et qui par conséquent pénalisent un certain nombre d'associations caritatives, puisque on a cité des chiffres tout à l'heure, elles en étaient attributaires pour des sommes très importantes, j'ajoute que ces associations voient aussi disparaître peut-être pas tout de suite, peut-être pas cette année parce qu'il y a eu des mesures transitoires, mais dans les années qui viennent, les emplois aidés par conséquent les seront doublement pénalisés, alors qu'elles remplissent une fonction essentielle essentielle dans notre pays en terme de lutte contre la pauvreté, d'aide à tous ceux qui sont marginalisés et qui sont en situation de vulnérabilité, par conséquent, je ne voterai pas ce un amendement qui est proposée pour les raisons que j'ai évoqué il y a quelques instants, mais je demande au gouvernement de rétablir d'une façon ou d'une autre les crédits qui étaient affectés au type de la réserve parlementaire et d'autres apporter une attention bienveillante parfaitement compréhensif à la situation des associations qui se voient privés des emplois aidés. Merci, cher collègue Monsieur qui aboutit presque vote. Oui merci monsieur le président moi je, je comprends ce qui vient d'être dit, de la part d'un certain nombre de collègues et j'approuve tout à fait le raisonnement du du rapporteur le le rabotage continue sur sur les mêmes postes qui sont des postes n'ont pas d'intervention mais des postes support c'est quelque chose qui a aussi effectivement ses limites, donc on arrive dans des choses qui sont pas complètement logique, c'est-à-dire que rétablir des fonds à un certain endroit, c'est très bien mais on regarde pas bien comme on les enlève, de l'autre, dans quelque chose qui risque d'être gênant à terme en termes de fonctionnement donc là la bonne solution, madame la ministre serait que effectivement vous plaît pour un effort supplémentaire sur les crédits qui ont été prévus à en en direction de du fonds associatifs, en direction des associations puisque on s'aperçoit aujourd'hui quand même que la suppression de la réserve parlementaire la réserve parlementaire n'était pas quelque chose qui était qui partaient comme ça dans la nature, on s'aperçoit concrètement des manques, elle, à la fois en direction des collectivités locales et du Milia ceci hâtif en est si on aide conciliant, essayer de trouver une solution, je ne suivrai pas totalement la Commission sur sur sa position de, de, de, de rabotage un petit peu, un petit peu aveugle qu'on peut parfois reprocher à un gouvernement, donc c'est pas à nous de le faire non plus, mais il faudrait que le gouvernement fasse un geste en direction du milieu associatif, parce que d'autres vous l'expliqueront aussi bien en voir mieux que moi, elle joue un rôle dans le lien social, de manière très importante au niveau des différentes associations auxquelles les uns et les autres, on peut penser. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur Bazin. Merci monsieur le président, le ministre, chers collègues, j'entends parfaitement le reproche qui peut être fait cette proposition, d'aller chercher des crédits ailleurs, on est bien obligé de le faire, c'est la règle, mais je vous fais observer que l'essentiel des reprises de crédit sont sur les affaires immobilières, plus de 4 millions 400 et que, on assiste à des rendus de crédit sur ses lignes de 60 à 70 millions d'euros, selon les années, donc je pense que la critique en l'occurrence, si elle est fondée en en intentions, elle ne laisse pas dans les fêtes, considérant donc les rangs du crédit qui ont eu lieu les années passées, donc je pense qu'on peut sans problème visés cet amendement et le voter je vous irons gage merci. Merci, cher collègue, Monsieur le Président ma gras. Merci monsieur le président, madame la Ministre, chers collègues. la suppression de la réserve parlementaire est quelque chose que je je n'arrive toujours pas à expliquer au Sénat tout le travail avait été fait pour cette réserve parlementaire soit parfaitement dans les règles, à titre personnel, j'ai toujours utilisé cette réserve parlementaire. Par le biais du ministère des Outre-Mer et au bénéfice exclusif les associations pour de l'événement, ciel c'était suivi les dossiers étaient contrôlés par le ministère, avant et après utilisation, donc je veux dire par là, je ne vois pas ce qu'on reproche à la réserve parlementaire, aujourd'hui nous sommes ce qu'on reprochait puisqu'elle est supprimée, aujourd'hui nous sommes en train de nous battre pour trouver des solutions alternatives de remplir, solution de remplacement qui serait confié sur des dotations qui serait confiée à des préfets pour attribuer à leur place, mais de quel droit un préfet a-t-il est-il plus compétents que les élus locaux pour attribuer dès réserve parlementaire au milieu associatif les solutions que nous apportons, je ne les trouve pas non plus satisfaisante, moi je suis très gêné par rapport à l'amendement et par rapport aux positions que nous faisons ce que je trouve qu'il est pas acceptable, c'est la démarche unilatérale du gouvernement qui pour moi est de l'amateurisme parce que c'est pas sérieux de faire ça, c'est plombé l'activité des parlementaires et je trouve ça inacceptable, on a une fonction, on est respectable, on l'accomplit normalement je ne comprendrais jamais pourquoi cette démarche et je tenais à le dire aussi sincèrement que je m'exprime, parce que la démarche, elle n'est pas bonne. Si chers collègues. Je n'ai plus de demandes d'explications de vote, je n'ai donc on voit l'amendement 225 de la commission des finances, qui a recueilli un avis défavorable du gouvernement qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient, il est adopté, nous passons à 2 amendements identiques. D'abord le 92, défendue par monsieur le rapporteur Moulinier oui. Oui Monsieur président mais Ministre donc cet amendement déjà été largement commentée dans les différentes prises de parole au monde la discussion générale, il vise à rien bondé de à Daegu tue 8 millions d'euros l'action 15 du programme 137 concernant l'égalité entre les femmes et les hommes d'une façon générale, la lutte contre la prostitution comme ça a été dit, la loi du 13 avril 2016 et juste mis en place et les différents outils et moyens sont se déroule, je dirais sur le territoire national et que nous voyons très naturellement arriver les premiers effets de cette, de cette mission, et donc de cette loi et je pense que c'est à Amman avait difficile de donner un signe de diminution des crédits alors même que nous espérons que l'effet bénéfique de la loi et l'arrestation des personnes qui sont aujourd'hui en situation donc donc difficile, hé bien puissent être accompagnés est aidé dans la réinsertion, c'est pourquoi nous proposons de revenir au crédit au niveau des crédits 2017 alors concernant la provenance de ces crédits, on est de nouveau dans le jeu des des transferts entre programme mais je veux purée je reprendrai pas le le l'argumentaire de notre rapporteur monsieur Baeza This piquant les disponibilités ou des possibilités à travers le programme notamment programme conduite et soutiennent des politiques sanitaires sociales du sport, de la jeunesse et la vie associative, notamment concernant tout volet immobilier je remercie. Merci, monsieur le rapporteur, un amendement identique le 172 défendue par Madame Meunier. Président, madame la ministre, et messieurs, chers collègues, c'est le même état d'esprit qui sous-tend cette amendement et qui représente donc un soutien sous 3 formes : 3 formes d'intervention une une forme pour l'aide aux associations qui sont de véritables partenaires de l'État en matière de prévention et de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, une autre forme, qui est le versement de l'allocation financière d'insertion sociale et professionnelle, ce que nous avions largement débattue ici au moment du vote de la loi et puis d'autres formes, qui sont des des crédits au service des comptes déconcentrés de l'État d'apporter un soutien à ces associations agréées, donc c'est Besson, on l'a dit, ces baisses cumulées qui représentent donc une somme d'un 1000000 8 ne ces baisses ne sont pas du tout comprise par le secteur associatif et comment les justifier, à l'heure où l'année prochaine sera donc la première année pleine de mise en oeuvre de cette donc les associations ne comprennent pas à à nouveau cette cette diminution et et nous soutenons comme cela a pu être dit au moment des débats dans la discussion générale, le maintien de ces crédits à haut niveau, tels qu'ils avaient été annoncés en 2017. Merci, cher collègue, et quel est l'avis de la commission des finances. Avis favorable, Monsieur le Président. Merci monsieur rapporteur et quel est l'avis du gouvernement.

voudrais vous rappeler que les crédits inscrits à l'action, 15 ont été calculés sur une progression graduelle du nombre annuel de bénéficiaires de la FIS entre 2018 et 2022 correspondant à la montée en charge de ce nouveau dispositif, en fonction d'une évaluation plus conforme au nombre réel de dossiers présentés à ce jour dans la la mise en 9 de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes en situation de prostitution, a été progressive sur l'année 2017, du fait des délais induits par la publication des textes réglementaires, la nécessité d'identifier l'ensemble des acteurs locaux pour installer les commissions départementales et d'agréer les associations chargées du parcours de sortie de la prostitution au 30 novembre 2017 24 demandes d'entrer dans le parcours ont reçu un avis favorable de commissions départementales et plus d'une vingtaine de dossiers devraient être examinés avant la fin de l'année, la dynamique qui s'est enclenchée va désormais se traduire dans la montée en charge du dispositif, la programmation budgétaire tient compte de cette trajectoire avec 2 4 millions c'est 600 parcours qui pourront être financées sur une année complète donc pour cette raison, je suis défavorable à cet amendement. Merci madame la ministre madame Ben Basat pour explication de vote. Monsieur le président, comme les auteurs des amendements viennent de le dire, justement, les crédits alloués à la prévention et à la lutte contre la prostitution et la traite des être humains qui s'élève aujourd'hui à 5 millions d'euros sont en forte baisse par rapport à 2017 mois 26,7 or cette argent est notamment destinée à financer le parcours de sortie de la prostitution, ce dispositif, mis en avant lors de l'examen par le parlement de la loi de lutte contre le système prostitutionnel devait contrebalancer l'inéluctable mise en danger des personnes prostituées induite par la pénalisation des clients que je me suis attaché à combattre sur ces bancs, on nous annonçait la fin des problèmes de violence envers les personnes prostituées la fin des problèmes sanitaires dus à l'isolement et à la précarisation puisqu'elle se verrait proposer des aides financières à la réinsertion sociale et professionnelle et pour être enfin trouver un véritable emploi, la pénalisation des clients a déjà montré ses effets pervers, les observations de la mission France de Médecins du monde sont de ce point de vue en revanche, le parcours de sortie n'a été mis en place, Cannes, avril 2017 madame Schiappa ayant elle-même indiqué qu'au 1er novembre le sol 5 personnes en avaient bénéficié, la baisse de ses crédits pour 2018 aura pour conséquence très concrète d'abandonner un peu plus les personnes prostituées qui voient leurs conditions de travail et de santé considérablement aggravée l'ironie de cette situation quand on prétend faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité pourrait prêter à sourire, malheureusement, la situation de précarité de grand danger dans laquelle se trouvent ces personnes nous oblige au contraire à faire preuve de la plus grande gravité merci. Merci Monsieur Président oui, madame la ministre, je vous ai entendu et j'ai écouté également les débats alors lors de lorsqu'ils ont eu lieu à l'Assemblée nationale et cette question de sortie de la prostitution et de l'accompagnement au parcours de sortie, comme vous l'avez dit être en en puissance en montée et donc je trouve que le signal donné est vraiment très regrettable puisqu'au moment de la discussion de ce texte, c'était vraiment un des piliers, hein, de lutter contre le système prostitutionnel de lutter contre les réseaux de pénaliser les clients mais aussi d'accompagner les personnes prostituées vers la sortie de la prostitution et je trouve très regrettable que cette diminution de crédit ne puisse pas permettre à la loi de d'exercer d'exercer de vivre et d'être pleinement soutenus, donc je maintiens mon amendement. Merci, cher collègue Madame Cohen pour l'explication de vote. bien merci Monsieur le le président je, je pense qu'il y a quand même un paradoxe dans l'attitude du gouvernement, c'est-à-dire on a entendu une prise de conscience, visiblement au plus haut de l'État, samedi 25 novembre lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, or la prostitution est une violence extrême exercée à l'encontre des femmes et le gouvernement bien diminuent les Les les crédits qui sont destinés à l'accompagnement des personnes qui souhaitent sortir de ce système prostitutionnel, donc nous nous sommes battus au niveau de de notre groupe. Pour la la d'options de de cette, de cette loi et nous ne comprenons pas aujourd'hui que le gouvernement finalement par c'était Titudes va empêcher l'application pleine et entière de la loi, on est là dans quelque chose de l'or de la prévention et donc je, moi je, je, j'appelle à nouveau, comme plusieurs de mes collègues le gouvernement à réfléchir notamment Madame Schiappa mais aussi le président de la République parce que effectivement les discours sont importants mais, au-delà des discours, il faut des moyens pour mettre en application la lutte contre les violences faites aux femmes qui, qui constituent un véritable fléau, donc voilà, après ce qui consiste un peu à essayer de d'aménager des erreurs du ou des manques du gouvernement sur des enveloppes qui sont en quelque part des enveloppes fermées, ça ne règle pas le problème, c'est pourquoi nous nous abstiendrons. Si chers collègues, je n'ai donc on voit ces 2 amendements identiques qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission des finances, et d'un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient ils sont adoptés, nous allons procéder au vote des crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, figurant à l'État B. je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite je mets où voit les crédits de la mission. Qui s'abstient.

et 64 et les amendements qui sont rattachés pour leur examen au crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. Merci monsieur le président, la vie, ce sera très rapide, puisqu'on a, on vient d'avoir le débat donc avec le 205, il s'agit maintenant de supprimer l'article 63 pour que les personnes titulaires de pensions d'invalidité ou de rente AT-MP puissent bénéficier de la prime d'activité : avis favorable de la commission des finances. Merci, monsieur le rapporteur, 208 est identique et défendu par Monsieur Touraine. Il est défendu. Si chers collègues. Le 226 rectifier également identique Madame Dindar il défendu. Merci, cher collègue. l'avis du gouvernement, puisque la commission la présenter. et de rentes accidents du travail, maladies professionnelles à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité, je rappelle que cette dérogation a été inséré par la loi travail du 8 août 2016 postérieurement à la mise en place de la prime à n'est pas complètement cohérente avec l'esprit de la prime d'activité, la prime d'activité en effet bien pour objectif et seul objectif d'inciter les bénéficiaires augmenter les revenus tirés de leur activité, or ni les rentes AT-MP ni les pensions d'invalidité ne sont des revenus en lien Direct avec l'activité du bénéficiaire, ce sont des prestations sociales et des revenus de remplacement, elles n'ont pas vocation à être assimilés à des revenus d'activité pour le calcul de la prime, le gouvernement propose donc de revenir à la logique initiale de la prime, j'ajoute que l'impact est limité, moins de 10 1000 foyers 9358 pour être précis, ont bénéficié de cette disposition sur 2 1000000 580000 foyers de bénéficiaires par ailleurs la dérogation de calcul est en revanche maintenue pour l'allocation adulte handicapé dans les mêmes conditions qu'actuellement, puisqu'il s'agit d'un minimum social, versé sous condition de ressources en 2016 66000 foyers ont bénéficié à la fois de lâche et de la prime d'activité, aucune modification n'interviendra Pologne le renvoie un décret, et non plus à la loi pour fixer le seuil est purement formelle, ce seuil n'a pas vocation à évoluer pour toutes ces raisons je suis défavorable à cet amendement. Merci madame la Ministre je mets donc on voit ces 3 amendements identiques avec un avis défavorable du gouvernement, un avis favorable de la commission, le même amendement qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient ils sont adoptés par voie de conséquence, l'article 63 et supprimer je mais on voit l'article 64 qui est pour. qui est pour. Il est adopté, j'appelle en discussion les amendements tendant à insérer des articles additionnels qui sont rattachés pour leur examen au crédit d'émission Solidarité, insertion et égalité des chances. Après l'article 64 l'amendement 147 rectifier Madame Mehdi. Si Monsieur le Président, Madame la ministre. L'application de gestion des dossiers de ressortir sans étrangers en France, régie par les articles R. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le système d'informatique qui permet la tenue des dossiers individuels des étrangers par les préfectures et la production des autorisations et titre de séjour

le système permet de rendre disponible au service de police, de gendarmerie et des douanes, un processus de contrôle avec consultation automatique du système d'information Schengen et authentification biométrique des voyageurs ainsi que de contribuer à l'identification des personnes en situation irrégulière depuis 2013, certains agents des services fiscaux ont accès à la GDR F. ainsi qu'au traitement VISA bio l'évaluation sociale de la minorité et de l'isolement de jeunes se déclarant mineurs non accompagnés, actuellement à la charge des départements pourrait être facilitée par la mise en place des mêmes disponibilités pour certains agents du service du service de l'aide sociale à l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités, il s'agirait ainsi d'avis comme cela peut-être le cas aujourd'hui, que des étrangers majeurs qui ont fait une demande de VISA ou auxquels on a refusé un titre de séjour régulier s'adressent aux services de protection de l'enfance, en se déclarant mineurs non accompagnés, dans la mesure où l'accès à ces fichiers doivent être scrupuleusement réglementée, il conviendrait que les services de l'État évalue, dans quelles conditions et selon quelles modalités pourraient être ajoutés à la liste des bénéficiaires d'un accès en consultation de ces fichiers, certains agents des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance. Merci, cher collègue, quel est l'avis de la commission. Monsieur le Président, Madame la Ministre des chers collègues, nous avons tous souligné à tour de Roland de la discussion générale. La dramatique actualité de l'augmentation du nombre de mineurs étrangers isolés ou appeler maintenant mineurs non accompagnés, ce que j'ai un peu de mal à faire pour mon compte parce que ces mineurs sont parfaitement accompagné jusqu'à nos services sociaux puisque les filières qui les amène, assure un service complet jusqu'à, jusqu'à nos services à nous, ce qui n'est pas étonnant vu les tarifs qui sont pratiqués par ces mêmes filières puisque on sait que l'arrivée en France est tarifé 4000 à 7000 euros selon les pays d'origine, donc ce problème est un problème que nous dénonçons, nous dénoncions quand j'étais présidente département avec l'Assemblée des départements de France depuis plus de 3 ans nous avons averti tous les ministres de la Justice successifs sur le caractère exponentiel du phénomène qui va continuer puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets que nous accueillons évidemment selon nos règles et nos lois, ces mineurs étrangers isolés comme il se doit et que le marché évidemment fonctionne est parfaitement rentable pour filières le 1er ministre donc quand il est venu au congrès de l'Assemblée des départements de France à Marseille au mois d'octobre, a annoncé plusieurs choses intéressantes et forte, il faut le reconnaître, la 1ère c'est que c'était à l'État de prendre en charge la mission de premières accueil et l'évaluation de ces mineurs et qu'ensuite. Pour ceux qui sont reconnus mineurs car nombre d'entre eux ne le sont pas sur ceux qui sont reconnus mineurs doivent être accueillis au type de l'aide sociale en France par les départements, ce que les départements ne conteste pas, à ce jour, même s'il s'inquiète quand même de la masse d'enfants qui vont avoir à accueillir, dans ces conditions, aux premières annonces fortes du 1er ministre la prise en compte du premier accueil et la prise en compte de l'évaluation elles-mêmes qui sont actuellement très mal prise en compte, puisque c'est à hauteur de 5 journées à 250 euros la journée, on est très très loin du compte de ce que cela coûte au département, deuxièmement, il a été décidé une mission partagée entre l'Assemblée des départements de France et les services de l'État pour rendre compte de propositions en diagnostic d'abord partagé et ensuite des propositions pour que chacun prenne sa part sa juste part entre l'État et les départements de cette mission qui reste évidemment incontesté dans ces conditions, comme la mission doit rendre ses conclusions pour le 15 décembre, me semble-t-il, je vous demande ma chère collègue de bien vouloir retirer votre amendement ce rapport arriverait bien après les conclusions de cette mission, merci. Merci, monsieur le rapporteur, quel est l'avis du gouvernement. J'ai le même avis que monsieur le rapporteur si vous retirez votre amendement, compte tenu du rapport qui arrive, merci.

défendu, je ne sais pas, parce que finalement j'ai déjà des réponses qui viennent d'être donnés un amendement qui portait sur la volonté d'avoir une visibilité et une évaluation parfaite de la question des mineurs accompagnés comme ça a été dit, on est dans une situation qui est fortement exponentielle avec de plus en plus de mineurs concernés avec des départements qui doit faire face à une situation je dirais particulièrement tendue et et malheureusement il faut-il trouver des bonnes réponses, donc nous avions ici souhaité proposer un amendement qui permettait de lancer un rapport d'information qui nous aurait donné plus de visibilité, mais vous avez à l'instant même donner des éléments de réponse et donc nous retirons cet amendement. Et chers collègues, je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 18 heures 30 pour l'examen de la mission défense la séance est suspendue.

La séance est reprise, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances adoptées par l'Assemblée nationale pour 2018 : nous poursuivons l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances des différentes missions : le Sénat va examiner les crédits de la mission défense,

Monsieur le Président Madame. La ministre, le président de la commission des finances, monsieur le président de la commission de la Défense et des Affaires étrangères mais chers collègues permettez-moi de m'abstraire tels que l'instant d'une approche purement comptable du budget 2018 pour le remettre en perspective un quinquennat vient de s'achever avec sa loi de programmation militaire un nos débuts qui nous seront dans quelque temps, d'une nouvelle LPM, quel bilan tirer de ces 5 dernières années une LPM 2014, 2019 qui réduisait les moyens financiers et humains alloués par rapport à la précédente LPM, qui elle-même avait été. Initiée avec une forte réduction des effectifs et engage vers une profonde restructuration de notre dispositif de défense dans le même temps, une mobilisation sans précédent de nos forces, tant par le nombre d'opérations extérieures que par leur intensité et longue durée aujourd'hui, nous sommes engagés au Sahel, où le vent dans des opérations de sécurité qui mobilise l'ensemble de nos dispositifs aériens terrien et sur mer, sans compter le territoire national, tout ceci, bien au-delà du format d'engagement initialement prévu, chacun sait ici que malgré tous les efforts et l'habileté et la détermination de votre prédécesseur, sans compter son art de la communication, les infections qui ont été données ont été très en deçà des besoins. En renvoyant la résolution des problèmes à plus tard, c'est-à-dire au prochain quinquennat et à une prochaine LPM vous héritez madame la ministre, de cette situation doublement préoccupante préoccupante sur le plan de nos forces, la régénération des matériels n'est pas assuré le maintien en condition opérationnelle des hommes et des matériels est compromis par une suractivité qui n'est pas compatible avec l'entraînement des personnels et, d'autre part, l'entretien les conditions matérielles de nos soldats sont insatisfaisantes et l'état de notre Patrimoine immobilier dans lequel ils évoluent et déplorable expliquant largement les difficultés de fidélisation. Préoccupante aussi à la situation sur l'état de la menace, nous vivons dans un monde de plus en plus dangereuses, l'objectif d'attente de 2 pourcent du PIB en 2025 doit être appréciée à l'autre d'une réalité inquiétante, les dépenses militaires mondiales représentent aujourd'hui du PIB mondial, le budget militaire de la Chine est 4 fois supérieur au nôtre et les États-Unis envisagent d'augmenter le leur de 54 milliards de dollars pour avoisiner les 700, jamais on a vendu autant d'armes dans le monde, peu de pays vivent vraiment en paix, la menace est diffusée sur notre sol les modes opératoires de nos adversaires et leur détermination ne nous permettent plus de différer nos décisions, on ne peut plus demander toujours plus à nos armées pour protéger les citoyens face à une insécurité accrue sans leur donner les moyens de cette exigence, c'est au cours de ce quinquennat madame la ministre de la prochaine loi de programmation militaire que tout se joue cette situation, vous la connaissez et je veux saluer ici votre détermination qui se traduit par quelques avancées dans le budget 2018, d'abord à l'effort de sincérité du budget avec une provision, hop exporter de 450 millions 650 même si la dépense finale devrait dépasser le milliard une majoration significative de 1 milliard de des crédits d'équipement avec un effort particulier sur l'entretien programmé des matériels et les infrastructures, je veux également saluer le plan famille qui constitue le début d'une réponse à la question de la fidélisation du personnel et l'amorce d'une revalorisation de la condition militaire, ces évolutions sont les bienvenus mais quelles perspectives nous propose-t-on à moyen terme, soit une augmentation, soit un budget de 50 milliards à cette échéance, hors pensions pour atteindre cet objectif, il faudrait une majoration annuelle régulière de 2 milliards 25 par an pendant 8 ans on vous nous proposez un virgule 8 cette année et 1,7 jusqu'en 2020, 2 pour atteindre 40 milliards à cette date, c'est donc un effort de 2 milliards qui devraient porter sur les 3 années suivantes, soit le double de celui réalisé dans la période précédente, je ne puis que déplorer une fois encore ce renvoi de l'effort à plus tard au prochain quinquennat pour 2018 les crédits passerait de 30 2 milliards 4 à 34 2 soit 1,8 de crédits supplémentaires, je salue cette avancée mais doit être relativisée au regard de 850 millions de crédits purement et simplement annulée annulée en juillet dernier, par ailleurs, si la majoration de 100 millions de la provision pour OPEX constitue un élément positif participant d'une amélioration de la sincérité budgétaire, elle ne constitue pas pour autant une augmentation des moyens. L'effort réel et donc plus près de 800 millions que d'1 milliard 8 il est insuffisant, mais notre commission a voulu retenir pour ce 1er budget du quinquennat et dans l'attente des précisions qui ne manqueront pas de venir à la faveur de la prochaine LPM, nous avons voulu retenir ses bonnes orientations c'est le sens de son avis positif toutefois: il est assorti d'une réserve, je veux parler de la fin de gestion 2017 car la sincérité du budget 2018 et son caractère opérationnel en dépendent très largement de points ont retenu l'attention de notre commission le surcoût OPEX, estimée à 350 millions pour lequel nous avons reçu l'assurance qu'ils seraient pris en charge par la solidarité inter- ministériel, dont acte, l'autre point et le gel de 700 millions de crédits du 1017 qui ne sont toujours pas débloqué à l'heure où nous sommes, nous savons que malgré vos relances sur le sort qui leur sera réservé, Bercy est aux abonnés absents, je ne peux pas croire, nous ne pouvons pas croire qu'à un mois de la clôture budgétaires, Bercy n'est pas une idée des arbitrages qui seront rendus, le fait que le ministre en charge des comptes publics rende sa sentence après le vote du budget est inacceptable et ne peut que nous inquiéter, si l'on se souvient de la manière dont a été brutalement annoncé en juillet la suppression de 850 millions le vent du Nouveau Monde, visiblement, ne souffrent pas sur Bercy qui continuent à recourir avait passe passe budgétaire qui nous conduisent dans des impasses et pourtant il s'agit de notre sécurité et de la vie de nos militaires aussi, Madame la Ministre, sauf si vous pouvez, dans quelques instants nous annoncer une bonne nouvelle, nous ne pourrons pas voter votre budget,

Nous nous abstiendrons à regret par ce vote, nous voulons vous accompagnez, Madame la Ministre dans votre détermination à obtenir les crédits nécessaires à nos armées exprimé à nos militaires notre refus de poursuivre les errements du passé qui constitue à reporter à plus tard les décisions des certes à l'exercice de leur mission, je vous remercie.

et ceci pour 3 minutes, veuillez respecter le délai si nous voulons terminer la séance à des heures acceptable. Monsieur le Président, Madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, le budget de la Défense pour 2018 : est-il vraiment un budget de remontée en puissance des moyens des armées, la ministre où l'avait affirmé à plusieurs reprises ces derniers temps, certes tous les indicateurs sont orientés à la hausse des effectifs, les investissements, les équipements, mais il y a aussi un effet de trompe l'oeil car 90 pourcent de l'augmentation prévue est d'ores et déjà consommé bien sûr par rapport à la prévision initiale de 2017 pour 2017 la mission défense et doté de 1,7 milliards d'euros supplémentaires, mais cette hausse est absorbée pour 420 millions d'euros par le report des charges ni de mesures que vous avez dû prendre la ministre en juillet dernier par 200 millions d'euros de Reso budgétaire de surcoût de OPEX et par un milliard d'euros pour le financement des mesures arrêtées en 2016, c'est-à-dire en dehors de la loi de programmation militaire, on peut donc parler de stabilisation des moyens mais il est difficile de trouver un réel accroissement d'ailleurs la trajectoire prévue pour 2000 19 et 2020 reste en deçà des besoins militaires que nous avions évalué nous à 2 milliards d'euros par an, l'augmentation annuelle nette ne serait que de 1,5 milliard car j'ai déduit la poursuite du recyclage des OPEX. Et justement de ces obsèques, j'aimerais dire quelques mots, les surcoûts d'OPEX, ne sont pas une ligne, comme les autres dans le budget de la défense, ce ne sont pas des, ce ne sont pas les armées qui décident de leur engagement, c'est le président de la République d'abord et le Parlement, ensuite, c'est le principe de solidarité, de la solidarité, prévu par la loi de programmation actuelle militaire actuelle pour financer les surcoûts en rapatriant ces surcoûts dans la mission défense, le gouvernement ne fait que transférer la charge au détriment du ministère des Armées, il ne faudrait pas que cette nouvelle orientation conduisent à faire financer les surcoûts nette d'OPEX par des crédits destinés initialement à l'équipement des forces, c'est malheureusement la traditionnelle variable d'ajustement budgétaire, comme l'a bien montré encore à l'annulation de 850 millions d'euros cette année, ce schéma reviendrait en effet à déployer nos militaires en OPEX, tout en diminuant leurs moyens d'action afin précisément de financer leur mission, autant dire que ce serait une aberration avec de graves conséquences pour notre outil de défense à plus court terme, nous sommes préoccupés, au plus haut point par les 700 millions d'euros de crédits pour 2017 encore gelés par Bercy pour le programme 146 la DGA la cette cela empêcherait évidemment la DGA d'assurer la poursuite normale des programmes d'armement et c'est le risque pour le budget de la défense d'aggraver encore et ça a été dit à l'instant un report de charges qui pourraient atteindre un niveau historiquement élevé de plus de 3,5 milliards d'euros comment voter le budget de l'année prochaine sous une telle menace, en l'absence de dégel des 700 millions d'euros, c'est le programme 146 d'équipement des forces qui financerait alors les OPEX, j'espère, Madame la Ministre, que toute l'énergie que vous déployez à convaincre Matignon de débloquer ces sommes portera ses fruits et que dans l'intérêt de nos militaires vous y parviendrez mais dans ces conditions, et principalement, compte tenu de l'absence de dégel notre commission en responsabilité, a décidé de s'abstenir sur le vote des crédits de la mission défense. la parole est à madame Hélène Conway Mouret, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées pour le programme d'équipement des forces pour 3 minutes chers collègues.

Madame la Ministre, Monsieur le Président et monsieur le rapporteur général chers collègues. Ce débat budgétaire est un moment de vérité pour nos armées pour le Parlement et pour les Français que les enjeux de sécurité préoccupent aujourd'hui puisque jamais madame la ministre, nous nous réjouissons de la tenace IT avec laquelle vous défendez votre budget c'était gare vous inscrivez dans les pas de votre prédécesseur et je puis vous assurer ici que la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées et, plus largement, le Sénat, de même qu'ils ont soutenu les efforts de Jean-Yves Le Drian, pour consolider la trajectoire financière et capacitaire de la loi de programmation militaire en vigueur sont eux à vos côtés pour la bonne préparation de la prochaine LPM, l'état d'esprit dans lequel nous travaillons résolument en positif au service de la défense nationale et dans l'accompagnement de vos efforts, nous sommes également attaché à une certaine éthique de la responsabilité politique et à ce titre, nous veillons à ce que les réalités soit bien conforme au discours de ce poids ne vu je dois vous dire notre inquiétude quant au décalage qui semble s'instaurer entre d'une part et prometteuse annonce de remontée en puissance des moyens militaires et d'autre part la froide vérité des chiffres, alors qu'il est utile de restaurer les moyens nécessaires pour nos armées dans le contexte de menace accrue que vient de décrire la revue stratégique et qu'il importe de soutenir au mieux notre base industrielle et technologique de défense, je constate que c'est année 850 millions d'euros ont été annulés sur la mission défense pris sur le programme 146 et que l'on s'attend par ailleurs un report de charges d'au moins 3,5 milliards d'euros, on attend toujours, enfin le dégel de 700 millions d'euros, sans lesquels la DGA ne peut pas conduire ses programmes d'armement l'année prochaine la hausse budgétaire inscrite dans le projet de loi de finances sera largement absorbés, si l'on considère l'aggravation du report de charges, l'Euro se place des OPEX et les décisions hors LPM à financer, alors que le reste à payer de la Défense excède déjà 50 milliards d'euros, dont plus de 35 milliards pour le programme de 146 dans quelles conditions de soutenabilité l'entrée dans la gestion de la future LPM pourra-t-elle se réaliser, d'autant que les investissements à conduire dans les prochaines années seront lourds pour la dissuasion, comme pour les forces conventionnelles, la programmation envisagée par le gouvernement reporterait à la prochaine législature et concentreraient sur 3 années de 2023 2025, plus de la moitié de l'effort à accomplir pour atteindre un budget de la Défense, représentant 2 pourcent du PIB suivant l'engagement du président de la République lors de la campagne présidentielle pareille trajectoire est-elle vraiment crédible nous appuierons, Madame la Ministre, toute initiative qui aurait pour effet de nous rassurer, ainsi que l'ensemble des acteurs de cette politique de défense pour l'heure, nous sommes encore dans l'expectative, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole. Jean-Marie Bockel, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées pour le programme de préparation et emploi des forces savait 3 minutes monsieur rapporte. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le programme 178 qui constituent le coeur de la mission défense voit ses crédits de paiement, augmenté de 10,6 pourcent par rapport à 2017 pour s'établir à 8,4 milliards d'euros l'année 2018 marquera le début du Reso clash budgétaire annoncées des surcoûts des OPEX, pour 125 millions d'euros sur le programme 178 ceci a induit de fait, le basculement du financement des OPEX, de l'interministériel vers les armées qui se poursuivra sur la prochaine programmation, une telle évolution, si elle améliore la sincérité du budget diminue aussi la remontée en puissance des mois il y a des armées notre souhait aurait été d'augmenter l'enveloppe budgétaire à due proportion la location de 450 millions d'euros supplémentaires en faveur de l'entretien programmé du matériel en 2018 mois l'effort nécessaire au vu des besoins immenses et doit impérativement être poursuivi dans la prochaine loi de programmation. Si l'exportation de nos armements permet de maintenir la base industrielle de défense nécessaire à notre souveraineté, il conviendra de prévoir dans la prochaine loi de programmation, contrairement à la précédente, les crédits nécessaires au financement du soutien à l'exportation sous-texte par les armées et la modulation à la baisse des coûts des élus de l'entretien programmé des matériels supportée par l'armée, une fois les objectifs d'exportation des industriels atteint les armées n'ont guère toucher les bénéfices des 14 à 17 milliards d'exportation de ces dernières années, pourtant soutenus par leurs performances au combat, la prochaine loi de programmation militaire ne doit pas faire l'économie d'une profonde réflexion sur ces enjeux, sous réserve de ces remarques notre commission a adopté les crédits du programme 178 comme le dira tout à l'heure, Olivier Siou le petit pour le groupe UDI, nous irons à l'instar de ce qu'a dit le le rapporteur de la commission des finances et de ce que nous avons évoqué, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, la défense lors de notre dernière réunion, nous associons à plusieurs des des groupes qui considère que nous devons être madame la ministre, dans une abstention de soutien à votre engagement de l'occasion d'ailleurs différents porteurs de vous rencontrer d'évoquer cette question avec vous par le passé, la commission, que ce soit à l'époque où Monsieur Raffarin la présidé cher est cher est encore bon que ce soit Jean-Luc Carrère avant a eu à plusieurs reprises dans des moments difficiles, une attitude de soutien du ministre aujourd'hui de la ministre, donc nous sommes évidemment dans un état d'esprit très très très positif à votre égard à l'égard de nos armées qui sont engagés, mais je ne répète pas ce qui a été dit ce sera répétée alors aujourd'hui les je pense que le meilleur service reporter votre combat, c'est d'être dans cette abstention positive. Merci, Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Christine Pruneau, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées pour le programme de préparation et employes des forces pour 3 minutes.

aux objectifs fixés de près de 10 pourcent l'amélioration attendue de la mise en place d'un régime d'entraînement différencié tarde à se concrétiser, la Commission le déplore et s'inquiète à ce sujet, autre point de vigilance, la trop lente remontée de la disponibilité. Technique opérationnel des Thilo la par exemple, des hélicoptères de l'armée de terre permet de remplir que 58 à 66 pourcent du contrat opérationnel la au des équipements de l'armée de terre est à la peine, tout comme celle des équipements aéronautiques, il faut poursuivent les efforts rigoureux trop tardivement entrepris pour soutenir la lente amélioration des résultats, l'externalisation également complète du MCO ne semble pas. La bonne solution, enfin, la Commission s'inquiète de l'état des services de soutien éternel sacrifié, subissant de plein fouet les réductions de personnel, il est impératif de suspendre Madame la ministre, la déflation des effectifs du service du commissariat des armées et du service de santé des armées notre visite avec mon collègue Jean-Marie Bockel auprès du ça a vraiment montré que les personnels sont sur sollicités mais complètement à la disposition des blessés et des blessés et et vraiment défendu leur point d'énormes valeur sur leur travail, mais ils sont au bord du Bernard c'est peut-être trop exagéré mais on les sent vraiment extrêmes limites, ce qui était une grande force française au déploiement en opération est aujourd'hui, apparemment sans trop exagérer un talon d'Achille qui ne tient que par le dévouement des personnels, c'est notre sentiment, donc il est urgent et indispensable de placer les services de soutien au coeur de la réflexion de la prochaine loi de programmation militaire pour éviter justement l'érosion de la capacité de de projection de nous armer Madame je remercie. Merci madame la rapporteure, la parole est à monsieur Joël E rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées pour le programme de soutien de la politique de défense et pour 3 minutes. Madame la Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, les crédits de titres de inscrit au programme de 212. Qui regroupe l'ensemble des crédits du personnel du ministère de la défense s'établissent donc pour 2018 à 20 milliards Wielun. 37 2 roues en n'augmentation de 3,24 pourcent par rapport à 2017 cette augmentation continue de la masse salariale traduit plusieurs évolutions dont nous nous félicitons, il en est ainsi de la poursuite de la hausse des effectifs plus 518 emplois équivalents temps plein qui accentue dans un sens favorable la trajectoire, approuvé par le Conseil de défense du 6 avril 2016 au bénéfice, cela a été dit cela a été dit la sécurité du territoire de la cyberdéfense des services de renseignement et de la protection des emprises. Militaire je note également la progression de. 50,8 millions d'euros des crédits destinés aux réserves ainsi que la hausse de 75 millions d'euros de l'enveloppe de titre 2 destinées aux OPEX dans un effort de sa série station Duroc budget des armées, même s'il faut souligner qu'il s'agit là en quelque sorte d'un transfert de la solidarité. Car ministériel un financement par le budget de la défense, comme d'autres collègues l'ont dit à l'instant, pour autant, ce projet de budget appel à mon sens, 3 mises en garde en 1er lieu la baisse des crédits moins 35 millions d'euros destinés à l'accompagnement des restructurations au financement des aides au départ. Si elle est justifiée par l'arrêt des déflation ne le doit pas pour autant occulter la poursuite du processus de transformation de l'armée et la nécessité d'accompagner cette démarche, deuxièmement en ce qui concerne le volet rémunération des militaires, les militaires ont fait part pâtiront en 2018, comme l'ensemble des agents publics de la suspension du protocole parcours professionnel carrières et rémunérations alors même qu'ils aient. Entrée dans le dispositif avec un an de retard. Par rapport à la fonction publique, nous serons vigilants à ce que cette mesure d'économie qui vise cette année à financer une indemnité compensant la hausse de la CSG ne se prononce pas au-delà de 2018, naturellement nous ferons aussi attentif aux effets que pourrait avoir sur les rémunérations des militaires, le chantier de la simplification des primes engagée par le ministère, ainsi que le basculement de Louvois vers le nouveau système de paye enfin enfin dernier point d'attention dont il ne faudrait d'ailleurs pas occulter les effets potentiels sur la masse salariale, la transposition de la directive européenne sur le temps de travail, il faut l'admettre l'encadrement du temps de travail. Paraît difficilement compatibles avec les spécificités du statut militaire et notamment le principe de libre disposition de la force armée, cette idée et même. Contradiction tout. Total avec l'obligation de disponibilité et l'esprit d'engagement qui caractérise le métier des armes, alors que l'échéance pour transposer la directive approche. La commission des Affaires étrangères, sous l'impulsion de notre président. S'inquiètent légitimement de cette perspective, pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, comment évolue ce dossier et quel dénouement vous entre nous espérons en tout cas une solution réaliste et ne mettant pas en cause les fondements de la fonction militaire sera trouvée prochainement mais nous savons que vous pouvez nous pouvons compter sur votre détermination et je me sens merci. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Gilbert Roger, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées pour le programme de soutien de la politique de défense pour 3 minutes. Madame la Ministre, Monsieur le Président mais chers collègues en Express le programme 212 regroupe aussi les crédits de personnel du ministère, les moyens transversaux de soutien de la politique de défense, ces moyens connaissent une augmentation significative, environ 20 pourcent principalement liée aux besoins de la politique immobilière dont les crédits augmentent cet Euro c'est bienvenu, elle était même urgente alors que nous n'avons cessé de souligner, année après année la dégradation préoccupante de l'état du Patrimoine immobilier de la Défense et ses effets sur les conditions de vie et le moral des militaires, ça a été rappelé à l'instant, nous restons vigilants sur plusieurs points en 1er lieu l'augmentation des crédits immobiliers ne doit pas permettent ne permettra pas en réalité le qu'un début de rattrapage en effet les besoins sont estimés à environ à 2,5 milliards d'euros pour les 6 prochaines années, nous serons aussi attentif à ce que l'augmentation soit 7 fois inscrite dans la durée sans déformation de l'effort en exécution au profit d'autres priorités, seul un effort soutenu et persistant permettra réellement de changer de cap en 2ème lieu s'agissant des recettes de cessions immobilières, vous le savez, madame la ministre, il y a la loi Duflot qui entraîne aujourd'hui d'importantes moins-values pour la défense, près de 25 millions d'euros en 2 ans peut-être 50 millions supplémentaires avec la vente de la partie centrale de l'îlot Saint-Germain et la défense a obtenu en contrepartie ce qui nous paraît inadmissible la réservation de seulement 50 logements sociaux sur les 250 alors que nous savons qu'il manque 400 logements au moins pour les militaires, en région parisienne, quant à la vente du bâtiment de l'Epita le Val-de-Grâce, ne serait-il pas plus sage, en tout cas c'est notre avis madame la ministre dit renoncer afin d'assurer la à la Défense, le maintien de surface immobilière conséquentes à l'intérieur de Paris Source solde, vous le savez, on en parle souvent, doit succéder à partir de 2018 à Louvois, le logiciel Louvois, on nous dit serait sous contrôle, raison de plus pour ne pas basculer vers son successeur qu'avec la plus grande prudence est le plus grand discernement gardons en mémoire le désastre financier et humain que fut Louvois et pour toutes les régions qui ont tenté, annoncés par nos collègues en particulier les 750 millions qui manquent, nous proposons l'abstention, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Pascal Alizart, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées pour le programme environnement et prospective de la politique de défense pour 3 minutes chers collègues. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le programme 144 environnement et prospective de la politique de défense avec 1,4 milliards d'euros pour 2018 ne représente en fait que 3 pourcent des crédits de la mission défense cependant il constitue le coeur de la préparation de l'avenir de notre outil de défense, une fonction cruciale depuis 2014, le budget annuel moyen des études amont 727 millions d'euros s'avère en ligne avec l'objectif fixé en la matière par la loi de programmation militaire, c'était 730 mais ce budget est insuffisant pour l'avenir aussi nous soutenons votre ambition Madame la ministre, d'amener ce budget dans la prochaine LPM à hauteur d'un milliard d'euros en moyenne et nous y veillons, la France est aujourd'hui le pays d'Europe qui consacrent le plus gros effort budgétaire à sa recherche et développement, défense, il faut qu'elle le reste et à cet égard je salue la récente création d'EDF Invest, fonds avait qui, statistiquement, pour soutenir le développement des PME stratégiques pour la défense, dans ce contexte positif, nous restons préoccupés par la situation de l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, la situation s'améliore mais avec lenteur, la gouvernance se trouve à présent entièrement refonder un plan général de rénovation est nécessaire pour maintenir au meilleur niveau les souffleries de l'honneur après une pièce pardon maîtresse de nos grands moyens technologiques, d'autre part, il faut organiser la rationalisation des implantations francilienne de l'établissement, dans ces 2 dossiers, les arbitrages financiers semble tarder à venir madame la ministre, quel calendrier envisagez-vous par ailleurs la situation financière Delaunay Rassat, Verts, encore fragile, le fils doit certes poursuivre l'adaptation de son offre aux besoins industriels et s'efforcer de mieux valoriser sa recherche mais, compte tenu notamment de la structure actuelle de marché sur lequel s'inscrit cette établissement nous sommes inquiets de voir son pilotage déterminées, peu ou prou par les économies madame la Ministre, pourriez-vous nous rassurer sur le soutien de l'État continuera d'apporter à cet outil essentiel pour la filière aéronautique et spatiale et qui contribue à faire de la France, un des très grands acteurs mondiaux et pour terminer, un mot sur Djibouti, puisque les programmes, les crédits du problème 144 finance entre autres l'aide versée au titre d'un peu l'implantation des forces françaises et alors que la Chine dispose aujourd'hui à Djibouti de sa première base militaire à l'étranger, il est important de ne pas laisser notre influence décroître dans cette zone stratégique même la ministre quelles des assurances, pouvez-vous nous en donner, je vous remercie par avance de vos réponses. Merci, monsieur le rapporteur, la parole est à monsieur Michel Boutant. Rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées pour le programme environnement et prospective de la politique de défense et ce pour 3 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chaque Oleg, le dernier livre Brandt blanc, pardon la vite affirmé la revue stratégique, l'a confirmé dans un monde de plus incertain, plus dangereuse, la France doit poursuivre ses efforts dans le domaine du renseignement, conditions de son autonomie stratégique, le projet de loi de finances pour 2018, ça, ce qui d'ailleurs dans ses objectifs. Premières observations que l'on peut faire, c'est que les 2 services qui dépend du ministère des Armées, à savoir la DGSE, savoir la DGSE, les services extérieurs et la DRS des Direction du renseignement et de sécurité de la Défense, poursuivent la montée en puissance de leurs effectifs. La DGAC bénéficie pour sa part sur la période de 822 créations d'emplois 2014 et 2019 410 ont été déjà réalisés, l'effort principal reste à conduire ou, tout au cours des 2 prochaines années la DRS des bénéficie sur la même période de 534 créations d'emplois, dont seulement 243 ont été réalisés, la difficulté du recrutement et de fidélisation des personnes globalement surmonter à la DGSE, tient à la spécificité de certains profils recherchés et à la faiblesse des viviers. La DRS des confrontés de surcroît à une véritable transformation de son activité de sa structure d'emploi par manque de visibilité, il s'agit d'un petit service, mais aussi de capacité à proposer des niveaux de rémunération suffisante, elle éprouve des difficultés à assurer cette montée en puissance dans les 2 services la fonction ressources humaines devrait être confortée et des solutions devraient être apportées pour leur permettre de recruter dans de meilleures conditions. Des améliorations suite aux missions d'audits sont en cours, mais elle reste timide par rapport aux enjeux madame est ministre, quelle solution pouvez vous esquissé dans la perspective de la prochaine loi de programmation militaire qui verra sans doute un nouveau renforcement en effectifs des services 2ème observation pour héberger ces nouveaux effectifs mais aussi leurs capacités techniques, les 2 services ont engagé sur son propre budget pour la DGSE ou envisagent d'engager avec le concours et le financement de la direction du Patrimoine pour la DRS d'importants programmes immobiliers à cette fin, la DGSE à renforcer son expertise technique, la DST, elle cherche à regrouper ses différentes entités dans un bâtiment unique plus fonctionnel pour améliorer son efficacité et son fonctionnement horizon ce projet sera-t-il soutenu par la programmation militaire 2019, 2025 3ème et dernière observation la DRS dit a pu répondre, non sans difficultés, avec l'appui des réservistes à l'explosion des demandes d'habilitation et David sécurité suite aux attentats terroristes, il faut en effet s'assurer de la loi, il tout noté et fidélité des militaires, en revanche, en matière d'inspection de sites, le respect des programmes de visites pour identifier leurs vues ni la vulnérabilité s'avère compliquée avec l'accroissement du nombre de sites inspecter le ratio c'est effondré en 2016 et à peine redressé en 2017 même si la priorité donnée au point d'importance vitale a été respectée, le Centre d'inspection amorcé sa remontée en puissance, là aussi, les créations d'emplois sont nécessaires, mais le temps de formation est longue et les résultats se font attendre, surtout, il faudrait que les préconisations soient effectivement mises en oeuvre, ce qui n'est pas toujours le cas dans les délais requis, on l'a vu avec le malheur aux épisodes du vol survenu dans le dépôt de munitions de Miramas, s'il faut conclure, j'y arrive, j'ai encore 2 phrases président notre commission demande depuis plusieurs années, la mise en place d'un indicateur de performance spécifique est tout disposé à le mettre en place qu'est-ce qui pourrait éventuellement s'y opposer. Merci, monsieur le rapporteur, la parole est à monsieur Christian Cambon, président de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées, vous avez 9 minutes Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues de la commission des finances, mes chers collègues. Puisque c'est l'occasion de ce 1er exercice budgétaire de notre commission je voudrais tout d'abord réaffirmer ici notre respect et notre confiance pour fort pour nos forces armées l'heure même où nous parlons, 30 1000 de nos soldats sont déployés sur notre territoire, comme dans les zones de crises les plus dangereuses, nos armées sont un élément vivant de la nation elles remplissent avec professionnalisme, engagement et courage, une mission particulièrement difficile, je veux ici au nom de la commission leur rendre un hommage confiant et sincère, mais au-delà des paroles, notre soutien passe par des actes, des actes, c'est-à-dire des moyens à la hauteur des missions, c'est tout l'enjeu du débat budgétaire, alors Madame la Ministre, nous sommes perplexes perplexe devant une équation budgétaire aussi énigmatique. D'un côté, le gouvernement nous annonce Des hausses de crédit sans précédent qui montrent clairement que l'on s'engage sur la bonne voie, l'hémorragie est stoppée, mais de l'autre côté, nous pointons avec inquiétude les trop nombreuses dépenses non financées, report suppression gel de crédits qui rendront bien aléatoire l'effort annoncé 850 millions perdus en juillet et ce gel de 700 millions qui s'ils ne sortent pas rapidement des congélateurs de Bercy finiront par ne plus être consommable, nos soldats en ont besoin pour assurer leur mission et leur propre sécurité et nos 4000 entreprises qui attendent aussi, pour faire vivre un secteur économique riche de plus de 200000 emplois aussi, nous nous interrogeons quelle est la valeur du vote du Parlement, nous avons voté ici il y a un an, ces crédits sont-ils bloqués par des arbitrages gouvernementaux, mais quelle est dans ces conditions, la valeur du débat que nous avons chaque année sur le budget et ça débat A-S un débat virtuel, Madame la Ministre, nous aurions sincèrement aimé accompagner vos efforts personnels par un vote favorable, malheureusement, à la commission que j'ai réuni à nouveau hier préconise désormais, à l'instar de nombreux groupes l'abstention sur les crédits de la mission défense au vu de cette incertitude insupportable sur la fin de gestion 2017 enfin au nom de quoi fait-ont pesé sur la défense, c'était de Damoclès nous soldats qui risquent chaque jour leur vie n'ont-ils pas le droit de disposer des ressources que le Parlement a voté pour cette prospects station ne s'adresse évidemment pas à vous, madame la ministre des armées, si vous êtes bien sûr tenue au principe de la solidarité gouvernementale, nous mesurons et je peux en attester : ici, aujourd'hui, votre détermination personnelle et votre pugnacité pour obtenir ces crédits et c'est pour vous aider que nous lançons cet appel au gouvernement pour qu'il aille au bout de son engagement, certes, le projet de loi de finances pour 2018 affichent une augmentation d'1 milliard 800 millions d'euros, il poursuit : les programmes d'équipement, les recrutements dans le renseignement et la cyberdéfense il accentue la protection des hommes et des emprises, ils mettent en application ce plan famille et conditions de vie militaire qui porte, Madame la Ministre votre marque personnelle et nous vous en félicitons mais nous sommes perplexes, car si on nous annonce en 2025, un effort enfin rehaussé à 2 pourcent certains ont même le culot de nous expliquer qu'on y est déjà aux 2 pourcent et qu'il suffit simplement d'compter les pensions, mais mon Dieu, pourquoi n'y avons il n'y avait-on pas pensé plus tôt, de même la remontée en puissance saura si concentré entre 2022 2025 avec une courbe de croissance qui s'accélère vertigineuse vertigineusement après ce quinquennat que sa source que sa soutenabilité peut-être sérieusement mise en cause perplexe aussi car enfin les sommes affichées 1 milliard 8 puis 1 milliard cette de chaque année sont hélas siphonné par le refus au clash des OPEX, derrière ce mot abscons, il faut comprendre un transfert pur et simple de leur financement, de la solidarité inter-ministériel vers les armées, sans parler des subterfuges pour freiner tout investissement futur, je parle bien sûr de l'utilisation de l'article 14 de la loi de programmation des finances publiques dont nos amendements neutralisé les effets mortifères pour nos armées, le sort de ces amendements est désormais confiée cher président à la commission des finances, elle saura nous en sommes persuadés en défendre la rédaction auprès des députés lors de la commission mixte paritaire je n'énumère pas toutes les questions en suspens, les rapporteurs pour avis les ont magnifiquement décrite et je veux saluer leur travail d'approfondissement dans un délai extrêmement court que chacune et chacun ont pu réaliser, je les en remercie, qu'il me soit juste permis de reléguer 3 points noirs, ils ont mis en avant, l'immobilier, cela vient d'être évoqué, il manque 400 logements au moins aux militaires en région parisienne et nous regrettons la proportion très faible de logements sociaux pour les militaires au sein de l'îlot Saint-Germain, un sur 5 avec un cadeau de 50 millions d'euros à Madame la maire de Paris après le cadeau fait à Sciences Po pour l'hôtel de l'artillerie, tout ça fait beaucoup, notre commission avait tenté de protéger ses recettes, l'Assemblée ne nous a pas suivis, Madame la Ministre, nous pensons qu'il faut absolument conserver le Val-de-Grâce comme réserves immobilières pour nos armées obtiendrez-vous que ce soit la position du gouvernement disponibilité des matériels ensuite les rapporteurs ont décrit les effets désastreux de la fameuse courbe en baignoire qui frappe à la fois les matériels neufs comme les anciens, chacun connaît ici les prouesses qu'il faut réaliser pour maintenir en service des matériels d'âge canonique, alors que dans le même temps, des hélicoptères de toute dernière génération et les tout récents A400M connaissent eux aussi des défauts de de maturité qui les cloue au sol noir, le soutien, le soutien éternel sacrifié qui est, aujourd'hui, à force d'être laminés, devenu un véritable talon d'Achille, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le service de santé des armées qui est au bord du haute il mène de front une vigoureuse réforme comme bien peu d'administration en sont s'y sont engagés, et dans le même temps, une activité très intense en opération, la rupture n'est pas loin, or c'est vraiment la capacité de projection de nos armées et le secours, il convient de leur porter qui est en jeu, en résumé : Madame la ministre, qui est frappant, c'est évidemment le décalage le hiatus pour ne pas dire la contradiction manifeste entre cette somme d'incertitudes sur le moyen de sur les moyens des armées et l'aggravation de la menace décrite par la revue stratégique français, le président Macron a été accueilli à Ouagadougou par des jets de grenades sur des soldats français, la revue stratégique a décrit la dispersion des crises depuis les immensités sahéliennes où le terrorisme est toujours actif jusqu'aux confins de la mer de Chine à l'espace extra-atmosphérique au cyberespace est au coeur même de nos propres sociétés démocratiques abreuvés de désinformation et comme pour appuyer nos craintes, ce missile InterContinental nord-coréen vient nous rappeler la triste réalité, face à ces menaces, c'est bien le maintien d'un modèle d'armée complet, équilibré, qui est l'enjeu de la prochaine loi de programmation annoncée pour février, cela impliquera il faut le mesurer pleinement un effort considérable sur les moyens car le modèle est bon, mais nous sommes exempt et à l'issue d'une décennie des raids des rendements et de sous-investissement, il va falloir prendre les bonnes mesures et si tenir cet effort requis pour notre sécurité sera aussi rentable pour notre économie, nos collègues de la commission des finances, le savent bien : la défense, c'est 200000 emplois de haute technologie non délocalisables, c'est le 1er budget d'investissement de l'État, ce sont des investissements de rupture d'innovation qui tire toute l'économie, c'est une quinzaine de milliards d'euros d'exportation par an, combien de secteurs de l'économie peuvent en dire autant alors Madame la Ministre, au moment du vote, ce sera le choix le triste choix de l'abstention, paradoxalement, ce sera un moyen de vous soutenir, vous personnellement dans vos efforts mais nous voulons surtout dire au gouvernement qu'en matière de défense, il faut tenir le langage de la vérité, car il en va du moral de nos soldats, mais aussi de la sécurité de la France. Merci monsieur le président, dans la suite de notre discutent. Donc, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque discussion prend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote par ailleurs le gouvernement dispose au total de 20 minutes pour intervenir. La parole est à présent à monsieur Claude ou du groupe, la République en marche pour 6 minutes. C'est le président, madame la ministre, messieurs les présidents de la commission des finances et de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Avant tout, vous me permettrez d'adresser solennel hommage à nos forces armées. Qui, dans un contexte international sous tension impliquant au niveau de sollicitation et de mobilisation répondre présente et accomplissent leur devoir avec courage, abnégation et dévouement. Seul à moins de 3 jours et ça a été rappelé à l'instant, avant l'arrivée du président de la République a ou à Ouagadougou, nos militaires ont dû faire face à une attaque terroriste, je tiens à ce titre à transmettre mes pensées les plus émues à leur famille. Ces actes nous rappelle le devoir de vigilance qui s'impose à nous, si nous voulons combattre efficacement cette menace permanente qui pèse sur nos armées devant une telle situation, il apparaissait indispensable que les moyens budgétaires alloués à la défense soient renforcés, à cet égard je souhaite souligner l'ampleur de l'effort réalisé par le gouvernement en faveur d'une budget à la hauteur des ambitions définies par le président de la République, les crédits inscrits type de la mission défense sont conformes à ses engagements, consolidation des reconstructions de l'capacité et réaffirmation de la grande ambition pour notre pays en Europe et dans le monde, il s'agit des effectifs et des investissements en matière d'équipement ou en faveur des conditions de vie de nos soldats. Ce budget présente des avancées que notre groupe ne peut que saluer. Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, ce budget n'est autre que le début d'une remontée en puissance exceptionnelle 8 milliards d'euros supplémentaires étant accordée cette année à la mission défense, il s'agit là d'une augmentation inédite depuis 20 ans, qui s'inscrit dans la durée puisque chaque année 1,7 milliards d'euros supplémentaires sera accordée, avec comme objectif de consacrer les fameux 2 pour 100 de notre PIB à la Défense en 2025. Elle nous permet d'inscrire le budget des armées dans une dynamique durable. Nous voyons bien, mes chers collègues, que ce budget est une réponse à la hauteur des âges stratégiques qui s'impose à nous, une réponse aux défis de l'avenir de nos armées, une réponse enfin pour leur engagement pour leur courage. Si on devait trouver 2 axes forts à ce budget, nous pourrions qui répond aux préoccupations immédiates tout en préparant l'avenir. Comme je le disais précédemment, le projet de loi finance prévoit une hausse de 1,8 milliards de crédits budgétaires en 2018 par rapport au budget 2017, soit une augmentation de 5 pourcent pour rappel, 8 milliards d'euros, cette profond, plus que la roche s'intervenue en 2017 qui était de 600 millions d'euros. Avec 190 millions de recettes issues des sessions qui s'ajouteront crédits budgétaires, le montant des ressources de la défense sera à 34,4 milliards d'euros. Entre 2018 et 2022, ce sont donc près de 190 milliards d'euros que la nation consacrera à sa défense. La hausse significative du budget de la défense, vous permet de dépasser aujourd'hui très largement la barre symbolique de 1,8 pourcent il s'agit là du 1er jalon pour Athènes dans l'objectif fixé par le président de la République de porter le budget des armées à 2 pourcent du PIB, soit 50 milliards d'euros hors pensions et à périmètre constant, d'ici 2000 c'est donc la première étape d'une trajectoire financière qui sera décrite dans la future loi de programmation militaire 2019, 2000 Evensen qui sera présenté au Parlement en 2018, madame la ministre, comme vous l'avez justement précisé devant la commission des Affaires étrangères de la Défense, au début du mois, cette loi de programmation militaire droit porter une vision. Et ne pas se réduire à dos simples ajustements. Vous pourrez compter alors sur le soutien du groupe pour la République, Armand. En résumé, la mission défense que nous étudions aujourd'hui donne d'une part des moyens au maintien en condition opérationnelle des équipements et, d'autre part, préparent leur remplacement. ce budget préparent également l'avenir avec plus de 4,7 milliards d'euros consacrés à la recherche et développement, nous permettant d'anticiper les mutations technologiques de demain, ce sont, pour toutes ces raisons que vous pouvez compter sur l'engagement des sénateurs de République en marche qui approuveront sans aucune réserve, votre budget, mais j'ai cru comprendre que nous serons bien seul à le faire ici au Sénat, sur ce que j'ai pu entendre jusqu'ici. En fait, Madame ministre groupe leur à qui a rappelé qu'il partage pleinement la volonté du président de la République de voir émerger une véritable Europe de la défense. Il y a de cela plus d'un mois, je précise à cet hémicycle les conclusions de la revue stratégique mettez un exergue les mutations que connaît le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde de plus divisée plus changeant un monde aussi où les nouvelles technologies ont pris toute leur place, offrant à la fois des opportunités exceptionnelles et de nouveaux défis. La zone telle contexte : la France ne pourra agir seul pour assurer sa défense si le maintien d'une autonomie décisions au niveau hexagonal apparaît indispensable, l'Union européenne et l'échelon d'avenir en matière de défense notre avenir passe par la construction d'une Europe de la défense qui puisse intervenir, qu'il puisse nous compléter et puis nous pousser à innover et à réussir. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Yvon Collin pour le groupe RDSE pour 6 minutes chers collègues. C'est le président, madame la ministre, chers collègues. Le Tir de missiles InterContinental effectuée mardi par la Corée du Nord de tragique attentat dans une mosquée du nord-est égyptienne, sont les plus récents événements. Qui témoigne d'un contexte international dégradé et sous tension, ce dont nous, d'autres qui ont pas, hélas, même si on peut se satisfaire, bien sûr, Madame la Ministre, du recul de Daech Syrie ou en Irak. En effet, la revue stratégique de défense et de sécurité nationale dont nous avons discuté ici à quelques semaines, fait état de cet environnement instable, incertaine d'un ordre multilatéral remis en cause et du naufrage exposer au du cirque durcissement du terrorisme djihadiste dans ces conditions, notre pays ne devrait pas ralentir ses agrège Marnaval longtemps le niveau de mobilisation de nos forces et très important sur les théâtres extérieurs des théâtres d'opérations qui durent bien souvent au-delà de ce que l'on prévoit. Par ailleurs, parce que l'ordre dit BASF et de notre temps, nos soldats doivent aussi concourir à la sécurité du territoire national, avec l'opération Sentinelle. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous examinons ce soir une émission particulièrement sensibles et pour laquelle les moyens doivent être à la hauteur des défis. Cameroun devant conserver notre rang de puissance militaires pour garantir notre autonomie stratégique, bien sûr, mais aussi, madame la ministre, pour rester crédible, tant au sein de l'Otan, que de l'Union européenne aussi le projet de loi de final ce pour 2018, 5 ce qui est-il la mission dans une 3G/3 ascendant qui pourrait conduire à porter l'effort de défense à 2 pourcent du PIB d'ici 2025, c'est une question, la réponse est oui sur le papier, avec une hausse de 8 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2017, les crédits seront au rendez-vous seront-ils, ils sont même 5 6 mois supérieur au monde pas inscrit dans la loi de programmation militaire pour les années 2014 et 2019. Et ce progrès, Madame la Ministre, mérite d'être salué, tant du côté de la commission des finances que celle des Affaires étrangères de la Défense et les rapporteurs ont émis des doutes. Et j'en partage certaines vous le savez, madame la ministre, plusieurs points interroge mais vous allez sans nous apporter des réponses, il y a la question des crédits encore gelés, soit 700 millions d'euros mais surcoût des OPEX suscite aussi, comme chaque année, des inquiétudes, bien que la dotation initiale soit augmentée, nous l'avons noté de 200 millions dans le budget toutefois un septembre dernier le montant de ces surcoûts était évalué, vous le savez, 53 milliards d'euros, cette hausse n'améliore pas complètement la budgétisation des OPEX, qui reste à la merci du financement interministériel, la Cour des comptes d'ailleurs rappelé tout récemment. Mais comme je l'ai dit, il y a un effort certain et celui-ci permettra de répondre à plusieurs urgences tout d'abord celle des équipements et les infrastructures, la hausse des crédits en faveur de la capacité des cyber défense et de renseignement de la dissuasion nucléaire ou de l'entretien programmé des matériels contribuent à maintenir un modèle d'armée sans abandon capacitaire. Je voudrais également Madame la ministre, souligné l'effort budgétaire en faveur de la condition militaire, notamment au travers du plan d'amélioration de la condition des en marge de celui-ci, le plan famille est une très bonne initiative que nous saluons, je le rappelle à la multiplication des théâtres extérieurs conjuguée aux opérations de sécurité nationale sollicite fortement les ressources humaines, le dernier rapport annuel du Haut comité d'évaluation de la condition militaire, a constaté un certain nombre d'obstacles à la fidélisation des soldats, à un moment où nous avons, nous avons de plus en plus besoin d'être Les conditions de vie, que ce soit le quotidien sur le terrain sont de plus en plus difficile, vous le savez, pour les militaires sur le terrain, le fort engagement opérationnel fragilise à la fois les capacités et la sécurité, les militaires, le manque d'entraînement et le sous-équipement ne font que s'accroître au sein de nos armées, selon le rapport du Haut comité des équipages de blindés n'avait ni tirer ni manoeuvrer avec leur matériel, de dotation depuis près de 2 ans, s'agissant de la vie quotidienne des infrastructures immobilières et la qualité des de restauration ne sont pas non plus à la hauteur des besoins j'ajouterai enfin que la question du versement des sols Bentham perturbé par le trop célèbre logiciel Louvois ne doit pas être totalement réglé, vous apporterez sur ce point des il réside, il résulte maintenant ministre ces difficultés, un problème de fidélisation des armées pour ne citer que l'armée de terre, seuls 65 pourcent des militaires de rang signer un nouvel engagement. C'est pourquoi madame la ministre, c'est un vrai sujet sur lequel nous devons être plus attentif car l'armée, c'est peu de le dire, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui sacrifient beaucoup au service de notre pays, le président de la République l'a rappelé à Istres en juillet dernier, je le cite : il faut que les militaires et les moyens de leur mission et que les ressources nécessaires soient engagées voilà un objectif, madame la ministre que nous partageons, nous comptons sur vous pour engager la mission façades dans ce sens sur ce budget, personnellement, je voterai apporterai mon soutien un celui, tout comme Jacques pauvreté requis et président de notre groupe, d'autres plus réservés s'abstiendront sauf si madame la ministre, vous nous apporter un temps de débat de bonne réponse, je vous remercie par avance. Merci, cher collègue, la parole est à madame Christine Pruneau. Le groupe CRCE pour 6 minutes.

Madame la Ministre, chers collègues, le groupe CRCE, que je représente donc ce budget est en trompe l'oeil, certes, une augmentation des crédits et proposer mais elle cache la nécessaire compensation des crédits annulés c'était et sans oublier la revalorisation insuffisante mais réelle du surcoût des opérations extérieures, dans ce budget, la dissuasion nucléaire tient toujours une place prépondérante, puisqu'elles représentent 22 pourcent des dépenses d'équipement et 10 pourcent du budget total de la défense d'équipement, hors pensions, ce sont 3,6 milliards d'euros mobilisés cette année dans le cadre du plan de modernisation qui nous engage sur 20 ans à l'heure où les discussions de l'ONU ont amené 122 pays à adopter un traité d'interdiction des armes nucléaires, en vertu de l'article 6 du traité de non prolifération, nous l'avions déjà évoqué Madame la ministre lors d'un débat et où le prix Nobel de la paix a été décerné aux initiateurs de cette démarche, il est retraité table que la France est boycotté des discussions et refusé de de signer le traité untel niveau de dépenses nucléaires pour une modernisation s'avère plutôt être un renforcement nucléaire car on sort clairement du domaine de la maintenance et du maintien des conditions de ce qui de sécurité qui sont tout à fait normal lorsqu'on équipe un nouveau sous-marin 2 missiles M-51, alors mon groupe a souhaité interpeller monsieur François Hollande, il fut un temps, là maintenant, le président Emmanuel Macron sur cette question et les réponses, bon nous laisse perplexes mais nous nous comprenons aussi, je cite, le poids de la menace nord-coréenne empêche tout démantèlement ou encore des discussions menées par des États nos détenteurs ne saurait être légitime c'est surtout cette dérive dernière phrase qui me m'interpelle, madame la ministre, je me permets de vous poser cette question, mais que vous vous êtes posé, si j'ai vendu, quelle est la la légitimité des états détenteurs donc par exemple nous-mêmes interdire les autres pays à développer des programmes nucléaires si eux-mêmes refusent d'arrêter leur programme, moi je trouve que c'est un gros dilemme sur lequel il pourrait y avoir plus de réflexion dans notre commission, par exemple, la seconde critique sur ce budget est relative à l'intégration de la France dans l'Otan depuis 2009, notre pays a perdu en grande partie sa souveraineté en matière de défense, en effet, l'Organisation de coopération de défense s'est vite transformé en UNOG, organisation transe régional militaire, la raison de notre défiance vis-à-vis de l'Otan, qui n'est pas une situation nouvelle tient 2 éléments suivants que je souhaitais vous repréciser premièrement l'organisation Atlantique est aujourd'hui à l'initiative d'une véritable course aux armements ainsi le fameux seuil de 2 pourcent du PIB est d'autant plus contraignant depuis l'élection de Donald Trump il a d'ailleurs déjà annoncé sa volonté de conditionner le recours à l'assistance mutuelle au respect par les États demandeurs du seuil de 2 pourcent cette course aux armements est une lecture très partiale de l'article 51 de la charte des Nations unies sur le droit à la défense, c'est un mépris pour l'article 26 de la même charte sur la nécessité de limiter au maximum les armes en circulation, je vous rappelle également que la multiplication des matériels de guerre sur le marché légal entraîne le développement du marché parallèle 90 pourcent des armes illégalement circulation sont fils du marché dit classique, deuxièmement et pour faire le lien avec la charte des Nations Unies, on assiste à une situation où une organisation militaire supplante totalement l'organisation internationale souveraine quelle ONU combien d'États se sont rendus coupables d'infraction aux règles des Nations unies en intervenant en Irak par exemple, en 2003, parce que les États-Unis et donc le temps avait décidé il y a les comment en 2011 : avons-nous pu passer d'une résolution de mise à l'abri des civils libyen à une opération de renversement du pouvoir nous avançons ainsi dangereusement sur le terrain du droit international d'ingérence, enfin, une dernière critique sur ce budget au sujet de la maîtrise de nos moyens opérationnels, la situation est paradoxale puisque notre pays n'a jamais autant produit de matériel de guerre, mais nos militaires, je pense qu'ici, nous l'avons tous répété n'ont jamais été autant dans des conditions si difficiles, des ligues d'équilibrer la balance commerciale de la France avec la vente de demain derrière de guerre, quelles que soient les acheteurs nous sommes inadéquate ainsi : comment expliquer que nos soldats continuent d'utiliser des véhicules d'avant, rôle blindés mise en service en 76, vu que ça m'a énormément surprise ou des gilets pare-éclats faute de gilets pare-balles, je sais que la situation, vous avez repris le dessus, de plus, la multiplication des opérations, a conduit à une surexploitation du matériel et du personnel, à titre d'exemple, citant les services de santé des armées Pour conclure, chers collègues. hors service, faute d'une politique immobilière inadapté, je termine justement je voulais terminer cette intervention en ayant une pensée pour nous, soldats mobilisés en France ou à l'étranger revenir aussi pour preuve comme ont dit mes collègues sur le gel de 700 millions d'euros sur le programme, qui assurait la sécurité ne soldats, ce n'est pas une critique de votre volonté de votre investissement qui est mis en cause le nommé ministre, mais pour toutes ces raisons,

Monsieur le Président, Madame la ministre, messieurs les présidents de commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, depuis quelques années, comme nous le savons tous la défense nationale est revenu plus que jamais au coeur des priorités de notre pays à ce titre, ce projet de budget constitue la trame financière des ambitions élevées et des engagements pris par le gouvernement en matière de défense pour permettre aux Français de vivre en sécurité et à notre pays de garder son statut. Je salue bien évidemment la progression de 1,8 milliard d'euros, des crédits de paiement permettant de passer de 32,4 milliards d'euros en 2017 à 34,2 milliards pour 2018 c'est une hausse historique qui constitue un premier efforts significatifs pour atteint l'objectif de porter les ressources désormais à 2 pourcent du PIB, soit 50 milliards d'euros à l'horizon 2025, ce budget comporte cependant plusieurs points de vigilance qui n'ont pas manqué de souligner durant nos travaux en commission mais également par nos collègues députés, je parle ici de l'annulation de 850 milliards d'euros intervenu en jeudi en juillet 2017 et des 700 millions d'euros de crédits reportés en 2016 et 2017 qui sont encore gelés San financement interministériel du surcoût des OPEX et démission intérieures et sans un dégel, au moins partielle, de ces crédits la portée et la sincérité de ce budget serait totalement remis en cause, je ne reviendrai pas sur la totalité des crédits que nous remporterons déjà fort bien détaillé, je me contenterai d'évoquer simplement quelques points incontournables : il y a 4 programmes de la mission défense tout d'abord, le financement des OPEX, cela me semble être une des questions centrales de ce budget, nous constatons actuellement que la contribution nationale à l'effort de défense entre tous les ministères est incertaine, une part croissante de cette somme relèvera désormais du budget des armées avec 650 millions d'euros de provision pour le financement des OPEX en 2018, il faut souligner que cette hausse de 200 millions va dans le sens d'une meilleure prise en compte des réalités et des enjeux, cependant, dans un souci de lisibilité et d'optimisation de budget ne serait-il pas, Madame la Ministre, nécessaire de créer une véritable section budgétaire spécifique pour les OPEX adossé bien évidemment au budget de la défense, avec une prévision d'au moins 1 milliard d'euros, dont 850 millions seraient financés par les administrations habituellement mises à contribution, madame la ministre, schéma serait bien plus clair et permettrait donc de préserver en parallèle avec certitude les augmentations de crédits pour nos équipements ceci m'amène à évoquer le programme 146 relatif à l'équipement des forces qui concentre l'essentiel des investissements de l'État, la hausse significative de 34,7 pourcent des autorisations d'engagement permettra d'encourager l'élan indispensable du renouvellement des matériels actuellement, le taux de renouvellement des équipements militaires n'est pas suffisant, malheureusement pour empêcher leur vieillissement, les chiffres sont extrêmement inquiétant 60 pourcent des véhicules de l'avant blindés en OPEX sont vieillissants et non pas de protection suffisante, ce qui expose nous soldats à des dangers certains, en effet, nous avons des véhicules qui sont en service depuis plus de 30 ans, voire 35 ans, je pense notamment au VAB et quand les prochains véhicules arriveront, ces derniers pourraient avoir entre 40 et 45 ans d'utilisation, si nous ne prenons pas décision forte rapidement Madame le Ministre, ce sont des pans entiers de mission qui pourrait ne plus être rempli sur certains théâtres d'opérations, par ailleurs, plus les achats sont là, en plus des dépenses sont importants, puisque les pénalités versées aux industriels pour le non respect des contrats s'ajoutent au coût toujours plus élevé de l'entretien et du maintien en condition opérationnelle des matériels et 10 ans compte tenu du retard accumulé des alertes incessant de nos armées, sur ce sujet, l'accélération du programme Scorpion sur lequel vous êtes très mobilisée, Madame la Ministre, doit être une priorité absolue ainsi l'achat de nouveau matériel permettrait de disposer de capacités techniques et tactiques bien supérieur aux caractéristiques actuelles, sans parler du niveau de protection que nous pourrions alors garantir à nos militaires une diplomatie forte sans une armée à l'auteur ne peut garantir le rayonnement de notre nation et la sécurité escompté nous reviendrons évidemment à ce sujet, Madame le Ministre, lors du projet de loi de programmation militaire prévue au printemps 2018 un point maintenant sur le programme 144 dont les crédits sont en progression de Calzaghe 5 pourcent essentiellement consacrés au renseignement qui permettra de renforcer les actions de la DGSE et de la DRS des services très sollicités dans le contexte de lutte contre le terrorisme que nous connaissons. Veillons cependant à ne pas négliger la conduite des relations internationales et la diplomatie défense action 8 de ce programme pour maintenir également la capacité d'influence de la France qui prête actuellement quelques inquiétudes, je pense notamment à l'Afrique où j'étais encore il y a quelques jours, sommes-nous encore en capacité de maintenir notre influence et de protéger nos intérêts français en matière défense sur ce continent avec plus de 1000 soldats au Soudan du Sud, avec près de 700 au Libéria et 400 au Mali, la Chine est déjà très très présente sur le continent africain, ce qui lui permet, selon le Conseil européen des relations internationales de développer sa connaissance des terrains extérieurs et protéger ses intérêts économiques, comme au Soudan du Sud je pense également à la 1ère base militaire de la Chine, installés à l'étranger et plus précisément à Djibouti, ce pays n'a pas été choisie au hasard puisqu'il a une position stratégique dans la Corne de l'Afrique et ce territoire est la porte d'entrée vers l'Afrique de l'Est et l'océan Indien, autant d'exemples qui montrent qu'aucune action du programme de doter d'exiger enfin pour conclure, je souhaite aborder les enjeux liés au programme 212 au 1er chef desquels les ressources humaines, le 11ème rapport annuel du Haut Conseil d'évaluation de la fonction militaire publié le 6 octobre 2017 pointe la difficulté récurrente pour l'armée de fidéliser ses effectifs près de 62 pourcent des militaires envisage aujourd'hui de quitter la fonction, les raisons sont multiples de l'obsolescence du matériel à la mobilité géographique, en passant par les conditions d'hébergement ou les parcours professionnels, difficile parfois pour les conjoints l'excellente initiative du plan famille madame la ministre, doté de 300 millions pour 5 ans devrait permettre à n'en pas douter de répondre progressivement au besoin d'amélioration de la condition des personnels sur certains aspects incontournables d'autres défis restent à relever, comme la création de plus de passerelles entre armée et fonction publique ou encore une réflexion à mener sur la concurrence du secteur privé qui offrent généralement des salaires et des conditions de vie plus attractive pour les spécialités très technique mais aussi pour les professionnels de santé, tels que les médecins dont les effectifs sont très insuffisants, notamment en OPEX, nous espérons, Madame la Ministre, que ce budget pourra garder toute sa sincérité, notre groupe Union centriste, conscient de l'effort budgétaire réalisé souhaitait apporter un soutien unanime, malheureusement, le maintien du gel des 700 millions d'euros à l'heure où nous parlons, nous conduit à une abstention sur les crédits de cette mission, je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue là. Parole est à Madame Hélène Conway Mouret du groupe socialiste et républicain pour 10 minutes chers collègues.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, sert collègues avant d'entrer dans le débat de ce jour, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos militaires et leurs familles, pour celles et ceux touchés dans leur Chair, blessé au combat ou ayant donné leur vie au service de notre pays, pour celles et ceux qui ont perdu un camarade, un ami, un mari, un frère, je veux saluer la dignité des familles dans ces moments de douleur, saluer l'ensemble de nos forces armées, ainsi que le dévouement de ces femmes et de ces hommes engagés dans les missions qui leur sont confiés, partout dans le monde pour maintenir la paix, garantir la liberté de la France et assurer notre sécurité à tous, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur des frontières, ce qui a aussi exprimé notre estime pour le général Pierre de Villiers qui a accompli un travail remarquable dans ses fonctions, nous connaissons l'extraordinaire proximité qu'il a su entretenir avec ses hommes au-delà des armes, son souci de garantir que chaque homme et chaque femme engagée sur une mission puissent la réaliser dans les meilleures conditions possibles matérielles et sécuritaires. à travers son départ, nous voyons une rupture avec la gouvernance exercées jusqu'alors je voudrais enfin exprimer nos encouragements à son successeur, le général François Lecointre, chef d'État-Major des armées dans les compétences et le dévouement sont reconnues par tous, à travers lui l'ensemble des chefs d'État-Major, terre, air et marine pour déterminer la position de mon groupe, il me semble essentiel de replacer nos débats dans le contexte actuel, nous pourrions y voir une forme de continuité, celle-ci n'est qu'apparente, en effet, la méthode par laquelle a été conçu la revue stratégique nous interpelle, alors que les 2 précédents livres blanc de 2008 et 2013 avait associé les parlementaires et, au-delà, les acteurs de la communauté de défense, nous regrettons leur absence dans les lobes ration de ce qui représente la Pierre angulaire de la doctrine stratégique de la France, il serait souhaitable que les parlementaires soient associés plus en amont dans le projet de loi de programmation militaire, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat ont démontré par le passé qu'ils étaient en capacité de fournir des contributions de qualité au service d'une démarche collective, il en va de notre cohésion nationale autour de nos armées, ce budget pour les forces armées et la défense s'inscrit toujours dans un contexte sécuritaire de tension, attention à l'extérieur nous forces reste engagée dans plusieurs opérations. Chammal au Levant ou Daech a été vaincu le point de vue conventionnel, puisqu'il a perdu l'ensemble de ces emprises territoriales l'engagement de nos troupes durera encore longtemps à la sécurisation totale de ce qui va se d'espace prendra du temps, par Cano Sahel où la situation sécuritaire est préoccupante des attaques régulières du groupe terroriste particulièrement à l'encontre des populations civiles appellent notre vigilance et puis nos troupes restent présentes partout, sur de nombreux théâtres, notamment au Liban, où nos soldats poursuivent l'engagement quotidien du maintien de la paix, nos forces interviennent aussi sur le territoire national où la menace terroriste est bien réelle avec l'opération Sentinelle nos armées sont intégrées au dispositif, regroupant l'ensemble de nos forces de sécurité, même s'il a été réadapter chaque jour ce sont des milliers de militaires qui sont présents dans nos rues et sur les sites sensibles afin de nous protéger toutes ces opérations appelle un budget en progression, afin de permettre à chaque soldat de réaliser ces missions dans les meilleures conditions possibles lors de la dernière campagne présidentielle, la plupart des candidats, dont l'actuel président de la République se sont engagés à consacrer 2 pourcent du PIB aux dépenses militaires, l'année dernière, notre commission avait confirmé la nécessité d'atteindre cet objectif et on avait posé les jalons nous constatons aussi que les différentes déclarations du gouvernement fixe c'est engagement dans la durée, puisqu'il s'agirait d'atteindre 2 pourcent du PIB en 2025, c'est-à-dire 3 ans après la fin du quinquennat actuel poursuivant ce raisonnement 1,7 milliards d'euros de crédits supplémentaires sont inscrits pour l'année 2018 dans une montée en puissance progressive avec des augmentations similaires pour les années à venir, 1,7 milliard en 2019, 1,8 milliards en 2020 sont annoncés dans le même ordre d'idée, aucun programme ne semble avoir été annulée le PLF 2018 ne présentent pas sur le papier en tout cas le grande rupture avec la logique de consolidation de notre outil de défense qui a prévalu ces dernières années par exemple le programme 144 continue d'être affiché comme une priorité dans un n'environnement incertain, nous ne pouvons qu'approuver cette démarche de renforcement de nos capacités de renseignement ainsi que nos moyens d'action en matière de cybersécurité je pense enfin à l'apparente stabilisation budgétaire pour les programmes 146 et 191 notre industrie de défense doit être soutenu, présente dans le territoire à travers un tissu de PME et l'état des secteurs clés qui tire l'ensemble de notre économie, notamment avec ses 200000 emplois. Pérenniser notre modèle de défense, c'est garantir à notre industrie de conserver ses moyens en matière de recherche et de développement, en effet, le risque de nivellement par le bas, voire de décrochage technologique existe bien, enfin, le programme 178, pivot de la transformation permanente de nos armées permet de soutenir l'effort porté sur la protection des infrastructures et des personnels, toutefois nous restons vigilants, d'abord en ce qui concerne la marine parce que nous assistons à une montée en puissance des forces navales d'autres pays dans la protection de leurs espaces maritimes ensuite pour l'armée de l'air qui a vu ses équipements très sollicités par de multiples déploiements opérationnels, il en découle une tension pesant sur le renouvellement des stocks des systèmes d'armes et des équipages, enfin pour l'armée de terre qui supportait jusque-là la majeure partie de la réduction des effectifs si nous partageons un certain nombre de perspectives figurant dans ce PLF 2018, il n'en demeure pas moins qu'il soulève des interrogations, en effet, nous devons prendre en compte l'ensemble des éléments financiers, la hausse affichée du budget de la défense sans précédent depuis la fin de la guerre froide, nous apparaît bien artificiel, à la lumière des arbitrages pris depuis l'été, comme l'avait souligné nos anciens collègues, Jean-Pierre Raffarin et Daniel Reiner, il s'agit également de prendre en compte le coût des décisions entérinées par le Conseil de défense du 29 avril 2015 et inscrits dans l'actualisation de la loi de programmation militaire, cela représente un milliard d'euros pour 2018, 1,2 milliards d'euros en 2019. Oublions pas que le ministère des Armées a subi une coupe budgétaire de 850 millions d'euros en juillet dernier, cela a été rappelé beaucoup, elle conduit au décalage dans le temps d'un certain nombre de programmes, je pense par exemple à la rénovation de nos Mirage 2000 D mais il n'aura échappé à personne que derrière ces reports budgétaires, il y a des hommes et des femmes à qui l'on donne d'une mission, ces dernières ne peuvent malheureusement pas être repoussé dans le temps,

cela entraîne d'ores et déjà des renégociations de contrats avec les industriels, madame la Ministre, mais je vous ai déjà se poser cette question en commission, pourriez-vous nous éclairer sur le montant des indemnités compensatoires qui leur seront versées. Enfin, je rappelle que 700 millions d'euros de crédits défense sont toujours gelés par Bercy, même si cela est de saison nous espérons les voir des gelées très vite sans ces crédits l'augmentation affichée dans ce PLF 2018 manque de sincérité, au total, ce projet de loi de finances pour l'année 2018 présente une réalité budgétaire quelque peu différente de celle affichée par l'augmentation de 1,7 milliards d'euros du budget de la défense c'est augmentation, nous la soutenons, mais sans garantie de la part de Bercy quant au dégel de 700 millions d'euros de crédits défense nous ne pouvons pas voter cette proposition budgétaire en conséquence, le groupe socialiste et républicain s'abstiendra sur les crédits de la mission défense. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Joël Guerriau du groupe, les indépendants pour 6 minutes. Madame la Ministre, mes chers collègues, ce président dans le cadre de la vue stratégique le 24 octobre dernier nous exprimer dans cet hémicycle, notre volonté de disposer d'une armée complète et crédible pour faire face à un monde où les menaces se propage comme un feu de brousse, ce budget ne permet-il dans la Seine, un arbre, capable de se dresser et de résister aux feux de brousse au cours de ces dernières années: le budget de la Défense a fait l'objet de sous-estimation de reports de charges d'annulations de crédits de promesses de recettes exceptionnelles sans lendemain et dans le même temps l'engagement de l'armée, aussi bien à l'extérieur que sur notre territoire n'a cessé de s'accroître, entraînant des besoins matériels et humains croissant, marque une nouvelle dynamique et je mettrai aussi l'accent sur 2 points de satisfaction, le 1er point de satisfaction concerne le volet humain, la défense et la sécurité nationale, c'est avant tout des femmes et des hommes qui s'engage pour notre pays, leurs engagements appliquent leurs familles qui en subissent les conséquences de plein fouet, difficulté à concilier vie militaire et vie personnelle mobilité reconversion hébergement sont autant d'écueils nous approuvons la mise en oeuvre d'un plan famille ainsi que l'évolution positive des crédits pour le personnel en faveur de la politique immobilière, le parc est en effet très très très dégradé sa main. Ayant été longtemps sacrifié pour préserver les dépenses d'infrastructure, des programmes d'armement, ce budget concrétise un effort en faveur de la condition du personnel. Pour autant, je dois vous avouer notre inquiétude quant à la bascule entre Louvois et source solde qui s'étendra entre 2018, 2020 et qui surtout va interférer avec la mise en place de la retenue à la source, voit, c'est un véritable scandale de l'État et nous n'avons donc pas le droit à un second échec, ce sera la toute la responsabilité du gouvernement le 2ème point de satisfaction, et dans l'augmentation accordée aux équipements, force est de constater le jour de matériels lié au niveau d'engagement de nos armées, la progression des crédits d'entretien du matériel pour un maintien en condition opérationnelle est une un juste retour des choses pour l'armée de l'air de dans ce budget, la livraison de matériel qui nous font cruellement défaut, il en va du 1er ravitailleur en vol MRTT la montée en puissance du transport aérien, le 1er avion léger, de surveillance et de reconnaissance, lancement du programme de recueil de renseignements électromagnétiques Lucu au niveau de l'armée de terre, ce budget qu'on compense des lacunes accumulées au cours des 15 ou 20 dernières années, nous équipons sont usés par plusieurs années de sous-dotation et de sur engagement parfois ils sont dépassés, comme le pistolet automatique de nos soldats qui date de 1950. Nous approuvons donc les efforts qui sont entrepris et pour autant il y a 2 domaines où nous devrions faire davantage. Le 1er domaine concerne notre capacité à innover au cours de son nez. Voir notre Nation assure relever les défis d'écologie, c'est injuste, une juste cause que d'accroître les crédits consacrés à la recherche cybersécurité et à la révolution numérique, la revue stratégique affiché l'ambition T. 2 logiques industrielles et je pense qu'il faut que nous attend si Fillon davantage nos efforts de recherche et de développement, il est temps de passer à des équipements de 4ème génération, c'est tout l'enjeu du programme Scorpion qui mérite d'être accélérée. En particulier au niveau des études environnementales et les travaux liés à l'innovation, mais je sais que vous il y a tout aussi convaincus, notre armée doit être doté d'un niveau de protection de haute qualité, le second d'un domaine qui me préoccupe et notre capacité à traiter les enjeux qui se jouent. Sur et sous les océans, la mer recèle d'immenses richesses énergétiques, halieutiques, bien sûr, mais aussi d'innombrables d'innombrables minerais indispensables, développement de haute technologie, or nous sommes payés mais surtout nous sommes convoité en termes de souveraineté notre Marine nationale. Et dans la capacité d'assurer une présence suffisante sur l'ensemble des océans pour couvrir le second espace maritime mondial qui est de notre ressort, désormais on croise plus souvent le pavillon chinois en Méditerranée. Plus que le nôtre, la Chine s'apprête à contrôler toutes les routes maritimes et donc les flux commerciaux ainsi que les communications intercontinentales, nous nous réjouissons, bien sûr, de livraison d'un barracuda sénats de la classe Club ont été rappelez-vous conçu pour une durée de vie de 25 ans aujourd'hui, ils ont presque 35 ans alors que la Chine, mais à la mer en 4 ans, l'équivalent de la totalité de la flotte française pour avoir navigué sur un Sénat, je tiens à rendre ici hommage aux équipages qui sont confinés dans les plus petits sous-marins du monde. Ils ont beaucoup de courage, croyez-moi bien, et ce sont des gens vraiment brillant, nous souhaitons que soit accéléré le programme Bach. Ciment de surveillance et d'intervention maritimes nous avisons sont usés et dans l'incapacité d'assurer une protection optimale de nos zones exclusives, nous saluons votre émission. Madame la Ministre d'engager la livraison de la patrie heures pour les Antilles de 2 bâtiments de soutien, d'assistance hauturier en 2018 et d'un bâtiment multifonctions mission B 2 cependant, reconnaissons-le, cela ne suffira pas pour assurer notre souveraineté outre-mer je suis également convaincu que nous avons besoin de 2 porte-avions, alors que même que le. Charles de Gaulle est en cale sèche pour 2 ans, la maîtrise des espaces aéro-maritime en dépend, nous ne pouvons pas continuer à courir le risque d'une présence discontinu, voire aléatoire, nos voisins britanniques l'ont bien compris et ont fait le choix de 2 porte-avions. Le terrain de jeu de l'économie et de l'écologie ne sera pas la mondialisation, mais la maritime mise nous disposons de formidables atouts industriels, nous devons mettre le cap vers la croissance bleue. Pour cela, notre Marine nationale est incontournable et doit être renforcé dans ses moyens d'action. Pour conclure, dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques et d'arbitrages difficiles, nous aimerions que l'effort affiché pour une augmentation, par une augmentation de 1,8 milliard d'euros de budget soit réel, l'annulation de 850 millions de crédits et puis maintenant le gel de 700 millions d'euros auxquels s'ajoutent 200 millions de plus pour les OPEX et les reports de charges risque une fois encore de masquer la réalité de ce que nous souhaitons. C'est la raison majeure pour laquelle le groupe des indépendants s'abstiendra tout en soulignant que nous croyons, Madame la Ministre à votre détermination à convaincre Bercy, nous souhaitons que les engagements pris soient pris soit strictement tenu ainsi nous démontrerons notre considération et ne provoque l'essence sans faire des femmes et des hommes engagés dans la défense de notre nation dans le même temps, entre 2 lois de programmation militaire, un contexte international sous tension. Une solidarité européenne encore trop timide ce de ce budget, nous invite à l'humilité. Merci, cher collègue, la parole. Et maintenant, à Madame Isabelle Raymond pas 0 pour le groupe, les républicains et pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la ministre, hein, Monsieur le Président, Cambon mesdames messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, tout d'abord, je souhaite rendre un hommage solennel aux femmes, aux hommes de la défense qu'ils offrent sur le sol national ou sur des théâtres d'opération à des milliers de kilomètres, nous les assurons de notre soutien indéfectible nous pensons particulièrement aux familles qui payent quotidiennement un lourd tribut à la défense nationale, permettez-moi également de remercier le président Christian Cambon pour son engagement et son fidèle soutien au travail des parlementaires au sein de notre commission je salue également l'application de mes collègues, rapporteur de la commission des finances et de la défense, je souhaite attirer votre attention sur le contexte dans lequel nous examinons ce budget en 1er lieu le contexte international, ces 5 dernières années ont été tragiquement rythmé par l'actualité le contexte géopolitique mondiale se caractérise par un accroissement des menaces et asymétrique en tant que puissance mondiale et membre du Conseil de sécurité de l'ONU, la France à continuer d'assumer ses responsabilités et son application dans les résolutions de crise, principalement en Afrique et on le vent a fortement et durablement mobilisés et fragilisé l'appareil de défense dans son intégralité de plus nos impératifs de souveraineté dans les territoires ultramarins le redéploiement des États-Unis et de la Chine dans le Pacifique, nous oblige à un recalibrage matériels, humains et stratégique afin de répondre aux défis majeurs de la maritime mise dans un second lieu, il importe d'être lucide sur la réalité de l'agenda gouvernemental là nous sommes dans un entre 2, à la veille de l'élaboration d'une nouvelle LPM et au début d'un nouveau quinquennat la réalité pour les comptes du ministère, c'est que nous arrivons à un mois avant la clôture de l'exercice 2017, plus pragmatiquement si leur état l'affichage d'ambitions internationales pour le président de la République, l'heure est aussi à celle du bilan comptable, notamment en terme de reports de charges et de calcul du surcoût des OPEX, le 1er devrait avoisiner les 3,5 milliards, ce qui est un niveau record, la projection d'objectif en termes d'investissements aussi louable soit-il, ne peut occulter le passif de la dernière année de la LPM à la fin de l'année 2017, de l'avis de tous, 3 mots caractérisent la situation des armées et de notre outil de défense excellence surtension usure comme l'rappelé mes collègues avant moi, initialement nous avions accueilli favorablement leurs plantations des crédits à hauteur d'1,8 milliards d'euros, si les 34,2 milliards de dotations pour 2018 laissé entrevoir des signaux positifs les mouvements comptables alternant annulation gel et dégel de crédits ne favorise pas la confiance, madame la ministre, nous savons les efforts que vous avez déployés pour compenser l'annulation des crédits de 850 millions intervenu cet été aussi nous regrettons que votre pugnacité se heurte à la rigidité du ministère de l'action et des Comptes publics alors que la revue stratégique ne réduit aucunement les ambitions de la France, l'incompréhension demeure face au gel de crédits de 700 millions d'euros, à quoi bon débattre dans cet hémicycle d'une revue stratégique presque idéale si nous ne décidons pas d'y consacrer les moyens conséquents, c'est dans ce cadre que s'inscrit de nos préoccupations concernant les OPEX et la politique de MCO la rebute, je dis à Sion à hauteur de 200 millions d'euros de la provision OPEX contraste avec la CSeries des 5 dernières années alors que le montant global des OPEX atteint systématiquement le milliard et que le surcoût surcoût dépasse les 600 millions chaque année, la remontée à 650 millions du budget OPEX témoigne du réalisme du ministère concernant les matériels, nous craignons qu'à terme, l'augmentation du report de charges pèsent lourdement sur le MCO et les programmes d'équipement, il ne s'agit plus du développement d'une base industrielle, technologique de défense mais de sa préservation vis-à-vis de nos partenaires européens, nous devons rester crédible performant et à la pointe de la recherche, d'ailleurs, Madame la Ministre, je vous avez interpellé sur les défis technologiques de la défense dans cette mixité la le 24 octobre dernier avant de conclure, et pour rester positif, je souhaite dire combien nous nous réjouissons de la mise en place du plan d'accompagnement des familles et d'amélioration des conditions de vie des des militaires, les 300 millions répartis sur 5 ans sont légitimement attendue car le mal-être des familles altère le moral et l'efficacité des soldats en mission, les mauvaises conditions de vie, il y a le ressenti pénalise les efforts de la politique de fidélisation que nous appelons tous de nos voeux aussi à la lumière de tous ces éléments, vous comprendrez que notre groupe s'abstiendra cette abstention n'est en rien hostile, elle révèle notre volonté de soutien pour les armées, et pour la préservation de notre appareil de défense. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Florence Parly ministre des Armées pour 20Minutes Madame la Ministre. Merci monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, en bon. La défense de la France avait besoin d'une réponse, elle est là. Le budget que je défends devant vous. être un budget de remontée en puissance. Il répond aux attentes de nos armées. Et il anticipe l'avenir. Nous avons déjà vu déjà, pardon, l'occasion de parler beaucoup ensemble de ce budget. Et j'aimerais cependant en quelques mots : rassurez vous en rappeler les grandes lignes. Ce budget, tout d'abord, c'est 1 milliard 800 millions d'euros supplémentaires pour notre défense, c'est une hausse historique. Jamais vu depuis 20 ans. Elle va permettre de donner à nos armées les moyens d'accomplir pleinement leur mission cette hausse va permettre de nouveaux équipements de nouveaux matériels et d'investir pleinement pour l'innovation. Cette augmentation va permettre d'honorer nos dettes du passé. Et de créer les conditions budgétaires saines et s'en sert pour bâtir la prochaine loi de programmation militaire en quelques mots, le budget 2018 permet de répondre aux besoins immédiats de nos armées par différentes mesures fortes. Tout d'abord, nous assurerons un soutien total à nos engagements opérationnels. L'intensité de notre engagement est forte, plus forte même que nous ne l'avions imaginée à l'origine. Mais ces engagements sont nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté des Français. Ces engagements use notre matériel. le PLF 2018 consacre donc 450 millions d'euros supplémentaires pour l'entretien programmé du matériel, cela permettra un retour de la préparation opérationnelle par les normes fixées par la loi de programmation militaire actuelle, la sécurité des Français passe par le bon exercice d'missions de nos soldats. Nous protégerons donc plus fortement et plus efficacement encore nos militaires, c'est le sens du paquet protection que je vous propose, dans le cadre de ce projet de loi de finances 2018 concrètement ce paquet protection, ce sont 200 millions d'euros pour la protection de nos forces, ce sont 49000 gilets pare-balles de nouvelle génération, et ce sont des véhicules blindés supplémentaires. Le projet de loi de finances pour 2018 places le soldat et sa famille en son coeur la condition de vie des militaires et leurs familles et une de mes priorités absolues s'est présenté il y a un mois un plan famille ambitieux concret qui va permettre, dès 2018, d'améliorer le quotidien de nos forces et de leur famille. Ce plan comporte des mesures pour mieux vivre la mobilité pour améliorer le logement des familles et l'hébergement des soldats ou encore pour faciliter l'intégration des familles au sein de la communauté militaire. Et ce plan est dotée de moyens financiers conséquents : 300 millions d'euros sur 5 ans et 22 millions d'euros supplémentaires déjà inclus dans ce projet de loi de finances pour améliorer le quotidien de nos forces, ce projet doit immense 2018 répond donc aux attentes du quotidien de nos armées. Mais ils permettent aussi de préparer leur avenir. D'abord, il prévoit des moyens supplémentaires extrêmement conséquent pour les équipements, les équipements de nos armées sont fortement éprouvée, parfois vieillissants Jean disait un mot il y a quelques instants, nous devons donc les renouveler, c'est une condition essentielle pour garder notre supériorité opérationnel et pouvoir continuer à intervenir partout où les intérêts de la France seront menacés. Le budget 2018 prévoit donc de porter à 18 milliards et demi les crédits d'équipement, soit une augmentation de 1 milliard 200 Un effort particulier sera également menée en faveur des dépenses d'infrastructures, elles ont trop longtemps été les variables d'ajustement des Budgets de la défense, c'est fini. Or, dissuasion et hors fonctionnement. Le projet de loi de finances pour 2018 porte à un milliard et demi les dépenses d'infrastructures, ce qui représente une augmentation de 25 pourcent par rapport à 2017. Ce projet de budget permet également de prendre en compte mon engagement pour l'innovation. Je place en effet l'innovation au centre de mon action, c'est le seul moyen que nous avons de répondre à des ennemis mieux armées, mieux équipées. C'est aussi le seul moyen de répondre à des menaces plus diffuses plus technologique. Je crois dans l'innovation et le budget 2018 consacrera donc 720 millions d'euros aux études dans un effort de R&D global, portée à 4 milliards 700 c'est un point départ et la loi de programmation militaire futur que nous discuterons au 1er trimestre 2018 prévoira une augmentation rapide et conséquente des Budgets, des études et du soutien à l'innovation. Le projet de budget 2018 nous lit pas. Certaines de nos priorités. Je pense notamment aux renseignements et à la cyberdéfense les moyens que nous y consacrons sont consolidés et nous connaîtrons de nouvelles augmentations d'effectifs dans ces domaines. J'aimerais conclure cette présentation générale, en ajoutant que ce budget est une étape. Chaque année jusqu'en 2020, 2 le budget de la défense va croître de 1 milliard 700 millions d'euros supplémentaires et nous gardons donc bien le cap vers l'objectif fixé par le président de la République consacrer 2 pourcent du PIB à la Défense en 2025. Cette présentation générale j'ai répond : je l'espère un certain nombres des questions que vous avez pu soulever lors de vos interventions j'aimerais néanmoins revenir sur quelques points que vous avez souligné le 1er d'entre eux portent sur la fin de gestion 2017, j'entends tout à fait vos interrogations. Je vois même que cette question pour serait certains à ne pas voter une hausse d'1 milliard 800 millions d'euros du budget de notre défense. Vous connaissez tous, l'enjeu de cette fin de gestion pour le ministère des Armées, il était doux. D'abord, il s'agissait de couvrir le surcoût des OPEX et démission intérieures. C'est chose faite, puisque j'ai obtenu un arbitrage favorable pour une couverture intégrale de ces surcoûts sans annulation sur le budget des armées dans le cas de projets de décret d'avance et de loi de finances rectificative de fin d'année. Ensuite, et c'est évidemment le point central, que vous avez souligné à plusieurs reprises, il s'agit d'obtenir le dégel de 700 millions d'euros de crédits qui ont été rendus indisponibles sur le programme, équipement des forces de la mission défense. Sur ce second point, les arbitrages sont en cours. Si vous me le voulait bien me laisser terminer. Comme certains d'entre vous ont la la gentillesse de le rappeler, je n'ai jamais rien lâcher sur le budget des armées et ce n'est donc pas aujourd'hui que je vais commencer. Mais vous comprenez que dans cette période de négociations, je ne suis pas encore en mesure de vous dire tout. Je peux néanmoins vous dire certaines choses. Ce que je peux vous dire. C'est que ces crédits n'ont pas fait l'objet d'une décision d'annulation dans le cadre de la fin du schéma de fin de gestion. C'est déjà une première. Sans préjuger du reste je constate donc que cela laisse ouverte l'hypothèse d'un arbitrage favorable pour le dégel de ces 700 millions d'euros de crédits qui sont, je vous la accord nécessaires au financement de l'équipement de nos forces et à la maîtrise du niveau de notre reports de charges en entrée de gestion 2018. Il s'agit évidemment d'un élément très important pour notre défense, mais aussi pour la prochaine loi de programmation militaire. Je peux donc vous dire que je reste totalement déterminé à obtenir le dégel de ces 700 millions d'euros de crédit. Un autre élément est revenu dans certaines de vos interventions qui concernent l'annulation de 850 millions d'euros de crédit intervenue en juillet 2017, je n'y reviendrai pas, je crois que tout a été dit sur notre détermination. Faire en sorte que ces annulations ne porte pas sur la substance même de ce budget. Je voudrais maintenant répondre à quelques points qui ont été abordés par les uns ou les autres, tout d'abord, Monsieur le Sénateur, Guerriau, vous avez exprimé votre attente en faveur des coûts, la condition de vie des militaires, les femmes et les hommes de la Défense, ainsi que leurs familles font preuve d'un courage et d'un engagement exemplaire qui sont au coeur de mon action et j'ai déjà détaillé telle tout à l'heure, quelques unes des mesures du plan famille vous avez également interpellé à propos de la directive temps de travail. Une transposition. De cette directive fragiliserait le statut militaire et son n'obligation de disponibilité le temps d'activité des militaires ne saurait en effet reposait sur une logique purement comptable. On n'est pas militaire quelques heures par jour, on l'est 24 heures sur 24 : la gestion de ce temps d'activité doit donc laisser dans un cadre réglementaire adapté une marge d'appréciation au commandement responsable à la fois de la condition du personnel et de la bonne exécution des missions. J'ai donc demandé au service d'expertiser les options possibles et qu'une étude approfondie me soient fournis afin d'en mesurer les impacts en tenant compte du retour d'expérience des pays européens qui l'ont mis en oeuvre, notamment l'Allemagne. Madame la sénatrice, vous avez vous aussi exprimer votre attention pour les conditions de vie de nos militaires mais vous avez également exprimé une interrogation au fond sur le bien-fondé de notre dissuasion. Je voudrais, pour ma part, réaffirmer mon plein soutien con, conformément d'ailleurs au au souhait du président de la République ou budget qui sera consacrée dans les prochaines années au renouvellement des 2 composantes de notre dissuasion nucléaire car c'est notre dissuasion qui permet de préserver notre liberté d'action et de décision en toute circonstance c'est aussi elle qui permet au président de la République d'écarter toutes formes de menaces de chantage qui viserait à nous paralyser, c'est donc une dissuasion défensive qui a pour but de préserver la capacité de notre nation à vivre, c'est-à-dire de protéger notre pays de toute agression d'origine étatique contre ses intérêts vitaux et nous aurons naturellement l'occasion d'y revenir, dans le cadre du débat sur la loi de proches programmation militaire, vous avez également madame la sénatrice attiré mon attention sur la réforme du service de santé des armées. Ce service de santé s'est engagé dans une démarche de transformation qui prévoit notamment une meilleure insertion de ces établissements dans le Tir dans les territoires de santé et permet de garantir un niveau d'activité permettant au personnel du service de santé des armées d'atteindre un niveau de performance technique optimales. De nombreuses mesures ont été prises pour 2018, à commencer par le dépôt à la fin du déploiement des 16 centres médicaux des armées, nouvelle génération, ainsi que l'amélioration de la performance et la consolidation des partenariats, des hôpitaux d'instruction des armées le sache. L'institut de recherche biomédicale aura pour objectif d'achever la mise en service de c'est la barre à Thouars, qui sont confinés NRBC et l'école du personnel Marks paramédical armées de Toulon, ainsi que l'école de santé des armées de Lyon qui seront regroupés sur le site dans enfin nous allons mettre en place une nouvelle gouvernance du SSA pour assurer une plus grande cohérence à sa tête, tous ces éléments et, évidemment, ne remettant pas en cause les appréciations que vous avez pu porter sur les difficultés que que collectivement, le service de santé des armées a pu éprouver face à une évolution qui a été rapide, voire même très rapide qui lui a été demandé, et je partage évidemment tout à fait votre préoccupation car c'est un service qui est atteint, Suliman essentiel au bon fonctionnement des armées. Je voudrais maintenant Monsieur le sénateur Alizart revenir sur les questions que vous avez soulevés, d'abord pour vous remercier d'avoir. Insisté sur l'importance de l'innovation, de la recherche et les moyens qui sont consacrés je suis très heureuse de vous en emmènera en parler car comme je vous le disais, c'est un thème que je porte tout particulièrement aujourd'hui le ministère des Armées Sangla j'pleinement pour l'innovation et je crois que chacun a maintenant pris la mesure des enjeux qui se cachait derrière, vous avez particulièrement attiré mon attention sur l'onéreux. Vous l'avez dit, dans une situation financière fragile, il doit donc se réformer pour dégager les ressources nécessaires pour afin de mener ses activités d'établissements de recherche et d'opérateurs de grands moyens techniques. Dans une logique de complémentarité avec les industriels du secteur, conformément au contrat d'objectifs et de performance 2017, 2021, qui a été signé à la fin de l'année dernière. Je suis ce dossier avec beaucoup d'attention et plusieurs orientations doivent être prises, conformément au contrat d'objectifs et de performance, je pense notamment à une réorganisation des implantations Delaunay rend, en particulier en Île-de-France avec le passage de 3 sites à un site centré sur Palaiseau à l'horizon 2020, 2 ou bien à une meilleure valorisation des résultats de la recherche de l'office, avec pour but une augmentation significative des recettes de ses Vous avez également attiré mon attention sur l'importance stratégique de la base de Djibouti en effet cette base est une base majeure dans une zone qui est marquée par le conflit au Yémen en Somalie où la France et ses armes compte bien rester implanté dans la durée, nous dit disposant de plus de 1450 personnes une base aérienne un régiment, une base navale, nous garderons nos positions sur place, en étroite coopération avec le gouvernement djiboutien. De là, nous continuerons à former les armées africaines qui sont impliqués dans la sécurité de la zone somalienne, nous continuerons à contribuer, avec nos partenaires européens à la sécurité des Detroit, tout en restant vigilant face à l'implantation récente que vous avez rappelé de l'armée chinoise sur place une implantation très conséquente Djibouti continuera donc et j'y veillerai dans la prochaine loi de programmation militaire, être une base essentielle dans notre dispositif des forces de présence, monsieur Bouton, merci d'avoir salué l'effort de renforcement des effectifs initié dans le cadre de la loi de programmation actualisée en faveur des services de renseignement vous avez attiré mon attention sur la DRS D, dont les missions ont été fortement accru au cours des années précédentes, ce qui a rendu parfois l'exercice de ces missions difficiles notamment dans l'exercice d'un d'un certain nombres de contrôles ainsi que sur la situation de ces infrastructures, alors j'ai pu moi-même prendre la mesure des choses, et me rendre compte de la transformation profonde à laquelle sa direction, c'est plié, une transformation qui mérite d'être pleinement soutenu dans ses efforts par une remontée en puissance de ses effectifs, et c'est ce qui est prévu, notamment dans le cadre de ce projet de loi de finances. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, j'espère avoir répondu non pas à toutes vos interrogations, mais à un certain nombre d'entre elles, et je crois très sincèrement que le budget pour nos armées pour cette année 2018 qui commence est une opportunité. Une opportunité rare pour nos armées pour notre défense et pour notre sécurité.

C'est la réponse qui est attendue par nos concitoyens face aux menaces qui pèsent sur la France et qui ont été parfaitement identifiés dans la revue stratégique de défense et de sécurité nationale, ce projet de loi de finances enfin constitue une base saine pour le prochain grand exercice que nous mènerons ensemble, c'est-à-dire la construction de la loi de programmation militaire, ce sera l'occasion de dessiner la défense de demain une défense que je veux plus forte, plus innovante, plus européenne et je sais que je pourrai compter sur vous, sur votre bonne volonté et sur votre détermination, je vous remercie. Merci madame la ministre. Nous allons à présent procéder à l'examen des amendements portant sur des crédits de la mission défense figurant à l'État de.

Merci Monsieur le Président, madame la ministre, chers collègues, hé bien écoutez votre intervention madame la ministre, mais fait revoir un peu tout ce que j'avais prévu dans dans cet amendement, je ne vais pas rappeler ce que j'ai dit dans dans l'attente, intervention générale, ce n'est pas la peine, bon je continue de d'exprimer quand même que avant-nous réellement besoin de produire autant d'armes de destruction massive, je pense que, avec vous, Madame la Ministre, le président de la Commission, nous pourrions avoir des des moments de de réflexion sur de de tels sujets quand on, quand on le peut, mais il faut aussi penser à cela, il faut aussi penser à cela pour l'avenir, pour sortir du nucléaire, c'est un point qui me qui nous tient à coeur, a beaucoup aussi d'entre nous, mais on n'a pas toujours les solutions comme je voulais préciser aussi, comme l'a montré dans ce rapport, notre collègue Dominique linge la situation immobilière de l'armée vous est très préoccupé plante mais mais mais vous nous avez là encore donner des réponses claires,

à reprendre, formé à être habitable would par nos armées mais je pense aussi à la promesse du président pour un futur retour du service national au service national universel, je voulais simplement vous dire que, vu le contexte déjà que de notre armée a actuellement de nos soldats, je pense que enfin personnellement un personnellement, ça ne semble pas envisageable

Merci, cher collègue, nous passons donc à l'amendement 174 que vous défendez également chers collègues. Alors un peu le même contexte, mais j'en reviens toujours sur notre idée sur le temps, je vous ai parlé de cela aussi dans l'intervention général par rapport à notre souveraineté par rapport aussi au droit de la charte des Nations ne sait ni qui avait été que

qui continue et partout où le temps se renforce la notamment, même avec les après la guerre froide avec le la séparation au niveau de différents États de de l'Union soviétique, en fait, la l'armement, la course à aux armements a elle aussi progressé, cite, c'est quelque chose de systématique comme vous le voyez, mais chacun, à chaque fois que qu'on développe l'offre au lieu de promouvoir la paix, parce qu'en fait, lorsque l'on parle de l'armée, on parle de guerre, mais où on doit aussi savoir faire la paix et gérer la paix, donc voilà, là, c'est aussi pour rediscuter de la participation de la France à l'Otan, je sais parfaitement que ça ne peut pas mais ce sont des réflexions qu'il faut que nous prenions le temps d'avoir parce que il y a d'autres possibilités, peut-être pour gérer ou du moins anticiper sur la note, réalisation de de ces conflits aussi où on on n'en parle pas beaucoup, voilà

Monsieur le Président, c'est un moment, vise à diminuer les crédits consacrés à la participation de la France à l'Otan 243 millions madame pruneaux, la France est un membre fondateur de l'Otan, et je crois que plus que jamais, nous ne pouvons pas être isolée et par conséquent, c'est un avis défavorable. Merci Monsieur le le rapporteur, quel est l'avis du gouvernement. gouvernement. Président Madame la sénatrice, je comprends que cet amendement d'appel, néanmoins je j'ai le même avis que la Commission défavorable. Merci madame la ministre, vous le maintenez. je le retire également. je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite je donc on voit les crédits de la mission. Des Qui est contre qui s'abstient, Des crédits sont adoptés. J'appelle en discussion des articles 52 7ème 52 obtient qui sont rattachés pour leur examen au crédits de la mission défense.

Merci Monsieur le Président, le président de la République, donc, s'est engagé à la mise en place au cours de son quinquennat d'un service national universel comme chacun sait, qui devrait être expérimenté en 2019, 2019, c'est demain, nous aurons bientôt en rediscuter donc dans un rapport de juin 2017, le Sénat avait le 1er chiffré le coût du rétablissement pur et simple service national entre 15 et 35 milliards d'euros sur le quinquennat et c'est, j'ai pas de cette, de ce rétablissement dans son comme il fut dans le passé, mais pour autant, ce rapport a heureusement contribuer à réorienter la réflexion vers des dispositifs plus réaliste, mais dont le financement demeurent floues, combien ce futur dispositif va nous qu'il nous coûter le financement sera-t-il interministérielle si oui dans quelle proportion, un grand nombre de questions, comme vous le constatez, peuvent se poser mais qui devrait être éclaircies avant le débat d'orientation des finances publiques de l'année prochaine, eu égard aux difficultés budgétaires au choix que nous devons faire, on le voit bien aujourd'hui puisque la satisfaction d'une augmentation du budget réel, mais pour autant, à Sainte-Anne nous interroge quant à l'ensemble des domaines qu'il faut traiter ce calendrier devrait en outre correspondre rendu travaux de la commission SNU, qui pourra ainsi contribuer à la rédaction du rapport demandé par le présent amendement, voilà l'objet de notre attente, un rapport d'information merci Monsieur le Président. Merci, cher collègue, quel est l'avis de la commission. L'avis de la commission, c'est que lorsque le le ministre est venue devant la commission des finances, la question lui a été posée, nous a indiqué que le secrétaire d'État travaille actuellement sur cet engagement, cette proposition du président de la République, vous nous dites un rapport dont 6 mois je sais pas où on en sera dans dans 6 mois et je ne doute pas un seul instant que le ministre associera les parlementaires et avant de remettre un rapport, ce serait peut-être bien que nous ayons une discussion et, donc, dans, dans ces conditions, chers collègues, ce que je vous propose, c'est de retirer votre amendement ou sinon ce serait hélas un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, qui de l'avis du gouvernement. Le président, monsieur le sénateur. Pour des raisons similaires, je ne suis pas favorable à cet amendement en effet le 1er ministre a confié à différents corps d'inspection, le soin de recenser les de recenser les dispositifs existants, les formations à la citoyenneté, les Budgets qui sont mises en oeuvre, bref de rassembler tous les éléments qui sont nécessaires à la décision afin de mettre en oeuvre cet engagement du président de la République de créer un service national pour promouvoir la citoyenneté et une culture de l'engagement ce rapport demandé au corps d'inspection sera prochainement remis au 1er ministre par ailleurs des missions d'information ont été initiés par chacune des 2 assemblées, le gouvernement associera naturellement les parlementaires à ces réflexions, une fois ce rapport rendu donc dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire pour la bonne information du Parlement de poser ce principe par voie d'amendements parce que cette concertation, elle aura évidemment lieu. Merci, Madame la Ministre Monsieur Grillot. Monsieur le président, nous aurons à coeur de nous impliquer dans ses missions d'information, et donc nous serons très attentifs et très présent et constructif dans cette, dans cette démarche et à ce titre donc je retire notre amendement.

Qui est contre qui s'abstient, il est adopté. Ordre du jour du vendredi 1er décembre 2017. 30 nouvelle lecture du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 à 15 heures et éventuellement le soir : suite du projet de loi de finances pour 2018 : examen de la mission écologie, développement et mobilité durable, la séance est levée.